La séance est ouverte le compte-rendu de la séance du jeudi 27 janvier a été publié sur le site internet du Sénat s'il n'y a pas d'observation, nous considérons le procès-verbal comme adopté j'informe également que le Sénat, que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à démocratiser le sport à améliorer la gouvernance des fédérations sportives et à sécuriser les conditions d'exercice du sport professionnel n'est pas parvenu à l'adoption d'un texte commun. L'ordre du jour appelle le débat sur les menaces que les théories du wokisme font peser sur l'université, l'enseignement supérieur et les libertés académiques demande du groupe, les républicains. Je vous rappelle que dans ce débat, le groupe LR disposera notamment de présentation de 8 minutes, le gouvernement a la faculté s'il le juge nécessaire de prendre la parole immédiatement après chaque orateur pour une durée de 2 minutes l'orateur disposera alors à son tour du droit d'répartis pour une minute, le temps de réponse du gouvernement à l'issue du débat est limitée à 5 minutes le groupe, auteur de la demande de débat du sport 5 minutes pour le conclure madame la ministre, vous pourrez donc, si vous le souhaitez répondre après chaque orateur, une fois que celui sur à retrouver une place dans l'hémicycle, la parole est tout d'abord à l'orateur du groupe, qui a demandé Monsieur Max Brisson pour le groupe Les Républicains pour 8 minutes. Madame la présidente, Madame le Ministre, mes chers collègues, j'ai d'abord à remercier le président Retailleau et le groupe, les républicains d'avoir ce qui se débat à notre ordre du jour, tant sont grandes les menaces que les théories du wokisme pour peser sur l'université, l'enseignement supérieur et les libertés académiques, comme vous le savez, mes chers collègues, la traduction littérale de stewards signifie rester éveillé popularisé aux États-Unis, à l'origine dans la communauté afro-américaine la notion est devenue récemment un projet politique d'ampleur, notamment à travers le mouvement Black lives Matter caractérisée par le scepticisme radical quant à la possibilité d'obtenir une connaissance ou une vérité objective l'eau qu'ils on perçoit le monde sous une vision manichéenne le partager entre oppresseur et oppressée dominants et dominés, cette idéologie ni en Amérique a depuis traversé l'Atlantique, de l'écriture inclusive au relativisme culturel de la déconstruction communautarisme de la culpabilisation à la victimisation, l'eau qui n'est devenu la bannière sous laquelle ces militants de fragmenter l'unité républicaine, en définissant la citoyenneté sur une identité fondée sur l'origine, la race, la sexualité ou le genre, je ne peux quant à moi, vous résoudre et qu'en France, pays des lumières, des droits de l'homme et de Victor Hugo, on puisse faire sienne une conception si différente de la citoyenneté que celles qui nous rassemble, depuis la Révolution française, je préfère celle que portait Ernest Renan, lorsqu'il écrivait en 1882 l'homme n'est esclave ni de sa race, ni de sa langue, ni de sa religion, ni du cours des fleuves, ni de la direction des chaînes de montagnes, il ne grande agrégation d'hommes saine d'esprit et chaude de coeur qu'il ait une conscience morale qui s'appelle une nation Renault affirmé ainsi ce qui fait le coeur même d'autres citoyenneté l'adhésion de chaque citoyen aux valeurs de la République sans un effacer pour autant l'identité personnelle cette conception française de la nation fondée sur une course constitué d'individus qui partagent une communauté d'idées d'intérêt d'affection, de souvenirs et d'espérance est au fondement de notre République, c'est pourquoi je crois que l'eau qui pourtant lui une radicalité qui heurte directement notre conception de la nation et en conséquence les principes constitutifs de notre République et c'est justement parce qu'il est porté atteinte au coeur de la République qu'elle se doit de réagir fermement aux attaques qui lui sont faites, comment des fruits ne pas réagir lorsque le communautarisme sous couvert de discours racialiste et indigéniste et invite à la repentance perpétuelle et à déboulonner les statues de nos personnages historiques les plus illustres, comment ne pas réagir face à des municipalités qui autorise l'organisation de manifestations non mixtes sur la voie publique, comment ne pas réagir lorsque le recours à l'écriture inclusive se vulgarise dans la segments supérieurs alors même qu'une circulaire indique aux administrations de ne pas en faire usage, lorsqu'université publique accueille dans ses locaux un colloque sur la déconstruction déstabilisant le caractère un et indivisible de notre République, comment ne pas réagir lorsque des visions idéologiques tente de soumettre l'enseignement de l'histoire au prisme d'une vision globale, entre-temps, les lunettes déformantes du présent pour la soumettre aux exigences présupposé de notre époque : comment ne pas réagir lorsqu'un professeur subit : harcèlement, pressions et menaces pour avoir contesté la réalité scientifique du concept d'islamophobie, suis profondément mal à l'aise d'observer la diffusion de l'idéologie ou gauchiste à l'université et dans l'enseignement supérieur et les procédés mis en oeuvre pour censurer les professeurs qui nous sert, ce qui ne veut pas dans ce courant de pensée, oui, je crois que dans d'autres pays, nos universités font rectrice d'un projet d'émancipation et doivent cultiver chez nos étudiants, une ouverture d'esprit nourri par la conscience de la pluralité des modes d'établissement de la vérité, oui, je suis convaincu que laisser cette idéologie nauséabonde prônant la dissolution de toutes normes se diffuser, c'est porter atteinte à l'essence même d'autres démocraties qui vit par le débat et la confrontation d'idées et non pas la censure et le relativisme et que l'université par excellence le lieu où il faut protéger le débat, la confrontation pacifique et régulée des idées afin que progresse la connaissance et que s'établisse la vérité scientifique pourtant mes chers collègues, si l'eau qui tient parfois le haut du pavé, force est de constater que cette idéologie ne portent les revendications quand une petite minorité d'individus comme le montre un sondage IFOP, de février 2021 plus de 86 % des Français disent ne jamais en avoir entendu parler et parmi les 14 % restants 8 % affirment ne pas savoir de quoi il s'agit finalement ces chiffres font apparaître le wokisme pour ce qu'il est un Opium des intellectuels comme l'écrit Pierre de lenteur qui ne se diffuse Cosset de minorités restreinte, appuyés par des théories américaines qui ne sont aucunement adapté, ni adaptable à la réalité de la France, il est donc grand temps de rappeler combien la réalité objective, dessiné par le travail des historiens, des chercheurs et des professeurs fait rarement bon ménage avec la réécriture historique aux fins de desiderata politicien, il est donc grand temps de combattre une idéologie qui tourne le dos à l'idéal des Lumières à l'apport de la Révolution française et au fondement même notre conception républicaine, permettez-moi de trouver Madame la Ministre, la nature de ce gouvernement, Bienne en demi-teinte, certes quelques déclarations ont pu donner l'impression de l'action, mais force est de constater que la prégnance et ces formes d'action les plus violentes ont progressé en 5 ans, comme si la fascination du président pour le modèle anglo-saxon, constituer un frein, un combat résolu contre une idéologie de la déconstruction qui peut malheureusement trouvé un écho dans certains propos présidentiels pour combattre le wokisme, il faut regarder notre passé, certes avec clairvoyance mais certainement pas avec suspicion et esprit de repentance, or c'est sur cette voie que hélas plusieurs fois le président Macron a voulu nous entraîner pour combattre le wokisme il faut réarmer intellectuellement nos professeurs pour qu'ils soient les garants de notre conception universelle de la citoyenneté, celle qui n'a assignent jamais un citoyen d'notre République à sa couleur de peau à ses croyances et à ses pour combattre le il faut mettre au centre le projet éducatif, l'apprentissage des savoirs fondamentaux pour combattre le wokisme il faut replacer, comme Pierre angulaire de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'ouverture d'esprit et le débat d'idées pour combattre l'eau qui, il faut tout simplement réassurer notre conception de la citoyenneté, mes chers collègues, la nation nous rassemble la République nous fédère une autre citoyenneté nous ouvre au monde ces concepts trompé au coeur de notre histoire demeurent d'une étonnante modernité, nous devons avoir ensemble, envie de les partager, j'espère sincèrement que le débat qui s'ouvrent, au-delà de la dénonciation des dérives fera l'occasion d'une vraie réflexion justement sur la modernité de notre conception de la République et sur les moyens que nous devons mobiliser pour la protéger et l'affaire prospérer la en particulier où se forme la capacité d'analyse critique des jeunes Français, là où le débat doit toujours être pluraliste, curieux, ouvert, car il est le garant du de connaissance scientifiques avéré, c'est-à-dire aux Serbes, même de notre université, je vous remercie. Madame la ministre, vous souhaitez vous exprimer maintenant mais je vous en prie. Merci madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Brisson. L'héritage des Lumières, c'est évidemment de regarder chaque citoyen, chaque individu de notre nation, comme il l'est par ses actes et vous avez rappelé aujourd'hui monsieur le sénateur, l'importance de la nation, ce qui nous amène à débattre aujourd'hui, ce sont les conséquences, les menaces que porte le wokisme c'est une idéologie politique qui vient des États-Unis, et vous l'avez rappelé. Notre enjeu le projet du président de la République, c'est un projet émancipateur, c'est un projet qui a qui aiguise l'esprit critique l'héritage des Lumières, celui qui garantit le pluralisme au sein de nos universités le pluralisme de la recherche, le pluralisme des enseignements et le plus important encore, Monsieur le Sénateur, c'est de permettre que chacun de ces étudiants en réalité débattent se construisent et là où nous luttons et sur quoi nous luttons cette garantir qu'il ne s'installe pas une idéologie plus qui qui imposerait finalement le débat au sein, évidemment, de nos universités, c'est évidemment de lutter pour ce pluralisme et défendent cette liberté académique cette liberté d'enseignement dont nous avons hérité depuis la IIIe République, c'est de permettre que on ne ne tombe pas dans cette facilité, finalement, de ne plus étudier un auteur d'aller revoir l'histoire qu'avec des lunettes d'aujourd'hui c'est effectivement revenir sur cette liberté académique absolument essentiel, monsieur le sénateur, nous avons un enjeu avoir des jeunes, des citoyens éclairés prêt au débat. Armer idéologiquement outillé historiquement et qui ne font qu'une chose qui fonde leur espérance dans la force d'une nation qui luttent en réalité contre les discriminations qui luttent contre les actes racistes, homophobes antisémites et qu'il n'est censé lisent pas les débats, c'est le projet universaliste du président de la République et c'est pour cette pluralité, merci les

je vous arrête sur votre chemin, c'est tout, c'est pas ce pouvoir et les autres s'il en avait, je n'en n'userait pas. Madame la Ministre je crois à la sincérité de votre combat personnel et vous l'avez souvent montré, permettez-moi, en revanche, de douter en la matière, de la volonté constante du président de la République et du et du gouvernement, lorsque le président de la République nous invitent constamment à la repentance lorsque dans ses aptitudes, en particulier par rapport à notre passé à la guerre d'Algérie, il invite à des réconciliations avec qui nous une partie en face qui n'a jamais eu l'intention d'être à la réconciliation, je crains qu'il ne soit pas autant à la hauteur de cette volonté farouche que vous avez exprimées en revanche, je veux bien reconnaître et vous l'avez fait à Poitiers, en particulier, votre courage dans des moments difficiles lorsque le wokisme empêchée par la censure, l'expression de la vérité, je doute profondément que le chef de l'État soient constamment sur cette position, le en même temps oblige à voir très large et malheureusement quand le en même temps bon aussi de temps en temps, pêcher du côté des gros kyste. Merci madame Benbassa c'est à vous. Nous, on ne on c'est une procédure de débat un tout petit peu nouvelle, donc, le temps que je m'adapte. madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la principale difficulté à laquelle nous devons nous confronter et celle de la définition du wokisme je connais certes celle établie par ses détracteurs, il ne serait pour eux qu'un agrégat des idées défendues par une certaine gauche animé par la volonté de démanteler notre culture et notre société. Cette vision for caricatural ne permet pas de saisir tous les enjeux de ce concept qui ne se limite pas opposés aux propositions extrêmes et peu constructive des promoteurs de la classe, caoutchouc, de la culture de l'annulation, l'origine du wokisme remonte aux années 1960 lorsque Martin Luther King, appelé lors du mouvement des droits civiques, la jeune génération noir à rester éveillé et à être une génération engagée popularisé dans les universités américains à partir des années 2000, période à laquelle, je les ai personnellement souvent le concept de Brock est en réalité très vaste, il intègre le boycott le déboulonnage des statues le des colonialismes l'antiracisme les appels à lutter contre la misogynie et le sexisme, la dénonciation auxquelles sont assimile le lynchage médiatique, ainsi que sur les réseaux. Je conçois que certaines actions et prises de position puisse interroger les unes relevant du militantisme politique et de la liberté d'expression et d'autre d'une volonté d'instaurer une pensée unique, tout comme je dénonce celles et ceux qui caricaturent ce mouvement, je dénonce des militants Walk, qui parfois par des pratiques inappropriées poussent à l'autocensure, laquelle doit rester étrangère au monde de la recherche et de l'enseignement supérieur, la richesse du monde universitaire, tient à la place qu'il accorde à la confrontation intellectuelle tenter de réduire au silence, celles et ceux qui ne partagent pas nos idées est inacceptable mon constat est donc le suivant : la liberté académique doit être préservé à la fois des pressions gouvernementales visant à encourager la recherche un enseignement officiel mais aussi de l'extrémisme susceptibles de donc découlait de certains partis pris idéologiques, comment envisagez-vous de garantir la préservation de cette liberté académique qui me semble d'un côté comme de l'autre menacé aujourd'hui, on a bien longtemps enseigné la French Theory Derrida, Foucault ont enseigné eux-mêmes et notre enseignement n'a pas été touché, n'a pas été dévalorisé au contraire nous avons. Ex-exporter nos idées et nos concepts dans d'autres pays, merci.

Vous souhaitez la parole n'administre. Merci madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Benbassa. Un des héritages les plus précieux que nous avons au sein de nos universités, c'est la liberté académique, c'est la pluralité de la recherche et tout l'enjeu, tout le travail de ce gouvernement et cette équipe gouvernementale et ça a été de poser des actes, ça a été par exemple le le grand combat de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui pose avec la loi de programmation de la recherche, plus de 25 milliards d'euros d'investis pour garantir garantir et stimuler cette pluralité, notre objectif, notre enjeu, c'est de garantir un climat serein au sein de misère de nos universités de simplement pas laisser s'installer une pensée autorisée pas une autre, et finalement finalement l'esprit critique de nos étudiants et ne pas laisser non plus s'installer ce que nous avons pu voir ces dernières ces ces derniers mois et ces dernières années, parfois des colloques chahuté parfois des enseignants pris à partie, quelle que soit en réalité la théorie ou leurs recherches où les sujets de leurs recherches, c'est la grandeur de la France que de permettre à des débats sans serein étayé et en en réalité qui pousse à l'esprit critique et pour cela, pas de nom placardé au sein de l'université, pas de colloques interdit, bien au contraire. L'esprit français, c'est l'esprit critique, c'est l'esprit des Lumières. : je m'y retrouve plus écoutez, Madame la Ministre, c'est ce que j'ai voulu dire mais enfin il ne faut pas faire à faire une obsession du fait qu'on puisse enseigner le racisme, l'antiracisme le féminisme à le néo-féminisme dans les universités, vous savez bien qu'il y a très peu de postes pour tous ces nouveaux nouvelles matières et au CNRS la même chose, ce n'est pas un danger après le le le l'islamo-gauchisme, maintenant c'est le wokisme non, mais l'université vous savez est un endroit encore où la pensée résiste et il est bon de préserver cette pensée critique comme vous l'avez dit vous-même, merci. Monsieur, il y a une centrale, vous avez la parole pour 9 minutes pour le groupe socialiste, écologiste et républicain.

nous ne sommes pas du. Nous ne sommes pas dupes de la manoeuvre opérée aujourd'hui par le groupe, les républicains en pleine élection présidentielle, vous avez décidé d'utiliser le Sénat afin d'avancer votre agenda démagogique en nous invitant à ce que Élisabeth Roudinesco appelle un banquet totémique, on pourrait même parler de séances d'exorcisme, nous sommes en quelque sorte invité aujourd'hui à conjurer le mal de ce point de vue, la droite conservatrice au sein de cet hémicycle emboîte le pas à la droite autoritaire au gouvernement hier le mal que combattaient les forces réactionnaires qui mine notre pays, c'était l'islamo-gauchisme, aujourd'hui c'est le wokisme et demain, ce sera encore un autre néologisme, vous êtes devenus maîtres dans l'art d'inventer de nouveaux mots censé couper court à tout débat et de créer autant d'écran de fumée sémantique pour ne pas parler des vrais dangers qui mine notre pays et, plus particulièrement, nos universités car ne nous y trompons pas, nos collègues de droite et leurs jumeaux au pouvoir n'ont cure de l'université de la liberté académique et de la recherche, vous n'avez jamais eu que mépris pour les chercheuses et chercheurs qui sont, qui, dans leur laboratoire, sur le terrain ou dans leur séminaire d'hypothèse en hypothèse travail le doute tente de comprendre le monde telle qui va et prépare notre avenir, encore une fois, l'université est instrumentalisée pour alimenter la machine à délire et polémique qui nourrit chaîne info et réseaux sociaux à longueur de journée, ce débat est donc un nouvel écran de fumée bien pratique pour celles et ceux qui, à droite comme au gouvernement, défendent le statu quo et son cortège de privilèges, plus grave encore, derrière ces écrans de fumée, vous cherchez surtout à ce qu'on en parle pas, à l'université ou ailleurs, des injustices et des discriminations qui frappent les jeunes lors de leur recherche d'emploi, de formation ou de logement, vous ne souhaitez pas que soient abordés les discriminations et l'injustice qu'ils subissent en raison de leur nom de leur adresse de leur accent de leur genre de leur sexualité, de leur couleur de peau ou de leur handicap, vous ne souhaitez pas que soit évoqué les violences symboliques verbales, voire physiques que constitue le sexisme et la misogynie, l'homophobie, le racisme, l'antisémitisme et la haine des musulmanes et musulmans de France, vous ne voulait surtout pas qu'on parle de tous les systèmes de domination visibles ou invisibles qui marginalise exclu oppresse et parfois tuent dans notre pays, à droite comme au gouvernement, on ne veut surtout pas parler de ces sujets, et c'est bien, a éludé toutes ces questions pourtant vital pour un grand nombre de nos compatriotes que sert l'écran de fumée du débat réactionnaire de ce jour pourtant, c'est bien cela, être républicain et universaliste, c'est vouloir l'égalité réelle des droits, une réelle justice et le respect pour tous les enfants de France, alors nous aurions pu boycotter ce débat ridicule qui nous plonge encore une fois dans les abîmes sans fond d'une campagne présidentielle qui peine à faire émerger les vrais sujets de préoccupation de nos compatriotes, mais c'est justement parce que l'université et le lieu du débat de la construction de l'esprit critique et de la contradiction que nous n'avons pas voulu leçon, laisser le Champ libre à la parole réactionnaire car et le paradoxe et il faut bien le dire, le grotesque de l'intitulé qui nous est soumis, aujourd'hui, c'est qu'il bafoue tout ce qu'il prétend défendre d'abord de quoi parle-t-on cette pseudo notion de wokisme magma conceptuel informe n'a pas le commencement d'une définition scientifique, c'est une énième chimère qu'il conviendrait de laisser sinon aux amis, aux animateurs de ses News plus largement à l'extrême droite, qui l'a popularisé utiliser leurs mots, c'est faire le lit des traditionnels procureur prompt à condamner par principe les universitaires et les universités, ensuite la forme de nos échanges qui loin de reposer sur des faits, des chiffres, des analyses étayées un rapport ou même une quelconque enquête de terrain mélange sans aucun discernement, rumeurs complotisme et autres accusations sans fondement, loin de reposer sur une analyse critique et une discussion contradictoire ce débat fait la part belle aux propos de comptoir aux vérités toutes faites et aux informations non vérifiées et pire encore, ce que ce débat bafoue et qu'il faut pourtant garantir et préserver en tant que législateur, c'est l'autonomie de la recherche et la liberté académique dans notre pays, vos interventions dans ce débat sont les lustrations même du vrai danger qu'il faut combattre, celui de l'ingérence du politique dans la recherche car, que faites-vous à droite, en coupant les subventions aux établissements d'enseignement supérieur, comme votre ami Laurent Wauquiez en région Auvergne-Rhône-Alpes ou au gouvernement, en enjoignant le CNRS de mener une enquête sur ses propres chercheurs si ce n'est une chasse aux sorcières, le nouveau maccarthysme la culture de la mise à l'aide de l'annulation que vous voulez, fustigeait ici c'est vous qui l'a pratiqué l'université, c'est le lieu où s'apprennent le doute comme la modération ainsi que la seule de nos institutions capables d'éclairer l'ensemble de la société de l'école aux médias par une connaissance scientifiquement établie, discuter et critiquer collégialement ces mots, vous les reconnaissez peut-être ce sont ceux de la ministre de la recherche, dans une tribune du 26 octobre 2020, il est loin le temps où le gouvernement défendait l'université face aux attaques dont elle est constamment victime alors puisque vous voulez parler des menaces qui pèsent sur l'université, l'enseignement supérieur et les libertés académiques hé bien parlons-en ce qui menace nos universités, aujourd'hui ce sont d'abord les idées d'Emmanuel Macron, qui propose d'augmenter les frais d'inscription, voilà une idée pernicieuse venus d'Amérique du Nord qui devraient vous offusquer à droite, autant qu'elle nous a l'arme à gauche ce serait l'assurance de voir l'enseignement supérieur, de moins en moins accessible aux classes populaires et, surtout, de condamner la jeunesse à devoir payer toute sa vie une dette accablante comme c'est le cas aux États-Unis. Ou au Royaume-Uni, ce qui menace l'université, c'est la culture du néo-management qui du ranking du re-branding s'immisce dans la gouvernance des établissements au mépris de la concertation de la collégialité et du dialogue social, voilà, des théories venus d'Amérique du Nord, qui devrait vous inquiéter à droite, autant qu'elle nous inflige à gauche ce qui menace l'université, c'est la baisse de 15 % du taux d'encadrement sur la dernière décennie alors que le nombre d'étudiantes et d'étudiants passés de un 800 1000 sur la même période, ce qui menace les universités, c'est la précarisation grandissante des contrats d'enseignants et d'enseignants chercheurs qui conduit nombre d'étudiants brillants à choisir une autre carrière, comme le prouve la chute du nombre de doctorants dans ce pays, ce qui menace l'université c'est la paupérisation grandissante des étudiantes et étudiants qui continuent à défiler, tard le soir dans des queues interminables aux guichets des banques alimentaires, ce qui menace l'université, c'est le manque de crédits récurrents alloués à la recherche au profit de l'ANR alors que de nombreux laboratoires sont d'un mauvais état ou ou manque de matériel, ce qui menace l'université, c'est le système dual de notre enseignement supérieur qui autorisent encore l'État a consacré 2 fois plus d'argent pour un étudiant en classe prépa que pour un étudiant en licence, ce qui menace l'université, enfin c'est Parcoursup et ses algorithmes dans le manque de transparence nourrit l'anxiété et le sentiment d'arbitraire chez les lycéens et leurs parents, voilà les vrais sujets que nous devrions débattre aujourd'hui

c'est un fondement intangible et nécessaire dans une démocratie et nous serons toujours au côté de la communauté scientifique pour le défendre. Madame la ministre dès que monsieur. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, chanterelles. Dans vos propos, 0 nuance ce qui menace l'université aujourd'hui c'est évidemment des propos sans nuance, ce qu'on apprend à l'université, c'est l'esprit critique Monsieur le Sénateur des précarités, nous luttons contre 5 milliards d'euros depuis le début de ce quinquennat pour l'université, la précarité, les précarités, elles sont multiples : quel est le gouvernement aujourd'hui qui qui qui va lutter contre les inégalités de destin, c'est le nôtre, monsieur le sénateur, qui accompagne la précarité menstruelle des étudiantes qui gèle aujourd'hui les loyers des Cruz qui a rénové les cross c'est nous, monsieur le sénateur, alors moi je veux bien avoir un débat, je veux bien avoir un débat sur les précarités et le bilan de l'accompagnement des étudiants parce que nous n'avons pas à rougir, par contre, Monsieur le Sénateur, en respectant cette cette cette autre chambre et respectant le sujet du débat aujourd'hui hé bien contre le wokisme puisque c'est le sujet qui nous anime, hé bien nous avons saisi le collège des déontologue nous renforçons les déontologue sur les territoires avec leur référent parce que oui, notre objectif, c'est de protéger ses libertés académiques et de ne pas laisser s'installer une pensée qui serait en réalité autorisé et pas une autre, et pour ça, monsieur le sénateur, nous avons 2 enjeux : le 1er c'est évidemment garantir le climat et l'environnement, nos universités pour que les étudiants oui étudie en bonne santé étudie dans de bonnes conditions, dans des logements dignes avec des enseignants qui sont protégés et qui n'ont pas peur qu'on les lynche ou encore qu'on les mette au pilori, monsieur le sénateur, les étudiants de notre pays, aujourd'hui ils ont envie d'une université qui rayonnent universités qui fait de la recherche et c'est ce que nous faisons en recrutant au sein du CNRS, c'est ce que nous faisons en renforçant réalité parcoursup pour ne pas laisser la place au hasard, parce que c'est cela Monsieur le Sénateur, la réalité c'est que il y a à peine quelques années le choix c'était le hasard qui le décider, hé bien ce n'est pas la promesse républicaine qui est la nôtre. La parole est à Monsieur André Gattolin pour 6 minutes à monsieur Chantrel pardon. ça arrive pas. Quand même, excusez-moi, madame la secrétaire d'État, mais votre réponse me laisse pantois. à quel point votre niveau des connexions et c'est un enfant de l'université qui vous parle, je viens de la banlieue française j'ai étudié à l'université de Villetaneuse et quand je vous entends, j'ai envie de vous dire : venez avec moi les visiter,

Allez sur le terrain, quoi, allez voir les choses parce que vous ne pouvez pas voir à quel point c'est violent que des étudiants et étudiantes et des chercheurs qui nous écoutent que vous dire que tout est beau dans le meilleur des mondes avec ceux qui vivent au quotidien et eux ils le savent ce que c'est la précarité et les les conditions de recherche et les conditions de notre pays, d'ailleurs, le sénateur des Français établis hors de France, je suis pourrait témoigner de nombreux talents

nous sommes tous d'accord, la vocation du politique c'est de débattre de tout, rien de ce qui se rapporte à la vie de la cité : la police au sens grec du terme ne serait donc plus être étranger tout peut et d'une certaine manière, doit être débattu en politique, je remercie donc l'initiateur de ce débat et je me félicite précisément qu'il s'agisse d'un débat et que dans un débat malheureusement débat uniquement entre parlementaires car il eut été intéressant d'y associer des universitaires et des chercheurs sur ce domaine et qu'il ne s'agissait pas d'une proposition de loi qui aurait immédiatement posé la question très délicate de la définition des concepts et surtout de la mise en norme précise les mesures publiques qui aurait pu être avancé. Je dis ça parce que je fais partie des gens qui ont toujours été très prudent, comme nombre d'entre nous contre ce qu'on appelle les lois mémorielles quand le politique réécrit l'histoire ou choisi des doigts d'histoire plutôt que d'autres, c'est toujours un problème en matière universitaire, les choix des contenus ne relève pas de la discussion politique relève du corps, Dieu, la recherche et du monde universitaire dans son pluralisme, alors bien sûr l'intitulé du débat met en scène une notion que je connais bien, celui des libertés académiques, nous aurons sans doute l'occasion ce soir d'en débattre lors du débat organisé autour de la mission information qui traitait de ce sujet, mais le concept de liberté académique lui-même, comme cela a été développé dans la proposition de résolution européenne afin de soutenir la liberté académique en Europe que nous avons adoptée au sein de la commission des affaires européennes en décembre dernier, cette définition est ce concept de liberté académique souffre encore de l'absence d'une définition précise invariable et d'un cadre normatif unanimement admis et surtout précisément écrit et inscrit dans la loi mal nommer les choses c'est ajouter au malheur du monde, a écrit un jour : Albert Camus et en ces temps de division bien nommer les choses, doit être une hygiène démocratique, le problème de l'absence d'une définition communément admise est encore plus vif lorsque nous parlons de Walk et de wokisme, de quoi parle-t-on en faisant des recherches maire tout un chacun constater que le terme woke, vient de l'anglais, qui signifie éveillé mais qu'il ne fait l'objet d'aucune définition académique, rien à voir en tout cas avec cet ustensile de cuisine le Walk, sorte de poil Bill et eu millénaire venus d'Asie et qui ont cantonnais signifie chaudron et qui permet de cuire toutes sortes d'aliments sans mettre trop de matières grasses, encore que, encore que, en l'absence de définition académique sérieuse, ce que nous qualifions le Walk celui-ci ressemble un peu à ces mélange de légumes d'hiver de graines et de viande qu'on cuisine ensemble sans trop il y ajouter cette fois-ci de la matière grise, alors il est indispensable de distinguer 2 choses, ce qui relève du Champ scientifique et ce qui relève du débat d'idées, le Champ scientifique est un lieu structuré de production de validation et de circulation des savoirs, dans le respect de la pluralité du pluralisme, il peut et il doit exister des controverses dans le monde académique, celle-ci s'exprime selon des règles précises de débat contradictoire et argumenté la liberté académique est consubstantielle à la liberté de recherche dans tous les domaines de la science, y compris, bien évidemment, dans le domaine des sciences humaines et sociales, elle est aussi consubstantiel à la liberté d'enseigner, pour peu que cet enseignement respecte les règles, dollars, c'est-à-dire qu'il admet l'existence et l'expriment les thèses opposées à celles développée par l'enseignant ou par le chercheur, cela signifie que la liberté académique s'accompagne d'une nécessaire responsabilité académique dont le fondement d'ailleurs le plus connu et pour le chercheur, ce qu'on appelle l'intégrité scientifique et pour l'établissement universitaire, la mise en oeuvre du principe de respect du pluralisme et pluralisme et pluralité des idées et des enseignements, l'existence d'une pensée critique, c'est-à-dire d'une pensée divergente et étayée, face à la pensée majoritaire ou Dominique dominante et tout sauf enfin compatible avec une culture académique démocratique sans elle, pas de controverse de voilà, d'Ovide et des générations de Galilée forcés à se défausser, alors je ne suis pas un thuriféraire quand on connaît bien, de Pierre Bourdieu, mais je dois admettre il disait juste lorsqu'il écrivait qu'un Champ scientifique authentique est un espace où les chercheurs s'accordent sur des terrains de désaccord et sur les seins instruments avec lesquels ils son t'en mesure de résoudre ses désaccords et sur rien d'autre : le problème se pose lorsqu'à côté ou parfois au-delà des écoles de pensée critique se développe ce qu'on appelle une pensée dénonciatrice agressive menaçante et ne respectant pas les règles s'académique exprimée précédemment ses pensées dénonce dénonciatrice qu'elles nous plaisent ou non relève du débat d'idées ou du débat public et rien que ça, mais elles doivent respecter cependant la loi et les principes posés par l'État de droit, le débat d'idées s'il fait vivre la démocratie n'est pas régi par les règles académiques, c'est pour cela qu'il peut parfois générer l'hystérie et des patients, triste, c'est pour cela aussi qu'on a besoin de la rigueur de la recherche académique alors y a-t-il une vraie résonance du wokisme aujourd'hui dans les travaux de recherche en France moi-même enseignant, je me suis renseigné à ce sujet, j'ai trouvé peu d'éléments et je voudrais savoir si derrière ce mot fourre-tout, le ministère de l'enseignement de super la recherche pour, à travers les travaux

Madame la ministre. Monsieur le madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Gattolin. dans vos propos nuancés vous définissez d'une certaine manière, la différence entre les éléments de recherche qui ont vocation à être très plurielle, très diverses, et au contraire, encore une fois, qui font l'honneur et la qualité de nos grandes universités françaises. Et le passage finalement de ces éléments de recherche donc d'un débat descriptif des sciences sociales, un comportement prescriptif celui qui viendrait imposer soit une pensée unique, une pensée autorisée une pensée dominante face à une pensée ou en tout cas des auteurs qu'on n'aurait plus le droit d'étayer ou pas, pour cela, nous avons aujourd'hui parce que c'est la volonté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche consolider d'une certaine manière, un certain nombre d'outils qui permettent de regarder la. Pluralité de ces éléments, je pense que nous serons en capacité de vous apporter c'est différents des mais ce qui est certain, c'est que, aujourd'hui, le renforcement du CNRS, l'augmentation des moyens, des laboratoires de plus de 10 % de 15 % en 2022 l'augmentation également du taux de succès des projets déposés dans leur diversité, ou encore la création de plus de 360 congé spécifique à la recherche ont vocation à garantir effectivement cette pluralité et donc dans les sciences humaines, en particulier le les, les, les, les recherches les plus descriptive et non pas ce qui amène à des comportements qui viendrait réduire en réalité ce petit joyau qu'on appelle l'université française. Merci madame la ministre, pour ces ces précisions et effectivement il est important de regarder cela, moi j'ai tous les ans une vingtaine d'étudiants, il y a 2 ans, on j'ai lancé un débat dans le cadre des politiques culturelles de la France, la question du langage et de l'écriture inclusive, j'avais les 3 quarts qui me disaient qu'ils y étaient favorables, quand j'ai proposé des mémoires ou d'écrire des travaux sur ce sujet, personne ne l'a développé parce que personne n'était capable de trouver aussi une argumentation scientifique organisé dans l'état de l'art d'un travail universitaire pour faire cela et par ailleurs les travaux qui aimeront été rendu personne n'a osé, même si j'ai pas fermé la porte à ce que ce soit écrit en écriture inclusive, je crois qu'il ne faut pas confondre le débat de d'une jeunesse étudiante qui est intellectuel et qui quote-part qui saute sur tous les courants de pensée et puis la réalité de ce que l'université dans son encadrement précis longue de docteurs de chercheurs produit réellement, c'est pour ça que je crois que si on veut avoir une vraie image de l'université de la recherche, il faut se baser sur les grands travaux les plus grandes publications scientifiques et les travaux de doctorat, je vous remercie. La parole est à monsieur Jean-Pierre de colle pour le groupe, les indépendants et pour 5 minutes.

c'est le titre d'un documentaire réalisé en 2016 par le Grant sur le mouvement Black Live mateurs, c'est devenu un mot d'ordre : aux États-Unis, pour tous ceux qui considèrent les sociétés occidentales comme structurellement raciste mais aussi sexistes islamophobe ou homophobe, c'était donc rester éveillé, restez vigilants soyez sur vos gardes la discrimination sont partout, nous les pratiquons sans le savoir, nous sommes coupables à notre insu, telle est le mot d'ordre du wokisme il nous renvoie à une faute que nous commettons sans même en avoir conscience, littéralement le wokisme renvoie d'abord à une faute d'orthographe dans la langue de Shakespeare, il aurait fallu dire que nous, et non au au commencement était l'erreur, déjà on pourrait considérer que l'étymologie du signifiant est anecdotique tant le signifier problématique j'en doute, j'en doute car, au fond, se cache l'idée que la langue en soi est un mécanisme d'oppression et de discrimination, on court aujourd'hui le risque de ne pouvoir s'exprimer sans blesser quelqu'un en France, nous subissons déjà les assauts de cette exégèse moralisatrice, elle revêt de multiples visages et répriment toute forme d'expression la censure frappe autant la langue du quotidien que le langage artistique concernant la langue du quotidien cette censure s'appelle écriture inclusive, ses promoteurs soutiennent que les règles de grammaire française constituent des mécanismes d'oppression à l'encontre de la gente féminine, mais à la vérité, l'écriture inclusive exclu et discrimine elle oppose sans cesse les 2 genres sans jamais les accorder, nous le constatons tous les jours cette écriture inclusive se propage partout, elle gagne même l'université, ses professeurs, ces élèves et son administration, le ministre de l'Éducation nationale avait pourtant été clair sur ce sujet, cette déformation du français n'a pas sa place dans notre administration, elle ne a pas non plus, a fortiori dans les lieux où se transmet le savoir, j'étais à l'initiative d'un débat organisé sur ce thème, ici au Sénat en mai dernier et je me réjouis que le débat continue, j'en profite pour saluer l'initiative de ma collègue Pascale Gruny, sa proposition de loi prolonge ainsi ces travaux nos discussions s'inscrivent donc dans une forme de continuité pour qui je me fais l'écriture inclusive ces dérives prospère à l'université Alger remettent en cause le véhicule du savoir, c'est-à-dire le langage en tant que telle, je l'ai dit, le wokisme n'accepte pas sa censure qu'à la langue du quotidien, mais aussi au langage artistique comme dans les Campus américain de plus en plus d'étudiants se posent en France à ce que certaines manifestations culturelles et lieu, au prétexte qu'elle perpétue des stéréotypes sexistes ou racistes ainsi en mars 2019 des groupuscules soi-disant anti-racistes manifester contre une représentation de la pièce, défilent les suppliant dans l'amphithéâtre Richelieu en Sorbonne la raison évoquée par ces jeunes créateurs, le metteur en scène avait décidé de couvrir le visage de masques, dont certains étaient noirs, ils il y aurait, qu'il s'agissait là de renouer avec la pratique classique du théâtre antique, je ne crois pas utile de rentrer dans un débat propres aux études théâtrales, y a de choquant dans cet événement qu'on vous a bien d'autres survenus depuis, c'est que les groupuscules s'attribue un rôle de censeur que personne ne leur a confié, il faut le dire tout Net : la culture doit rester libre de se censure, nous ne pouvons pas baisser la garde, nous devons au contraire explorer les voies d'action qu'elle soit d'ordre législatif réglementaire même culturel, pour y mettre un terme, nous devons également mener la bataille sur le plan des idées, il faut expliquer pourquoi on ne combat pas le racisme en interdisant des pièces de théâtre, il faut expliquer pourquoi on ne lutte pas pour l'égalité entre les hommes et les femmes lorsqu'on n'est plus exclu des hommes de certaines réunions, il faut expliquer enfin pourquoi on dégrade le débat intellectuel lorsqu'on interdit certaines personnes de s'exprimer au motif qu'elles ne pensent pas comme il faut l'université est par définition le lieu où s'ouvrent les esprits et où se transmettre les savoirs, le wokisme, il n'y a pas sa place, l'enjeu est d'autant plus grave que pour les générations actuelles et futures, l'université pourrait donner à cette idéologie l'apparence d'une validation éthiques et scientifiques, il en va de la préservation de notre langue et de notre culture. Merci. C'est optionnel à Madame la ministre, ce n'est pas optionnel, ça veut dire que vous avez un peu de temps, si vous le voulez. Merci madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, d'école, vous avez mis en lumière un sujet important, celui de l'écriture inclusive et de ce point médian, la position du ministre Jean-Michel Blanquer et vous l'avez rappelé de Frédéric Frédérique Vidal ont été extrêmement clair, il n'y a pas la place à cette écriture inclusive aujourd'hui dans nos universités au sein d'établissements d'éducation, de l'Éducation nationale pour une raison toute simple, hein, ce n'est pas la grammaire française, ce n'est pas du français, par contre monsieur le sénateur, vous avez également parlé de la pièce de théâtre des suppléants et. Nous sommes en accord total jamais dans notre pays, nous devrions nous accommoder de censure de censeur ou d'une moralité qui nous imposerait de nous priver de la grandeur de la culture française en particulier je sais que ça a été un enjeu important puisqu'il a créé du débat, mais elle a été rejouée en avril, en présence de Frédérique Vidal et à l'époque de Franck Riester ministre de la culture, je vous remercie. Madame la ministre, je veux vous remercier pour cette réponse, vous avez très justement rappelé la posture Monsieur le Ministre bancaires concernant l'écriture inclusive la pédagogie est l'art de la répétition, vous l'avez très justement fait je vous en remercie. Merci, la parole est à monsieur Jacques Grosperrin pour 4 minutes pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, la science et la connaissance doivent être respectés dans leur autonomie, leur indépendance, indispensables à la transmission n'admettent aucune pénétration idéologique le savoir n'est pas une opinion la vérité scientifique n'est pas une croyance, c'est une conviction politique l'université aujourd'hui, mais pas partout, pas partout le théâtre d'affrontements idéologiques, menée par les tenants d'une déconstruction assumé contre l'institution elle-même ceux qui me connaissent le savent, que mes propos ne sont ni un fantasme, dit une obsession, c'est une réalité vécue dans les exemples là abondent, un phénomène que dénoncent une majorité d'enseignants chercheurs qui constate une confusion croissante entre la liberté académique, la liberté d'expression, ma préoccupation et laïque et République a une je suis inquiet devant les dérives constatées, il ne faut pas baisser la tête devant la bien-pensance moralisatrice, celle d'une gauche communautariste, en panne d'idées très éloigné dans la réalité, d'égalité, d'émancipation et je pense à tous ces étudiants, c'est vieux travailleurs qui aspirent à penser par eux-mêmes et auquel on veut imposer un nouveau terrorisme intellectuel, ils subissent une atmosphère pesante, il constate une situation dans laquelle il n'est plus possible d'avancer l'idée que le voile est un symbole d'oppression de la femme par l'homme, ils se font traiter d'islamophobe de raciste et d'homophobe par un discours extrémiste qui sature l'espace universitaire comme à ce jour, jour, le montant, nous étions en avoir fini avec la contamination de la recherche par le militantisme, Madame la Ministre, nous avions tort certains de nos universitaires engagés tente à nouveau de conquérir les amphithéâtres, il délaisse le cadre, la démocratie et du bulletin de gosses certainement pas Gilles pour eux minibudget par leur égo et ne sachant pas où se tourner, ils ont jeté un coup d'oeil outre-Atlantique et décidé que la race, le genre les discours de domination leur permettrait à peu de frais en Laurent leurs étudiants d'exister, il recherche une revanche à tout prix mais sur quoi le militantisme académique dans la confusion à la provocation veut le beurre, l'argent du beurre, peu lui importe l'affaiblissement de tous L à devenir de ces étudiants, nous n'acceptons nous n'acceptons pas le monde social que certains chercheurs militants mettent en avant un appauvrissant d'autant les ressources conceptuel d'université, il tend sans prendre de risques excessifs statutairement de cumuler la posture du chercheur avec celui de l'acteur, personne n'est dupe de leurs techniques de déconstruction, même si l'intimidation empêche parfois de la dénoncer, car les menaces sont bien là l'état d'éveil le bloquiste permanent devant toutes les discriminations, c'est utiliser à plein la légitimité potentiel des causes défendues grâce à la sensibilité à l'égal l'idée des droits, la confusion recherche militantisme s'ajoute alors à la cancel culture pour imposer une conception égalitariste, comme seul critère de voies de production académique les toits, l'État doit apporter de nouvelles garanties devant les attaques dont la liberté académique et victime, il faut mettre un terme à la confusion qui s'est installée, les menaces internes et externes sont incontestables : nous attendons encore les conclusions de l'enquête dans la recherche universitaire, les moyens d'agir existe pour les services de l'État, de nombreux articles du code de l'éducation le disent clairement l'activité d'enseignement, de recherche doit s'exercer dans des conditions de totale indépendance et dans la sérénité indispensable à la réflexion et à la création intellectuelle, le service public de l'enseignement supérieur et laïque indépendant de toute emprise politique ou idéologique, les principes de je m'excite de tolérance ne sont pas négociables les possibilités de rappeler efficacement le code de l'éducation et d'opérer des contrôles qui s'impose, ne manquent pas pour autant que l'avant le thé politique ça n'exprime encore faut-il que les textes eux-mêmes ne soit pas modifié par l'État, une modification du code de l'éducation, en date du 24 décembre 2020 interroges par exemple quand elle affirme que les services publics d'enseignement supérieur, contribue à la lutte contre les discriminations à la réduction des inégalités culturelles ou sociales, mais comment ne pouvant pas être d'accord à l'autre article du même coup, de l'éducation a été modifié pour affirmer que l'enseignement supérieur mais une action contre les stéréotypes sexués, il y a parfois une forme d'inconscience des enjeux de l'autonomie scientifique et de la liberté académique, quand le ministère utilise lui-même un vocabulaire militants en terme de lutte et d'action à mener les aberrations administratives et humaines qui découle de l'évolution des tests textes sont innombrables, chacun doit prendre conscience de l'emprise croissante de ce militantisme dévoyés par certains et ne pas transformer les salles de cours ont lieu donc donc finalement merci madame la présidente. vous aviez 4 minutes mais vous regarder en face, on voit très bien. Merci madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur coopérants. Vous avez parlé de de choses je pense qu'ils sont absolument essentiels : l'égalité des chances, l'égalité réelle, l'émancipation par l'université, évidemment, c'est un projet c'est un projet d'une de notre c'est de notre République, c'est la promotion d'elle, de la valeur travail, de la méritocratie et de la grandeur finalement de nos universités et de toute notre système scolaire et dans ciment supérieur et monsieur le sénateur, vous avez rappelé les modifications au code de l'éducation. Ces modifications, elles sont le fruit de travaux qui ont été votées au sein de cette chambre comme au sein de l'Assemblée nationale et c'est bien le fruit du débat parlementaire, dans le cadre, finalement, de l'égalité et de l'accompagnement des étudiants boursiers que c'est ces évolutions ont eu lieu et je crois que c'est aussi la grandeur que note de notre pays que d'aller chercher finalement la lutte contre toutes les discriminations, le finalement, le fait que toute une nation se lève quand il y a un acte raciste, homophobe, antisémite, parce que finalement, monsieur le sénateur, et c'est peut-être la grande différence entre toutes ces théories, celle d'une France universaliste et celles qui n'acceptent pas l'installation de ces discriminations où finalement que le combat contre les discriminations serait exclusivement réservé à ceux et c'est bien la grande différence entre l'universalisme et l'essentialisme dans le débat politique et pas pour le coup, universitaire, la seule les seules limites en réalité à la liberté académique liberté d'enseignement au sein de nos universités, que ce soit dans la recherche dans l'enseignement, ce sont ce que le législateur a posé comme limite je pense évidemment au négationnisme je pense évidemment aux appels à la haine, mais rien d'autre et si nous cultivons la qualité de nos débats, alors nous trouverons je pense, hé bien, des citoyens éclairés demain dans leur expression et de leurs fondamentaux et nous ne regarderons plus de l'autre côté de l'Atlantique, je vous remercie. Merci madame la présidente, merci madame la ministre, pour votre réponse et comme mon collègue m'a expliqué son je connais votre engagement vis à vis de cela même si la CPU souhaite que justement cette liberté académique soit inscrite dans la Constitution, je tiens à dire que ce ne sont pas toutes plaisir qui fonctionna si ce ne sont pas tous les enseignants-chercheurs, qui fonctionnent ainsi mais ce moment des discussions permettra en tout cas au niveau de ça, de ce rayonnement de pouvoir parler de quelque chose qui est grave en France et j'aurais mais néanmoins je sais les difficultés que la ministre de l'enseignement supérieur a pu avoir, lorsqu'elle a rejoint Jean-Michel bancaire je voudrais une porte, petite partie pourrait là à ce moment-là, mais il dit aussi que je vais m'entendre le président de la République s'est exprimé sur ce sujet qui est tellement important pour l'avenir de nos étudiants et pour l'avenir de la France, merci. Monsieur Thomas de ce si vous avez la parole pour 5 minutes pour l'Europe Écologie Solidarité territoire. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, en prenant connaissance de l'ordre du jour, j'ai eu un ouf de soulagement : enfin, enfin le vrai débat, le vrai choc de société le vrai enjeu de ce nouveau siècle. Le danger, finalement nommé ou autisme enfin enfin notre droite front bien française importe la panique morale de la droite américaine, après j'ai Bolsonaro et Donald Trump s'est phare de la pensée néoconservatrice, il était temps que nous nous attaquions nous aussi à la recherche, à la recherche en sciences humaines et sociales en particulier, on avait eu les Gender Studies, la théorie du genre et on a fait un petit détour par l'écriture inclusive, puis l'islamo-gauchisme mais on se perdait un peu alors bienvenue aux nouveaux dangers celui qui unifie tous les réactionnaires français le wokisme. Certains, dans ma famille politique, pensait naïvement qu'il s'agissait d'un épouvantail qu'on agite pour parler d'un mouvement de jeunes gens éveillés qui interroge l'histoire et les déterminismes remettent en question la domination de nos sociétés se questionnent sur nos grands hommes demandent un égal traitement des humains, quels qu'ils soient ou s'intéresse par exemple à la manière dont le langage produit d'énormes mais, pour vous, on l'a bien compris, ce sont des extrémistes, des extrémistes que vous estimez même plus dangereux que l'extrême droite. Cette extrême droite bien réel pourtant aujourd'hui qui menace de mort, des personnalités politiques qui produit des tribunes appelant à la guerre civile qui a fomenté 10 attentats déjoués depuis 2017 ce danger-là, visiblement, ne mérite pas de débat dans notre assemblée. Et sur ce point, je me réjouis de constater que vous êtes sur la même ligne que le gouvernement, rendez-vous compte, au moment même où toutes nos écoles étaient dans la tourmente de la valse des protocoles sanitaires notre ministre Blanquer a posé un acte fort, ouvrir un colloque sur le wokisme. Un colloque où se libérer une parole de comptoir durant 2 jours sur la résistance à toute forme de progressisme toute forme de liberté académique, voilà la vraie priorité une priorité aussi pour la ministre de la recherche, ça a été dit au moment où les étudiants souffrait des mois de confinement de distanciel de précarité galopante madame Vidal a su justement, justement nommé le mal est commandé une enquête au CNRS sur l'islamo-gauchisme qui gangrène aux universités. Peu importe si le CNRS a condamné l'utilisation d'un terme qui n'a aucune réalité scientifique, il y a une enquête qui remet en cause la liberté académique, peu importe, cette enquête n'a jamais vu le jour, l'essentiel c'est d'en avoir parlé d'autres si on avait besoin d'en parler, prenons le cas de Laurent Wauquiez qui a promptement couper les subventions de la région à Sciences Po Grenoble principalement des aides aux étudiants d'ailleurs pour une affaire montée de toutes pièces, qu'importe que toute la communauté éducative, appelle à cesser la stigmatisation de cet établissement, ce qui compte, seul symbole et pourtant on a eu là une attaque directe, concrète sur les libertés académiques d'autres parlementaires ont voulu jouer voulu jouer avec ce totem, Julien Aubert et Damien Abad, à l'Assemblée nationale ont demandé début 2021, la création d'une mission d'information qui reprenait exactement les termes du débat d'aujourd'hui avec la finesse d'analyse qui les caractérise, ils se sont permis un parallèle entre le nazisme, stalinisme et le mouvement dont nous parlons aujourd'hui après avoir osé écrire Islam conservateur et écriture inclusive marchent main dans la main, ils ont suggéré tout simplement de remettre en cause la liberté académique pour traiter le mal à la racine, nous y voilà, mais je constate que cette demande d'émission n'a elle aussi été qu'une opération de communication qui n'a finalement mené à rien de concret et heureusement rien de concret, mais peu importe, car le mal est fait. Et cette fois-ci, chers collègues, je dis avec sérieux et gravité, c'est de votre faute, main dans la main avec le gouvernement, vous attaquez la recherche universitaire vous jeter le poison du soupçon de l'anathème principalement sur le, sciences humaines et sociales, sérieusement des menaces qui pèsent sur l'université et les libertés académiques alors la liste est longue et le prétendu wokisme ne figure évidemment pas la paupérisation de la recherche, notamment en sciences humaines et sociales, la précarisation des jeunes chercheurs, des milliers d'étudiants dont on ne permet pas à l'inscription en master, plus d'un jeune sur 10 sous le seuil de pauvreté des universités et des Cruz dans un état calamiteux des files d'attente d'étudiants devant les psychologues et les guichets d'aide alimentaire et la volonté d'influence des grosses sociétés polluantes dans les écoles et universités mais je constate que vous avez parfois un rapport assez hermétique avec le réel ainsi à 3 mois de la présidentielle, nous avons droit à notre débat au ras des pâquerettes, un front climatique stigmatisant et foncièrement inutile lorsque la recherche universitaire va en compte de votre projet politique, un projet devenu ici impossibles à distinguer de ceux de l'extrême droite, alors oui, vous faites peser des menaces bien plus grave que les libertés académiques. Sur les libertés académiques que quelques outrances militante, on le voit clairement aujourd'hui la volonté d'annuler d'interdire de régenter la pensée provient en vérité de votre camp, l'ordre et la morale, c'est ça votre objectif tout le reste, les moyens alloués à l'université, le soutien à la recherche de la lutte contre la précarité étudiante, tout cela n'est pas que ce soir, et nous en avons une preuve éclatante : aujourd'hui, je vous remercie. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur dessus. Vous appelez au pluralisme et vous condamnez des colloques vous appelez au débat et vous condamnez finalement l'échange là le débat, le débat à la française au sein de notre diversité, le colloque que vous avez cité auquel Jean-Michel Blanquer avait. c'est un débat qui permet de poser des théories de dépôt de poser des discussions de poser des principes, de les voir Challenge et aux yeux d'ailleurs des étudiants, et c'est exactement ça qui construit l'esprit critique, monsieur le sénateur, nous avons un seul cap et une seule boussole, protéger les libertés académiques et d'enseignement, garantir un climat le plus sain et le plus serein au sein de nos universités pour que nos étudiants puissent s'éveiller, travailler, se questionner et finalement se construire leur propre et unique pensée : ne laissez aucune pensée s'installer comme finalement la seule autorisée, ne pas laisser s'installer l'autocensure et nous voyons à quel point aujourd'hui dans des universités outre Marine, il se passe quoi il se finalement il se pose la question de comment finalement ramenés à nouveau un pluralisme, nous, nous l'avons, nous l'avons héritée et nous l'avons finalement bâti depuis le la 3ème République, à nous de le garder, Monsieur le Sénateur dessus ah non finalement, alors même que votre combat aujourd'hui et de poser la question de de défendre cette cette ligne, hé bien, aujourd'hui, au sein de nos diversités, nous nous défendons cette liberté académique nous la garantissons par contre ces colloques, ils sont évidemment bienvenus dans un pays qui aime le débat, qui aime la politique, et qui aime la société.

Monsieur Ouzoulias si vous avez la parole pour le groupe républicain, communistes, écologistes et pour 5 minutes. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, le Sénat unanime par sa résolution du 4 janvier dernier a alerté le gouvernement sur les difficultés structurelles que connaissent les étudiants, les enseignants, l'enseignement supérieur. Il a considéré que l'université n'avait pas eu les moyens de gérer le crois continue des actes des effectifs estudiantins et que la qualité de l'enseignement, on avait pâti. Nous avons plaisir à constater que le président de la République partage l'essentiel de ce jugement, puisque le 13 janvier devant la conférence des présidents d'université, il a reconnu que son gouvernement d'effet que colmater les brèches et qu'il n'avait pas réussi à conduire une transformation systémique de l'université, dans l'ordre des priorités, l'urgence est là, dans la nécessité de donner rapidement aux universités les moyens d'assurer leur mission de service public au profit des étudiants et de la nation, alors que le paquebot universitaire et comme le Titanic menacé par de multiples voies d'eau, je me demande si l'objet de ce débat n'est pas de déterminer si la musique jouée par l'orchestre d'serait responsable du naufrage, néanmoins je partage cher collègue, votre volonté de Millau défendent la liberté académique comme principe protecteurs de l'autonomie des universités, des universitaires et des connaissances qu'elles produisent lors de la discussion de la loi dite de programmation de la recherche, j'avais défendu ici même, plusieurs amendements pour la conforter ainsi mon amendement 97 portait proposé de garantir l'indépendance des universitaires de protéger leur liberté d'expression et de leur accorder une protection fonctionnelle de droit, vous l'avez repoussée, mais je comprends que vous seriez maintenant disposé à engager une réflexion pour conforter les dispositions législatives relatives à la liberté académique mon groupe déposera donc une proposition de loi sur le sujet que vous voterez certainement en juin 1968 depuis l'université de Nanterre occupée, Paul Ricoeur, qui avait vécu physiquement ce que pouvait être une atteinte à la liberté d'expression donner cette définition de la liberté académique, le droit de l'enseignant, c'est d'abord le droit afférents à la compétence et à l'expérience tels qu'il a été sanctionné, non par les étudiants, mais par les autres compétent ses pairs c'est ensuite le droit à la liberté de pensée et d'expression en dehors de toute censure politique et idéologique, c'est enfin le droit d'accomplir son propre dessin de connaissances et de sciences dans l'enseignement et hors de de l'enseignement, la liberté académique et avant tout la liberté professionnelle d'exercer librement son activité d'enseignants et chercheurs dans un cadre de normes et de règles déontologiques définies par ce qui constitue cette profession, elle est donc à la fois personnels et corporatifs, comme l'écrit excellemment le professeur Olivier Baud la liberté académique suppose donc l'autonomie professionnelle et aussi l'existence d'une communauté par discipline scientifique dans laquelle règne, les 2 grands principes de la collégialité et de la cooptation, c'est-à-dire tout le contraire du principe de la hiérarchie et de l'autorité, le même professeur Baud est alors obligé de constater que ces 2 principes de collégialité et de cooptation ont été transgressées par de nombreuses dispositions législatives depuis l'adoption de la loi dite relative au respect aux libertés et responsabilités des universités jusqu'à celle dite de la programmation de la recherche. Pour conforter la liberté académique, il faudrait donc restaurer les principe de collégialité et de cooptation c'est-à-dire refonder la véritable autonomie des universités, est-ce vraiment votre projet politique, chers collègues, pour en revenir au strict intitulé de ce débat, de contrôle, je me demande s'il n'y a pas une forme de contradiction à 12 courir à la fois de la liberté académique et des théories académique qui la menaceraient est vraiment au Parlement, au pouvoir législatif de déterminer ce que les professeurs dont l'indépendance est garantie par la Constitution doivent enseigner qu'il y ait des atteintes à la liberté d'expression sur les campus, nul ne le conteste, mais comme le rappelait très justement le collège de déontologie de l'enseignement supérieur et de la recherche, saisie par la ministre, dans son avis du 21 mai 2021, 2021, les présidents des universités disposent de tous les outils pour assurer dans leur établissement la libre expression des idées et des opinions, le Parlement, quant à lui, doit défendre l'État de droit, en protégeant la liberté académique et les franchises universitaires merci, cher collègue. Monsieur le sénateur, vous l'avez rappelé la priorité la priorité de la priorité, c'est cette liberté académique et sa protection et l'accompagnement des présidents d'université dans cet exercice, c'est pour ça, vous l'avez dit la ministre de lancement supérieur et de la recherche a saisi le collège de déontologie qui lui a qui lui même a remis un avis aujourd'hui sert de base complémentaires en tout cas d'outils supplémentaires pour l'ensemble des référents au sein des universités, au-delà de cette action, il y a une volonté farouche d'accompagner évidemment les présidents d'université à chaque fois qu'ils en ont besoin, à chaque fois qu'il exprime pour également puisque c'est la doctrine du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, pouvoir reprogrammer ce qui a pu être annulé parce que il y a eu des troubles au sein des établissements sur plus de plusieurs centaines de colloques ou de débats, il y a eu une vingtaine de colloques ou d'événements qui ont été annulés et à chaque fois, le ministère a été aux côtés des présidents d'des présidents d'université pour pouvoir les reprogrammer puisque c'est la stricte et unique doctrine je vous remercie. Un président à la ministre à la c'est vraiment dommage qu'on soit en fin d'exercice législatif parce que je pense que vous aussi vous auriez voté notre proposition de loi sur la liberté académique qui aura réintroduit l'article 97 que vous avez repoussé c'est c'est dommage, mais on peut se faire et pour ça, que le président Marc on sera réélu comme ça vous pourrez ici dans cet hémicycle, défendre l'article 4 ans 17 l'article 97, il était essentiel pourquoi parce qu'il a accordé la la protection fonctionnelle de droit, de droit, le droit et vous savez que c'est un problème qui est essentiel dans l'affaire pâti cette protection fonctionnelle droit, elle a manqué et je pense que l'on aurait pu sauver sa vie, si elle avait accordé, c'est le 1er point le 2ème point c'est la collégialité et la cooptation et là je suis obligé de vous dire que la la loi de programmation de la recherche, les a mis en danger les 2 merci. Merci, la parole est maintenant Monsieur Pierre-Antoine Levi pour le groupe Union centriste et pour 4 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le wokisme, la cancel culture et la pensée des coloniale bah ce sujet qui a fait irruption, ces derniers mois dans le paysage universitaire et politique de notre pays et qui nous réunit aujourd'hui. Pourtant, quel paradoxe que les tenants de la pensée des coloniale, soit tout de même l'objet d'une certaine façon une colonisation mentale et intellectuelle d'une pensée venus d'Amérique du Nord, non la France n'est pas les États-Unis, nous n'avons pas la même histoire : nous n'avons pas les mêmes clivages. Alors pourquoi vouloir calquer un mode de pensée qui ne correspond pas aux réalités de notre pays, si ce n'est une volonté acharnée de déconstruction de la société de la part de certains militants d'extrême gauche qui ont visiblement quitté le Champ républicain. Notre pays est laïc universaliste, il ne reconnaît pas en son sein différentes communautés, n'en déplaise aux tenants du courant de pensée des coloniale. Cependant, le passé doit être regardée en face sans repentance ni complaisance, c'est le travail des historiens, des chercheurs, des universitaires en cela la liberté académique de les protéger, c'était en partie le sens de la loi de programmation de la recherche que nous avons voté dans cet hémicycle le 20 novembre 2020, il n'est nullement question de transiger avec la liberté qu'elle soit académique ou d'expression ne tombons pas dans ce piège, pour autant, soyons réalistes et ouvrons les yeux, la liberté académique est aujourd'hui le prétexte pour certains, de développer des thèses qui mèneront à terme une régression de ces mêmes libertés. Les tenants de ce courant de pensée qui, je le pense et mortifère pour l'unité nationale savent parfaitement naviguer et utiliser le système au profit de leur idéologie afin de se voir attribuer bourses de recherche, les divers crédits universitaires, c'est peut-être politiquement incorrect, donc je veux dire cela, mais je l'assume. Qui aujourd'hui aurait pu très que le domaine des sciences humaines, a connu une politisation constante depuis 60 ans. Qui peut penser que la politisation de certains travaux de recherche est un fantasme. Cette question des libertés académiques se pose même aujourd'hui au niveau européen, avec le lancement d'un observatoire européen des libertés académiques. Mais comment être rassuré lorsqu'on entend des déclarations de la commissaire européenne Helena Dalli préconisant dans un guide à l'usage des fonctionnaires européens. De ne plus utiliser le terme Noël afin d'être plus inclusif pour les personnes ne le fait-on pas le préféré des prénoms comme Malika Julio au lieu de mariage pour ne pas présupposé que tout le monde et chrétien, ou encore pire, ne pas utiliser le terme citoyens pour ne pas froisser les migrants et apatrides, il y a de quoi être inquiet, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Alors, notre société est de plus en plus segmenté, de plus en plus opposés. Ayons mutuellement le courage de dénoncer tout ce qui porte atteinte à l'universalisme républicain. Il y a le courage de dire non à tous les extrêmes dans leur volonté de division et de déconstruction. Oui, on doit, pour défendre son pays sans être taxé de nationalisme. Oui, on doit pouvoir défendre l'histoire de France sans être accusé d'être un promoteur de la colonisation disque tabagisme encore oui, on doit pouvoir défendent la gastronomie française sans être vilipendés d'être raciste sous un suprématisme blanc comme cela est arrivé il y a peu, un candidat à la présidentielle. Entre républicains, soyons à la hauteur des défis que nous pose l'irruption du gauchisme d'ailleurs chers collègues accepter d'utiliser un mot est déjà en soi une acceptation de son concept. Face à cette horrible anglicisme wokisme et ce qu'il représente ne soyons pas naïfs et luttons ensemble contre la déconstruction de ce qu'est la France, je vous remercie. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, Libye, effectivement, nous partageons ce combat pour une République universaliste qui donne la chance à chacun de ses enfants, puisque ça a été rappelé la définition de la nation, se basant sur Rhône Ronan et la plus en réalité la l'héritage le plus beau qu'on ait c'est que devient français, celui qui le veut, qui rentre dans le combat de ces valeurs qui maîtrise son histoire et qui finalement fait de notre pays de notre grande nation, une des plus grandes au monde, c'est exactement ce que vous avez rappelées. Monsieur le sénateur effectivement l'opposé de ça, c'est d'accepter des propos comme ceux que nous avons pu voir sur certains nombres de travaux qui exclurait des mots, c'est ce qu'on disait tout à l'heure cette autocensure qui peut s'installer et qui n'a pas vocation à l'être, c'est un débat politique, idéologique et qu'il faut mener en tout cas que nous menons,

et si on est honnête vis-à-vis finalement de notre histoire et qu'on la prend dans sa globalité, s'il y a un état où il n'y a pas de racisme systémique, c'est bien le nôtre et il en a fait la preuve. mais, madame la présidente, Madame la Ministre, merci pour la sincérité de vos propos que rajouter après vos propos, je voudrais quand même simplement vous poser une question puisqu'on parle du wokisme plus très longtemps de l'université Frédérique Vidal devait il y a quelques mois, nous avait annoncé qu'elle rendrait un rapport demandé au CNRS sur les gauchisme et maintenant sur le gauchisme voudrions savoir où en est ce rapport et quand est ce qui va sortir. C'est la parole est maintenant Monsieur Bernard fédère pour le groupe RDSE pour 5 minutes. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. De quoi le gauchisme est-il le nom. Pourquoi nous faut-il être vigilant envers cette théorie de la vigilance et que se cache-t-il derrière ce terme qui nous vient d'Amérique. Il a le goût de la revendication des Noirs américains, l'odeur de la révolte des descendants d'esclaves, mais il n'ensemble, il ne semble en être qu'une indigeste mixture une usurpation une usurpation indigne et intolérante en France, nous ouvrons les maisons des adolescents jusqu'à 25 ans, rien d'étonnant à ce que nos universités recueille également les contestations nécessaires aux remises en question à l'adolescence, mais au-delà de l'indignation érigée en vertu suprême au-delà du ni pour, ni compte bien au contraire de Coluche s'insinue parfois et même s'impose une intolérance envers tous et tout Voltaire se serait battu pour le droit de s'exprimer, de ceux qui ne pensaient pas comme lui, aujourd'hui, les adeptes du wokisme peuvent partager des idées, mais se battre qu'on ne se qui les exprimerai sans leur légitimité. Barack Obama ne serait qu'un blanc à la peau noire et certains homosexuels des hétérosexuels en couple avec des personnes du même sexe que. Cette cancel culture comme il faut l'appeler serait risible si elle ne par l'intransigeance jusqu'à l'intolérance, on déboulonne des statuts en dehors de toute contextualisation historique cette déconstruction qui nous revient d'Amérique après l'exportation bien mal traduite de Derrida tente à éteindre nos lumières. Le disciple d'Alain que je m'efforce d'être ne rendra pas et je le cite, mépris pour mépris et pourquoi c'est qu'au fond du radical qui obéit toujours il y a un esprit radical qui n'obéit jamais, qui ne veut point croire qui examine et qui trouve dans cette farouche liberté quelque chose qui nourrit l'immense amitié humaine et c'est l'égalité, l'esprit d'égalité c'est d'un côté, la résistance, le refus d'acclamer le jugement froid de l'autre, c'est la confiance en l'homme, l'espoir dans une instruction et une culture égale pour tous, fin de citation. Comment tolérer l'intolérance de ceux qui interdisent à une universitaire de faire une conférence dans une université, parce qu'elle exprimerait des idées différentes. Le wokisme s'oppose à l'uniforme à l'universalisme en refusant le débat, les échanges, le brassage des idées d'où jaillit des concepts une pensée supérieure. Le wokisme sous couvert de vigilance accrue à toutes les formes de discrimination se révèle être une idéologie dogmatique, prenant le communautarisme, la culture du bannissement et du politiquement correct et pourrait porter atteinte à l'unité républicaine. à à trop avoir privilégié l'excitation d'esprit critique certes nécessaire mais qui doit s'exercer face à l'affirmation de nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité essentiel et que nous avons établis au fil de notre histoire et des progrès de la science nous laissons notre jeunesse dépourvus de repères entre ou contre lesquels se construire et qui se perd hors des limites que nous avons su tracer. Ayons le courage de les défendre plutôt que de laisser des imposteurs en redessiner les contours réécrire l'histoire, comme cette campagne présidentielle débutante nous en apporte de tristes exemples. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Philhar vous avez fait un plaidoyer à l'unité républicaine qui illustre qu'en réalité ce débat est un débat évidemment au sein de l'université, mais également dans notre société, et au-delà de la question de la recherche de l'enseignement, effectivement c'est où s'opposent 2 visions de notre société, quel plus beau plaidoyer que celui de l'esprit critique, celui de la Défense en réalité de toutes les expressions sans aucun angélisme sur la volonté finalement d'imposer une seule ligne puisqu'une autre, tout cela c'est bien les les esprits éclairés finalement d'illustres citoyens qui l'ont bâti, merci monsieur le sénateur. Merci madame la ministre, effectivement, notre société a besoin d'autorité mais d'autorité de compétence cette autorité qui réhabilite la science et éviterait qu'on puisse voir toutes ces, toutes ces lorsqu'on voit des gens porter une étoile jaune parce que on leur propose un vaccin gratuit, je veux dire qu'il y a des dérives qui sont importantes et Madame la Ministre, on attend, à la fois de l'autorité de l'État, l'autorité aussi des universitaires pour pouvoir pro-fixer des repères qui soit suffisamment étayant pour notre jeunesse. Madame la présidente, madame la Ministre, mes chers collègues, le terme wokisme n'ayant pas encore intégré le Petit Robert, je souhaite partager avec vous la définition qu'en donne Pierre Valentin dans son étude à l'idéologie Walk anatomie du wokisme être signifie réveiller, il s'agit d'ici d'être réveillée aux injustices que subissent les minorités dans les pays occidentaux, cette idéologie connaît une forte progression, l'émergence de cette nouvelle culture morale dans laquelle le statut de victime devient une ressource sociale requiert certaines conditions ces conditions sont plus plus ou moins présent dans les sociétés occidentales, bien sûr, mais plus particulièrement sur le campus des universités américaines où le wokisme, il est plus qu'influent le plus souvent, les militants sont issus de familles aisées, enfant, ils ont connu de trop bref moment de jeu libre et sans surveillance adulte, il peine à se débarrasser de l'attitude de la biture prise en consistant à rechercher une autorité instituée en cas de conflit avec une autre personne au lieu de le régler directement même l'une des conséquences et la croissance d'une bureaucratie universitaire chargé de poursuites et de prolonger cet état de surprenant voilà, cette définition est intéressante et à l'heure où l'idéologie Walk essaient de s'imposer dans le débat public et, plus grave encore, dans les rapports entre les citoyens, il me paraît important d'être vigilant sur l'américanisation de notre société et sur les tentatives hasardeuses et fallacieuses d'assimilation entre la France et les États-Unis et pour lutter contre ces dangereuses analogie, quoi de mieux que quelques faits historiques, la France n'est pas la mairie concentre nous sur le volet racisme de cette idéologie dont on a tendance à s'autoflageller il y a 80 ans, des Noirs, été lynché et pendu au nom de la justice dans certains États américains, le dernier lynchage recensés dans ce pays date de 1981 à la même époque, bien sûr, en France, des députés de couleur siégeait au Parlement pendant la Première Guerre mondiale, un régiment d'afro-Américains sera incorporé à l'armée française, suite à la demande du Maréchal Foch et malgré le commandement américain qui lui décrivait alors, et je cite le manque de conscience civique et professionnelle soldats noirs qui constituait, selon lui, et je cite encore une menace constante pour les Américains, ces considérations n'existait pas dans l'armée française, ils furent traités d'égal à égal, par leurs frères d'armes, ces hommes noirs sur les premiers américains a décoré de la croix de guerre française, j'aurais pu aussi parler de Jacques Bullard cet Américain, descendants d'esclaves qui s'engage dans la Légion à Paris en 1914 à l'âge de 20 ans il avait quitté son pays 2 ans plus tôt, pour échapper au racisme, il sera de tous les combats, avant de devenir le 1er aviateur noire du conflit en 1916 au sein de notre armée, les Américains refusant de confier un avion à un noir en 1940 il s'engage à de nouveau dans l'armée française mais sera blessés rejoindre New York d'où il soutiendra la France libre la Seconde guerre mondiale, parlons-en, lorsque la guerre frappa de nouveau les soldats de l'armée d'Afrique répondirent à l'appel du drapeau français ensemble, quelle que soit leur couleur de peau, cette conception était inconcevable pour nos alliés américains qui pratiquait là encore une politique s'égrènent à sioniste dans leur pays, mais aussi dans leur armée, cette politique conduira les Américains contraindre le général Leclerc de se séparer de certains de ses hommes, car ils étaient noirs au sein de la 2ème DB une fois de plus, la France se distinguait de l'Amérique à travers ces quelques exemples historiques qui sont très nombreux, il ne s'agit pas de nier l'existence du racisme mais d'argumenter et d'apporter de la nuance à ceux qui voudraient pour justifier leur idéologie, faire des raccourcis et de prendre la voie de la facilité sur un sujet si complexe, il est temps d'affirmer que notre pays et son histoire, non, rien ne comparable avec les États-Unis et ce qu'ils appellent le racisme systémique n'a jamais été n'est pas et ne sera jamais dans l'ADN de la France, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ce sont les menaces que les théories du wokisme font peser sur notre université notre enseignement supérieur et nos libertés académiques, même le ministre de l'Éducation nationale, monsieur bancaire avec je pas toujours d'accord, je le cite, il précise : déconstruire la déconstruction en cours, c'est ce qu'il a déclaré et je le soutiens lors du récent colloque sur ce thème à la Sorbonne le 7 janvier cessons de battre ainsi sa mort notre coulpe sur des faits du passé que nous analysons aujourd'hui avec les yeux d'aujourd'hui oui des inégalités ont existé existent et existeront malheureusement toujours entre les individus et nous devons les combattre, mais restons éveillés et fier de notre histoire et nos notre culture française restons fidèles à la France des Lumières qui combat l'ignorance diffuse de savoir et ne craint pas le débat, c'est l'ambition que notre université doit continuer à poursuivre l'université doit rester ouverte et libre, tout en sachant résister aux sirènes du Nouveau Monde, qu'il s'agisse du wokisme ou d'autres idéologies tout aussi dangereuses.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. J'espère que dans un futur proche, la société s'éveillera et sera le wokisme dans la rubrique du fait colonial. Ces coloniale le wokisme été introduit comme un cheval de Troie dans le milieu relativement perméable et pour eux, de l'université. Cette stratégie lui aura permis non seulement de se crédibiliser académique ment, mais aussi de gagner au passage quelques esprits pas suffisamment construit ou plutôt insuffisamment construits pour accepter finalement d'être déconstruit oui il y a bien une tentative de colonisation des esprits via le monde universitaire et ses enseignements, on pourrait dire, plus c'est gros plus ça passe, même si, à juste titre, on le sait, historiquement plus sensibles aux valeurs de justice et d'humanisme, ce monde universitaire et d'abord et avant tout fondée sur la rigueur du savoir et la fermeté de la raison. On pourrait en attendre moins de docilité et plus de résistance, le mot université contient le mot universel. Nous savons que la science et le savoir n'ont pas de frontières, le bouddhisme, la rupture avec l'humanisme, il dresse des catégories d'être s'humains les uns contre les autres, la liste est innombrable et il faudrait-il y ajouter celle des jeunes contre les vieux, sans que l'on sache jusqu'où doit aller la contrition la repentance et voire même si cela est possible. On se croirait revenu à l'époque des Cathares, tuez-les tous, le wokisme reconnaîtra les siens, lui, vers l'université n'a ni besoin de Qatar ni de carte Arcy Madame la ministre. Il y a quelques semaines, je vais interpeller madame Vidal, lors des questions d'actualité au gouvernement sur ce sujet, madame la ministre m'avait répondu que la main ne tremblait pas et qu'elle ne tremblerai pas dans le futur, notamment concernant le cas de Sciences Po qu'a fait le gouvernement depuis cette promesse, madame la ministre, parce que Anne ma soeur Anne ne tout voiture rien venir en tout cas, madame la ministre, nous ne nous voyons rien venir, nous attendons des actes aux promesses qui ont été faites au sein de cet hémicycle, je vous remercie.

Madame la présidente, monsieur, mesdames, messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, évidemment, à une demande une réponse sera établie et complétés, j'en suis certaine par les services du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais vous l'avez dit, quel plus bel endroit pour s'éclairer, pour débattre, c'est au sein de nos universités, s'il y a un combat à tenir, c'est celui du de la sérénité et de la qualité des travaux mais sans aucun angélisme. Bien, la parole est maintenant Monsieur Gérard Longuet pour 5 minutes pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, d'abord je voudrais franchement remercier Max Brisson, d'avoir demandé et obtenu ce débat car le Sénat est au coeur de ses responsabilités en évoquant ce qui peut impacter fortement dans les années à venir, notre pays et nous sommes en effet peut-être en avance. Je l'espère profondément d'un problème qui ne se poserait pas chez nous Jacqueline Eustache-Brinio avec beaucoup de raisons et avec de l'émotion à rappeler que notre culture, à l'égard de nos allez nos anciens colonisés n'était pas celle des États-Unis, et en l'ancien ministre de la Défense, que je suis tiens, effectivement, a souligné le sacrifice tentant la en première guerre mondiale que la Seconde Guerre mondiale, d'une part de nos ce n'y aller par exemple qu'on appelait sénégalais mais qui ne l'étaient pas tous, tant s'en faut, et l'intégration de troupes américaines noir lors d'or de la première guerre mondiale, donc les États-Unis ne sont pas la France, on a cependant le devoir de réfléchir pourquoi parce qu'il y a une idée absurde mais dévastatrice le savoir serait le résultat d'une oppression évidemment l'oppression au sommet de la pyramide de l'oppression, il y a un individu épouvantable, le mâle hétérosexuel blanc, j'en fais partie, pour l'instant, mais enfin, tout peut évoluer en revanche poser le principe du savoir comme une oppression poser le principe que toutes les minorités sont victimes et amener nos compatriotes puisque nous parlons de la France à essayer de savoir quelle est sa part de victimes mixing de d'être victime de victime risée c'est quelque chose d'extraordinairement dissolvant pour la société française, nous avons l'habitude de combat, nous avons l'habitude d'idées différentes, nous pouvons nous affronter et nous savons qu'il y a une règle qui est la majorité républicaine cette règle vole en éclats, parce que nous serions non plus des citoyens mais prisonnier de notre race de l'histoire de nos ancêtre s'et au fond le wokisme apparaît comme une sorte de renaissance du racisme le plus fermé le fermé le plus obstiné, le plus sectaire, on ne pourrait pas échapper à la fatalité de son ascendance alors que, justement, toute l'idée citoyenne de la République, c'est l'idée que l'on adhère à des valeurs qu'on ne les partage qu'on les vit qu'on les défend mais qu'on ait accepté, quel que soit son parcours et ce parcours d'ailleurs pouvant enrichir lui-même le tronc commun alors Madame la Ministre, pourquoi j'interviens à cet instant,

de Jean-Michel Blanquer hier dans ce colloque de la Sorbonne, il a eu raison d'y aller, était-ce trop tôt : était-ce trop tard en tous les cas, il l'a fait et il avait raison de le faire, en revanche, il y a 2 comportements qui sont singulièrement préoccupant le 1er, vous l'avez évoqué, j'ai pas tout compris, mais peut-être précise, vous les déontologues, je vois dans le déontologue se créer le risque de cette bureaucratie que Jacqueline Eustache-Brinio dénonçait et qui avait été dénoncée très bien par Pierre Valentin dans le document de la Fondapol cher Max, vue ces déontologue peuvent déboucher sur une bureaucratie du contrôle et ça il ne faut pas, il ne faut pas parce que quand vous créer une bureaucratie, elle cherche à se légitimer à se justifier et comme la victime toute toute expression s'adressant à elle comme une agression, vous allez avoir un débordement à peu près sans limite, c'est le 1er danger il faut clarifier les règles du jeu est renvoyé devant le droit pénal, ce qui se comportent par exemple avec des injures raciales ou bien du négationnisme, mais le reste, c'est un petit peu dangereux 2ème remarque : vous avez une réponse implicite au procès qu'adresse la domination du mâle blanc hétérosexuel bourgeois, si possible, c'est le recrutement des étudiants sur des critères qui ne rend de plus hommage au seul travail et à la seule réussite intellectuelle, j'ai été comme président de région avec le directeur de l'époque de Sciences Po, l'un des premiers à ouvrir les lycées professionnels, à des classes d'accès à Sciences Po, mais c'était des classes d'accès où il fallait travailler pour réussir, alors il y avait un soutien il y avait un appui mais il y avait du travail, aujourd'hui on s'aperçoit que des jeunes parce qu'ils ont le malheur d'être fils de bourgeois,

au profit de l'extérieur, ce serait une matière première qui affaiblirait notre pays et d'avoir des enseignants qui s'auto-censure aurait parce qu'ils auraient peur de s'exprimer librement.

pour 5 minutes. Impliqué à monsieur Longuet, ce qui lui permettra de vous répliquer et ensuite prendre vos 5 minutes. avec plaisir madame présidente puisque monsieur le sénateur Longuet a posé une question très explicite sur le rôle des déontologue et ce qui me permet également de rappeler l'importance et la qualité des propos de la sénatrice Eustache-Brinio sur le rappel historique fondamentale qui fait la grande différence de notre conception aujourd'hui de notre histoire et celle, anglo-saxonne, qui du coup amène en réalité une grille de valeurs, une grille de lecture qui n'est pas la nôtre et qui de fait fausse absolument le débat et le regard posé, c'était surtout un hommage rendu aux propos historiques de madame la sénatrice sur la question, monsieur le sénateur des déontologue loin de nous l'idée absolument de poser une bureaucratie évidemment nous envoyons le risque, comme vous l'avez souligné et l'objectif de ces déontologue c'est c'est d'accompagner les chefs, en réalité, les présidents d'université dans la lutte contre les conflits d'intérêts parfois la art les relations entre entre enseignants chercheurs d'entre eux, garantir l'intégrité scientifique des travaux mais surtout et avant tout, 0 censeurs 0 auto-censure, parce que c'est absolument le débat à tenir, il y a une liberté académique pleine et entière intégrée totale, ça veut dire quoi, 2 lignes rouges : elles sont définies par la loi et exclusivement par la loi de notre pays, c'est à dire non à l'appel à la haine et non au négationnisme au-delà de ça, liberté académique pleine et entière, monsieur le sénateur. Madame la Ministre vous interromps parce que Monsieur Longuet pour répliquer. Le diable se le diable se niche dans les détails et c'est la raison pour laquelle les parlementaires ont le devoir d'être exigeants et attentifs pour ne pas être débordé par des initiatives prises par ceux qui voudraient éviter les enquiquinent Oman et et qui achèterait la sérénité de leur établissement par des complicités inacceptable. Merci madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, ce débat a porté, posée par le groupe, les républicains au sein de du Sénat permet de poser des mots sur une réalité aujourd'hui dans notre pays mais poser également les protections. Hein, il ne faut absolument aucun angélisme aucun, c'est à dire que oui, il faut regarder les dérives que nous vivons parfois au sein de certaines universités et d'ailleurs je salue le fait qu'un certain nombre de sénateurs, quelle que soit leur banc ont rappelé ces dérives pour ne pas finalement globalisé naître dans un angélisme plan au-delà de ça nous avons un seul et unique enjeu liberté académique bien sûr protéger renforcer les moyens de l'université, et c'est ce que nous faisons avec la loi de finances, la loi programme de programmation de la recherche par l'accompagnement des présidents d'université, bien sûr, mais au-delà de ça, il ne faut pas se tromper de débat au-delà des recherches au-delà des enseignements, il ne faut pas laisser cette hausse censure s'installer au sein de nos universités, monsieur le sénateur Longuet, vous l'avez rappelé, je crois que c'est le climat au sein de muse diversité qui compte, nous ne pouvons pas laisser s'installer aujourd'hui en France, le risque de voir certains enseignants placarder leurs noms aux yeux de tous et finalement lancé une chasse aux sorcières qui amènerait à une chose, une sorte de régulation insidieuse par la peur parce qu'on vient très jetés en pâture le débat, l'échange, la controverse, hé bien non, ce qui est français, c'est le débat, la controverse, est évidemment l'étude de l'histoire dans sa totalité mais, mesdames, messieurs les sénateurs, se pose aussi la question aujourd'hui de la différence entre le combat politique dans notre société et effectivement les thèses de recherche, nous n'avons aucune vocation à réguler limiter le débat scientifique absolument pas, par contre, nous devons être les garants de ce climat de sérénité au sein de notre et de nos universités et dans le cadre de la vie étudiante, donc nous amèneront, avec évidemment la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'ensemble des moyens permettant ce climat apaisé et la protection des enseignants, des enseignants-chercheurs et évidemment des recherches et des doctorants la pluralité, un seul et unique objectif la pluralité des débats mais pour autant, pour permettre cette pluralité des débats, il faut évidemment des valeurs ferme des objectifs clairs et c'est pour ça que c'est tout au par c'est pendant tout le parcours de l'enseignement en réalité au sein de l'Éducation nationale jusqu'à l'arrivée, aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, qu'il faut accompagner les étudiants et en réalité, les citoyens de venir, c'est pour ça que. Aujourd'hui plus que jamais, il faut des repères, il faut de l'histoire, il faut des valeurs, il faut dire redéfinir des essentiel, c'est essentiel, c'est le rappel des un rappel historique, comme ça a été fait au sein à cette tribune, c'est évidemment une intégrité scientifique ce ne pas laisser finalement revoir toute une histoire ou l'installation de débats de combat visant à détricoter des héritages de cette histoire qui prennent parfois la forme de certaines statues ou encore le changement de titre d'Oeuvres littéraires ou encore l'interdiction de pièces de théâtre que nous avons vu, parce que ce combat en réalité ne doit pas nous lasser effectivement à chaque fois qu'il y aura une situation troublée ou un trouble obligeant une annulation de colloques, hé bien nous serons aux côtés des responsables et des présidents d'des présidents d'université pour permettre que ces colloques, puisse avoir lieu, ou encore ses pièces de théâtre et de se tenir, je crois que là est une ligne rouge à ne pas laisser franchir. Au-delà de ça, ça ne veut pas dire que nous ne luttons pas collectivement contre les inégalités compte la les discriminations ou encore contre le racisme, nous luttons contre toutes ces discriminations parce que nous regardons notre pays comme une nation, c'est-à-dire que nous regardons uniquement chaque personne comme un citoyen et rien d'autre, par contre, le racialiste est un nouveau racisme sera liste qui s'installe, qui prend qui prend ses racines dans un essentialisme posé en réalité oppose sépare fragmentent et créer des communautés, c'est évidemment le mal qui peut s'installer et qui s'installe dans un débat politique au sein de notre pays. Face à ça, il y a une vision qui s'opposent, celle de l'universalisme français républicain que nous portons au sein du gouvernement et que nous poserons comme en réalité un des sujets essentiels à l'unité nationale et c'est pour cela que tout à l'heure, il y a eu un certain nombre de questions sur la comment nous accompagnons l'université nous accompagne, diversité, par des moyens, les actes ont été posées, que ce soit des actes financiers qui soit le plan aujourd'hui pour le doctorat, que ce soit le renforcement du CNRS et j'allais dire la liste, elle peut être très longue de la précarité des étudiants jusqu'à l'accompagnement des enseignants chercheurs, ce n'était pas le fond du débat aujourd'hui, mais je crois que la négation des dérives que nous constatons, et évidemment un angélisme qui est particulièrement dangereux au sein de diversité mais au sein de notre société, donc une seule ligne, une seule, un seul combat évidemment la protection des libertés académiques le pluralisme et surtout et surtout une République universaliste, qui reconnaît, chacun de ses enfants comme citoyen et rien d'autre, je vous remercie.

Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, ça a été rappelé : Mal nommer les choses c'est ajouter aux malheurs du monde, or, selon un sondage IFOP, de février 2021, seulement 14 % des interrogé comprenait la signification du Maroc. Il faudrait pour donner du sens à ce débat, à commencer par arrêter avec cette paresse intellectuelle qui consiste à utiliser l'anglicisme wokisme pour masquer une idéologie qui a un nom : l'intersexualité pour les sociologues, il s'agit de décrire la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de domination ou de discrimination dans une société. bruissement d'un microcosme en mal de dessins positif il faudrait collectivement nous éveiller pour mieux prendre conscience de tout ce que l'humanité a produit d'injustice depuis la nuit des temps. Sommes-nous endormi, sommes-nous à ce point inculte pour mieux connaître notre histoire le privilège collectif serait-il l'apanage d'une petite minorité éclairée Tell Afar dans un océan baigné dans le brouillard. On le voit bien, ce courant est en réalité une vaste entreprise de déconstruction, qui consiste à diffuser la honte de notre identité, une autoflagellation intellectuelle et une repentance perpétuelle en jugeant avec les yeux d'aujourd'hui et le recul de plusieurs siècles. Tous les événements historiques Adam était-il misogyne, l'homme des cavernes étaient-ils respectueux de l'environnement, il suffit de poser les questions, les des constructeurs auront nécessairement une réponse. Ils savent sans doute aussi très exactement ce qu'ils auraient fait, s'ils étaient nés en 17 à Leiden. Le manque d'humilité de nuances et pour tout dire, d'objectivité et leurs caractéristiques essentielles et le pylône leur cible particulièrement les jeunes générations. Au pays des Lumières, le but n'est évidemment pas d'interdire une opinion, mais bien de permettre un débat contradictoire, notamment au sein de l'enseignement supérieur de prôner la liberté d'expression légale faculté d'exposer une diversité de pensée et de concepts. Et c'est là que le bât blesse car la censure et l'outil préféré des forces autoproclamé d'un soi-disant progressisme qui confère aux autres, c'est-à-dire à ceux qui osent émettre une idée contraire ou si seulement plus nuancée, un statut quasi automatique de fasciste, ainsi, nous ne pouvons que déplorer l'interdiction d'accès à nos campus universitaires, d'intellectuels ou de politiques ayant le culot de proposer des conférences qui ne s'inscrivent pas dans l'orthodoxie de penser d'une poignée de militants d'extrême gauche. Et il y a pire pour avoir osé affirmer qu'un homme n'est pas une femme, que notre pays n'est pas fondamentalement raciste pour avoir refusé de s'excuser d'exister, d'être blanc d'être Français d'être des étudiants se font traquer sur leur campus sont menacés de mort sur les réseaux soi-disant sociaux par quelques-uns qui confondent le comptoir des Indes avec celui du café du commerce, le coeur du problème, c'est bien l'inaptitude de cet idéal idéologie à combattre dans l'arène intellectuelle leur entre soi idéologique a fait fondre leur capacité à argumenter. Leur rhétorique repose sur la censure et la condamnation morale sans jamais discuter des fonds des problèmes soulevés. Vous le savez j'accorde une grande importance à la rigueur scientifique et je m'inquiète lorsque je vois des chercheurs en sciences humaines, défendre une idéologie qui ne conçoit pas la moindre objection. Ce progressisme de pacotille se complaît dans le confort de la mollesse des mots creux modelables à loisir on étire ses néologismes pour combler l'absence d'arguments est un mot qui n'a pas de sens, n'a pas de valeur. Islamophobie grossophobie transphobie en biphobie biphobie, psycho-phobie, c'est des constructeurs préfèrent médicalisé le débat en inventant de nouvelles pathologies afin de condamner moralement un adversaire sur l'autel de la modernité des mots utilisés à tort et à travers. Devenus caricaturaux, mots qui sont des mots qui ne valent rien, on peut légitimement s'interroger sur la finalité de la démarche qui devrait consister à protéger et aider les véritables victimes de discrimination. Mais le féminisme est il grandit lorsqu'on taxe de transphobes des femmes qui refusent de partager leur vestiaire avec des hommes est-ce de la grossophobie que de souligner que le poids est un facteur de mauvaise santé. Et favorise-t-on l'assimilation en affirmant à un immigré que le pays qui l'a accueilli. Et qui l'a vu grandir le méprise. Tous ceux qui sont attachés aux libertés académiques doivent s'émouvoir de la dérive que nous observons, mais bien peu s'exprime clairement, laissant la place aux extrémistes de tous bords qui parlent plus fort et souvent se rejoignent. J'accuse les tenants de cette pensée des constructifs de briser l'unité de notre nation de fragiliser la démocratie de dresser les citoyens les uns contre les autres en leur apprenant méthodiquement à se détester profondément a identifié dans l'autre un ennemi potentiel en le tenant responsable de tous ses malheurs, nous savons tous ce que la politique du bouc émissaire a produit comme catastrophe majeure par le passé, alors je conclurai par ces mots de Barbara fait que jamais ne revienne le temps du et de la haine. Je vais suspendre la séance pour quelques instants afin de permettre d'que la rotation.

La séance est reprise informe le Sénat que les commissions mixtes paritaires chargés d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la différenciation la décentralisation de la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, puis de la proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du défenseur des droits en matière de signalements d'alerte puis de la proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte, et enfin du projet de loi portant reconnaissance de la nation, réparation des préjudices subis par les harkis par les autres personnes rapatriées d'Algérie, anciennement de statut civil de droit local et par leur famille, du fait des conditions de leur accueil sur le territoire français est parvenu à l'adoption d'un texte commun que sont toutes parvenues à l'adoption d'un texte commun, voilà, nous allons maintenant poursuivre un ordre du jour qui appelle le débat sur le thème quelle politique ferroviaire pour assurer un maillage équilibré du territoire, c'est une demande de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, la parole est tout d'abord aux orateurs de la commission qui a demandé ce débat d'abord Monsieur Philippe Tabarot, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et ce pour 4 minutes. Madame la présidente, monsieur le président, l'enjeu, monsieur le Ministre, chers collègues, presque 4 ans après l'adoption de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire et plus de 2 ans après l'adoption de la loi d'orientation des mobilités rapportée ici par notre collègue Mandelli, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, a souhaité faire un point d'étape et prévoir un débat avec le gouvernement sur les orientations de la politique ferroviaire pour nos territoires et je dois vous dire Monsieur le Ministre, que les retours du terrain dont nous nous faisons l'écho aujourd'hui sont pour le moins contrasté malgré l'engagement du 1er ministre en décembre dernier à régénérer les lignes de desserte fine partout dans le pays, soit 9200 km, le compte n'y est pas des protocoles d'accord certes entre certaines régions l'état et SNCF, réseau ont bien été conclu afin d'identifier les lignes qui seront reprises, soit par les régions soit par SNCF, réseau et celle qui ferait l'objet d'un cofinancement comme actuellement, mais de quoi s'agit-il, sinon d'une manière pour l'État, comme souvent de se défausser sur les régions de l'entretien des petites lignes qui sont pourtant en complément du réseau plus structurants un gage d'égalité entre nos citoyens en matière de mobilité en dépit des promesses les montants consacrés par l'État à la régénération des lignes de desserte fine du territoire sont loin d'être à la hauteur des enjeux, le rapport du préfet Philizot évaluer le besoin de financement global à 7,6 milliards d'euros jusqu'en 2028 dont 6 4 milliards à engager à partir de 2020, ce qui représente plus de 700 millions d'euros par an, or et comme me l'a confirmé le ministre Jean-Baptiste Djebbari à l'Automne dernier à l'occasion d'une audition devant notre commission, environ 600 millions d'euros, il y aurait été consacrés mais sur les 2 dernières années soient seulement 300 millions d'euros par an, notre commission a bien proposé depuis 2 ans, de doubler les crédits investis par l'État dans les petites lignes afin de se rapprocher de la trajectoire définie par le rapport Philizot, mais ces amendements n'ont pas eu la chance de recevoir les faveurs du gouvernement, comment expliquer, monsieur le ministre untel décalage entre les engagements et la réalité de manière similaire, l'écart entre les intentions et les moyens mis en oeuvre en matière de développement de transports ferroviaires transparaît significativement dans le projet d'actualisation du contrat de performance entre l'état et SNCF, réseau, nous avons voté unanimement Sénat l'inscription de la loi dans la loi de l'objectif de l'augmentation de la part modale du transfert ferroviaire de voyageurs et de fret, pour autant, le projet de contrat qui devrait bientôt je l'espère en tout cas nous être transmis manque cruellement d'ambition et semble faire l'unanimité contre lui les nouveaux entrants régions de France ou encore la Fnaut ont tous déploré ses principales orientations, les moyens sont en effet insuffisants pour atteindre des objectifs que nous nous sommes fixés, monsieur le mini Giraud, il faut faire évoluer ce contrat pour donner au ferroviaire, les moyens de nos ambitions, enfin, toujours dans une perspective de maillage équilibré du territoire, je souhaiterais vous entendent, Monsieur le Ministre, sur le modèle de financement du transport ferroviaire et notamment en ce qui concerne le secteur conventionné et les petites lignes, nous savons le niveau des péages en France qui est très élevé, puisqu'il est en moyenne 2 fois supérieur à la moyenne européenne, région de France, a alerté le 1er ministre sur la trajectoire insoutenable d'augmentation des péages et invite à repenser le modèle de financement de SNCF, réseau à l'heure de l'ouverture à la concurrence, comment comptez-vous répondre à ces demandes, les régions déjà énormément investi en faveur du développement des transports du quotidien et dans une logique d'aménagement du territoire, comme l'a d'ailleurs rappelé un récent rapport de la Cour des comptes relatifs aux TER, monsieur le Ministre n'abandonnait pas ce Patrimoine national. La parole est à monsieur Olivier Jacquin, pour 4 minutes. Monsieur le Ministre, je tiens à saluer le président de la commission et mon collègue Tabarot d'avoir inscrit ce sujet qui m'est cher à notre ordre alors quelle politique ferroviaire pour assurer un maillage équilibré du territoire après 40 ans de tout TGV de terre sous-qui ont entraîné un grand nombre de fermetures de petites lignes et une très forte dégradation du réseau ferré national, je répondrai en 2 temps qui seront de questions Monsieur le Ministre, tout d'abord, relativement à votre méthode, enfin je parle, celle de votre gouvernement, vos priorités. Elles ont été tout d'abord consensuel lorsque lors des Assises des mobilités, il a été décrété que priorité serait donnée aux trains du quotidien, elles ont été un peu moins lorsqu'il s'agit d'ouverture à la concurrence et de réforme du statut vos méthodes ont été considérée comme acceptée et acceptable lors de la loi d'orientation des mobilités ou une loi de programmation. De nouvelles infrastructures, étaient considérées acceptables et raisonnables, ainsi qu'un plan de régénération du réseau ferroviaire, qui devait être confirmée par un contrat de performance de SNCF, réseau que nous attendons toujours depuis plus de 2 ans, mais alors, alors, vous commettez de têtes à queue majeur, à moins que ce ne soit des déclinaisons du en même temps tout d'abord, en juillet, le président Macron annonce de nouvelles lignes à grande vitesse non financées non programmés, certes nécessaires mais elles viennent déséquilibrer le programme et puis 2ème. Problème : ces fuites sur le contrat de performance de SNCF, réseau je salue la revue contexte qui nous annonce. Une très forte augmentation des prix des péages, Philippe Tabarot vient de le dire, cela n'apparaît pas sérieux après la crise des gilets jaunes après le Covid, qui a été une expérience de des mobilités. Il faudrait plus que jamais relevé le défi climatique : donner un vrai modèle économique au rail, que ce soit pour les voyageurs ou les frais en reconnaissant ses externalités négatives, je le dis en ce temps de crise de l'énergie que le faire, c'est mieux que l'aérien ou la route préserver cette précieuse énergie, vous n'avez pas profité du quoi qu'il en coûte, et des plans de relance, monsieur le Ministre, c'est ma première question, il manque environ un milliard d'euros par an au gestionnaire d'infrastructure pour envisager ce maillage équilibré du territoire 2ème temps de ma démonstration autour d'une petite victoire sénatoriale lors de la loi d'orientation des mobilités, nous avions obtenu un rapport de manière consensuelle sur l'avenir des trains d'équilibre du territoire et des trains de nuit grâce à la presse, merci Mobilettre nous l'avons obtenu il était rapidement validé par le ministère des Transports, cette étude est passionnante et démontre que dans cette étoile ferroviaire du TGV, il y a des besoins non satisfaits 5 grande transversale au niveau national, pourrait connaître des usagers, des besoins manifeste mais actuellement non plus de trains, il en est de même pour une dizaine de lignes de trains de nuit alors ma 2ème question Monsieur le Ministre, sur la mise en oeuvre de ce rapport, envisagez-vous de créer de nouvelles lignes d'équilibre du territoire, envisagez-vous de solliciter SNCF ou des opérateurs afin de les mettre en oeuvre, quelle stratégie pour acquérir le matériel et quel calendrier, je vous remercie. Merci, la parole est maintenant monsieur Joël Giraud, secrétaire d'État chargé de la ruralité pour 8 minutes maximum. Madame la présidente, monsieur le président de la. Commission aménagement du territoire et du développement durable, dames, messieurs les les rapporteurs, mais ces sénateurs Tabarot et Jacquet, mesdames, messieurs les sénateurs, je sais, vous le savez les, les, les Français sont attachés à un grand service public ferroviaire qui fait partie intégrante de leur Patrimoine national, le train à structurer le territoire jusqu'à ce que ce rôle soit concurrencé par celui des routes nationales, puis des autoroutes pour autant bénéficié d'une gare à proximité ou d'une liaison directe vers Paris reste dans l'imaginaire collectif, les outils qui sont indispensables à un maillage équilibré du territoire pour beaucoup de Français le train fait partie du quotidien qu'il en prenne tous les jours pour se rendre au travail plus plaisir que j'ai également pour rejoignent leur famille ou pour partir en vacances, plus que jamais, plébiscitée par nos concitoyens, le train est un outil puissant au service de la transition écologique et du désenclavement des territoires, le réseau ferroviaire souffrent de décennies de sous-investissements structurels en 2017, la moyenne d'âge du réseau a été de 30 ans, et les 3 quarts des petites lignes ferroviaires étaient menacées de fermeture ou de forts ralentissements entre 2018 et 2030, dès le début de ce quinquennat le gouvernement a souhaité redonner, au transport ferroviaire, ses lettres de noblesse cette stratégie que nous avons engagée répond à 3 objectifs : régénérer le réseau améliorer concrètement et les déplacements du quotidien et développer le fait ferroviaire et en fait accélérer la transition vers une mobilité propre pour tous, c'est une ambition qui s'est matérialisée par l'adoption du nouveau pacte ferroviaire pacte il y a pour objectif de donner un nouveau souffle à notre système ferroviaire en faisant de l'ouverture à la concurrence, une opportunité dynamisation du système en définissant également une nouvelle gouvernance permettant de clarifier les rôles de chacun et de positionner le gestionnaire d'infrastructure comme garant de la qualité du système ferroviaire en conduisant l'ensemble du système ferroviaire nationale à l'équilibre financier, avec une remise à niveau du réseau ferré, afin de répondre à à cet enjeu de maillage ferroviaire du territoire notre politique ferroviaire comprend 2 volets un volet investissement sans précédent pour régénérer l'ensemble du réseau ferroviaire et une nouvelle dynamique de développement des dessertes de voyageurs comme le comme du fret alors un investissement effectivement qui a été sans précédent pour régénérer l'ensemble du territoire du réseau ferroviaire puisque nous avons augmenté le budget de l'État pour le secteur ferroviaire de près de 60 16 7 milliards de dépenses sur la période 2013, 2017 contre 26,6 milliards d'euros sur la période 2018, 2022, l'État s'est également engagé à reprendre et les 35 milliards de dette de SNCF, réseau qui sont largement héritée de la construction des lignes à grande vitesse pour assainir sa situation financière et lui permettent de se concentrer sur sa mission de régénération du du réseau, il s'agit d'un d'un investissement qui est tout à fait inédit pour la régénération du réseau en moyenne 3 milliards d'euros par an sur 10 ans, soit plus de 50 % par rapport à la décennie précédente, en 2022 le soutien de l'État au transport ferroviaire se poursuit grâce à la mobilisation de 4,7 milliards qui sont alloués dans le cas du plan de relance et, en fait, nous sommes le gouvernement qui a triplé les investissements pour la mise en accessibilité du réseau pour les personnes à mobilité réduite alors cet investissement dans le réseau, il se traduit par une mobilisation inédite pour trouver une solution à l'obsolescence des petites lignes ces petites lignes irrigue l'ensemble du territoire national et sont à ce titre, essentiel pour faciliter les mobilités du quotidien et nos concitoyens et favoriser l'attractivité des territoires, nous avons fait de la régénération des lignes fines de desserte du territoire, une des priorités du quinquennat dès la remise du rapport sur l'avenir du transport ferroviaire par Jean-Cyril Spinetta, en février 2018, nous avons fait un choix très clair : l'avenir de ces lignes de desserte fine du territoire ne seraient pas décidées depuis Paris, c'est un véritable projet d'avenir que nous voulons bâtir pour les petites lignes ferroviaires à la croisée des chemins entre l'industrie, l'écologie et l'aménagement du territoire, nous avons donc mis en place un processus de décision concertée avec les territoires, et notamment avec les régions avec, après des décennies de sous investissement. Et nous avons engagé avec SNCF, réseau et les régions volontaires un plan de revitalisation des lignes de desserte fine du territoire 9 régions se sont déjà engagés dans cette démarche, preuve de l'intérêt pour les collectivités de de ce plan de revitalisation pour ne pas les citer la région Grand-Est Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire Sud Provence Alpes Côte-d Azur cher Philippe Tabarot Normandie Nouvelle-Aquitaine Occitanie Pays de Loire et France, ce sont 6000 kilomètres de lignes dans la pérennisation et désormais désormais sécurisé grâce à un investissement total de 5,2 milliards réunis sur 10 ans tous financeurs compris afin d'accélérer la mise en oeuvre et de de cette priorité du gouvernement l'État investit, vous l'avez cité tout à l'heure 300 millions d'euros pour accélérer les travaux les plus urgents, dans le cas du plan France relance le soutien public que vous pouvez trouver insuffisant en faveur des petites lignes, il n'a pour autant jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui, enfin l'assainissement financier du système ferroviaire permet à nouveau de de regarder vers l'avenir, le gouvernement a ainsi pu débloquer des projets de lignes nouvelles structurantes qui permettront non seulement qui permettront donc non seulement d'accélérer les liaisons entre Bordeaux et Toulouse, entre Marseille et Nice entre Montpellier et Perpignan, mais aussi d'améliorer les étoiles ferroviaire de ces villes, au service des transports du quotidien et des voyageurs, pour qui le train simplement indispensable pour venir travailler, il s'agit aussi d'assurer un maillage équilibré du territoire, qui passe par une dynamisation des services ferroviaires offert à nos citoyens certaines manqueront pas de déplorer le fait que les investissements dans le réseau que je viens d'évoquer ne portent pas leurs fruits ne sont pas visibles par les concitoyens le ferroviaire est une politique du temps long, où l'on récolte rarement sur un mandat le fruit des investissements faits ainsi le le transfert des petites lignes aux régions vise à leur permettent de développer une fois Céline rénové de nouveaux services au plus près des besoins des territoires, ça n'est certes pas encore tout à fait visible mais il fallait le faire dès maintenant pour voir un jour ses lignes redevenir des axes de développement, de l'ouverture à la concurrence des trains régionaux, la région sud a d'ores et déjà. De l'aube, suite à un appel dont un à un concurrent de la SNCF, Transdev Hauts-de-France Grand-Est, Pays de la Loire et vendredi dernier, c'est très récent en Bourgogne Franche-Comté on a annoncé qu'il lancerait prochainement des appels d'offres ces ces appels d'offres, ils vont permettent grâce à l'émulation entre opérateurs de faire bénéficier les voyageurs du. Une meilleure qualité de service et de plus de dessertes, nos 2 actions en faveur d'une amélioration des services se voit déjà concrètement, c'est la relance des trains Intercités de jour et de nuit, vous le savez, fait certainement, on vous le savent, j'y suis très attaché, j'étais d'ailleurs cette nuit dans le train de nuit Paris-Briançon avec 3 heures de retard, je dois le reconnaître : ce qui m'attend un petit peu désorganisée, l'emploi du temps, ce sont les trains de nuit et les trains Intercités de jour et de nuit, s'ils sont créateurs de Liens entre les territoires et les citoyens, ils sont écologiques, ils sont économiques, le train de nuit constitue une offre de transport adaptée aux enjeux d'aménagement du territoire et de transition écologique qui sont les nôtres, nous sommes le gouvernement qui a triplé le budget pour le renouvellement des trains d'équilibre du territoire, ce gouvernement a oeuvré comme aucun gouvernement ne l'a fait jusqu'à présent à la renaissance des trains de nuit, la réouverture de Paris-Nice en mai dernier du Paris-Tarbes-Lourdes rend décembre 21 21 également du Paris-Briançon le train de nuit Paris-Aurillac sera de retour d'ici à 2 ans pour réussir, réussir la la redynamisation des trains de nuit, le gouvernement a investi 100 millions d'euros dans le cas du plan de relance pour financer pour moitié la remise à niveau du matériel de nuit, de demain par le mariage, près de 10 lignes de train ni pourrait voir le jour d'ici 2030, le rapport du gouvernement remis au Parlement au printemps dernier, conformément aux engagements de la loi d'orientation des mobilités a permis de mettre en lumière plusieurs axes stratégiques, est de dégager des pistes pour trouver un modèle économique qui soit viable sur le long terme, je souhaite que le Parlement puisse se saisir de ce rapport et qu'un véritable débat puisse avoir lieu sur ce sujet, nous souhaitons également créer un véritable élan européen de relance des trains de nuit, l'ouverture du parisienne et du Paris Berlin d'ici respectivement décembre 21000 et 2023 enfin la la cohésion du territoire national, elle passe également par l'investissement dans la stratégie nationale ferroviaire comme j'arrive pratiquement à la à la fin de ce discours, je voulais vous vous dire également que nous avons parmi les objectifs importants, ceux de la PFUE, la présidence française de l'Union européenne, qui sera un temps fort pour notre pays, pour porter au niveau européen la décor The Nation, des transports, notamment l'accélération du report modal vers le faire, je vous remercie. Merci monsieur le ministre, nous allons maintenant aborder la suite du débat, je vous donne à règle du jeu, d'abord 2000, une question de minutes réplique comprise, système des questions au gouvernement du mercredi, vous connaissez ensuite la réponse du ministre : si vous n'avez pas utilisé les 2 minutes, vous pouvez répliquer ce après quoi le ministre peut répondre ou pour une minute ce après quoi vous pouvez encore répliqué pour une minute mais pas pendant 2000 peut répliquer en une minute.

Réponse et de nouveau réplique c'est le Sénat, que le dernier mot, voilà et ça commence par les 2 minutes si vous utilisez des 2 minutes dans la question, il y a juste la réponse du ministre. D'accord, après ça fait tomber l'éventuelle réplique suivante on vous allez voir, on va y arriver. Alors on commence avec monsieur Olivier Jacquin qui. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, en 2018 SNCF suspendait pour 5 ans les circulations de Nancy vers Lyon en TGV sur ligne classique en raison, nous avait-on dit de travaux en gare de Lyon, en compensation, 2 alternatives étaient mis en place une part Strasbourg. Et une par une liaison TGV directe Nancy Marne-la-Vallée, Lyon un tarif acceptable qui a été supprimé l'an dernier, sans autre forme de procès depuis le rapport sur les perspectives des trains d'équilibre du territoire fait la brillante démonstration qu'un besoin et des usagers existe entre le si on lorrain de Metz, Nancy, Dijon vers Lyon jusqu'à Grenoble alors qu'en est-il tout d'abord du rétablissement de cette liaison directe, les promesses de la SNCF seront-elles tenues. Deuxièmement, entendez-vous conventionnées avec la SNCF ou un opérateur pour instituer cet axe important comme une ligne d'équilibre du territoire et rétablir enfin ce service public, je vous remercie. Merci madame la présidente, oui, Monsieur le Sénateur Jacquin alors effectivement de nous des contextes généraux que vous connaissez bien le la loi d'orientation des mobilités il y a eu ce fameux rapport qui le rapport Philizot remis au Parlement en mai 1900 en 2021 et qui est relatif à l'étude sur le développement des nouvelles lignes de trains Intercités de jour et de nuit, c'est un rapport qui avait pour objectif, donc d'identifier au plus près les lignes THT qui permettrait de répondre aux besoins désenclavement des territoires les plus éloignés des grands axes de circulation. Moi, je, je veux, je tiens à souligner l'intérêt des nouvelles lignes de de très longues distances afin d'améliorer l'accessibilité des métropoles et des villes moyennes et je souhaite vraiment, je l'ai dit tout à l'heure mais j'insiste là-dessus, que la transmission de cette

il y a Toulouse Lyon il y a un Nantes, Rouen, Lille et des études complémentaires sont nécessaires pour définir précisément la la faisabilité technico-économique, il va falloir veiller aussi à la bonne articulation du du développement de ces lignes, avec le programme de régénération et de modernisation du du réseau ferroviaire

retour des services par par TGV bon pour autant en 2019, la fréquentation des services de terre fiction et était bonne, une centaine de personnes par par train pour autant la demande pour pour des trajets ferroviaires directes sur l'accident, si Lyon et au-delà, il existe, et cet axe a vraiment été identifiées dans le rapport que je viens de citer et il me semble important qu'effectivement nous puissions l'étude et de manière très précise et suivant la méthodologie que je viens d'exprimer qui plus générale sur les nouveaux sur les trains d'équilibre du territoire et lignes TGV. Alors Monsieur le ministre, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles, la mauvaise nouvelle, vous me dites clairement que SNCF aurait dit qu'elle n'envisageait pas de retour du TGV, or leur argument 1er c'est dès que le noeud lyonnais seraient désenclaver, hé bien ce service pourrait être rétabli, vous venez de m'affirmer, j'ai bien entendu que l'axe Nancy-Dijon avait plus vocation régionale donc TER, je ne l'entend pas du tout ainsi 2ème point vous me parlez du rapport Philizot, vous avez dû qu'on va confondre parce que le rapport Philizot, lui, on n'a jamais eu et la presse n'a jamais réussi à le faire chuter, on a eu un drôle de condensé de quelques pages n'était pas glorieux pour la communication et le respect du Parlement, alors je vous ai posé une question Monsieur le Ministre, vous m'avez confirmé qu'il avait bien 3 lignes de trains d'équilibre du territoire qui pourrait voir le jour, je vous ai demandé quelle était la méthode et le calendrier, vous me dites qu'il faut faire des études, ça ne me suffit pas. La parole est maintenant Monsieur Frédéric Marchand pour le groupe RDPI. Merci madame la présidente. Monsieur Jacquin, monsieur le ministre, fait ce qu'il veut de du voilà donc la parole est maintenant Monsieur Marchand. 2ème chance merci madame la présidente, monsieur le ministre, on a un état qui ne croit pas au réaménagement du territoire, nous nous allons sacrément investir 585 millions engagés pour la rénovation des trains 600 pour la sauvegarde des petites lignes 250 pour la modernisation des gares, voilà ce que déclarait le 27 janvier dernier le président de la région Hauts-de-France lors de la séance plénière du conseil régional, vous l'aurez compris évoquer le sujet de la politique ferroviaire et celui du maillage territorial équilibré dans ma belle région des Hauts-de-France est devenue, depuis plusieurs mois, chose impossible, pour nombre de raisons structurelles et conjoncturelles et d'une volonté politique manifeste d'hystériser un débat qui mériterait décidément mieux que le procès en sorcellerie fait de manière permanente à l'opérateur historique et à l'État accusé de tous les maux,

la situation que nous vivons aujourd'hui dans la région et le révélateur de ce qu'il ne faut pas faire, mais bien au contraire, la démonstration de la nécessité de travailler ensemble à la construction d'un vrai service public des mobilités ferroviaire au service des usagers du territoire le maillage territorial du territoire ne saurait se faire dans la méfiance et dans la défiance avec un opérateur montré constamment du doigt une région qui a souvent tendance à oublier bien vite qu'elle est celle qui a validé les orientations politiques de mobilité et un schéma de transport en lien avec les acteurs du territoire schéma transport remis en question au moindre Avatar la signature la semaine dernière du contrat de performance entre la région SNCF, réseau, c'est fait, vous le savez, dans la douleur et permet théoriquement en fin de graver dans le marbre les engagements des uns et des autres pour autant nombre de difficultés persistent et il faudra certainement encore du temps pour rétablir une situation qui permettent de travailler dans la sérénité et l'efficacité, monsieur le Ministre, dans une région comme celle des autres, France, la question des mobilités et du maillage ferroviaire des territoires et prioritaire ainsi le président de la République sera demain dans le bassin minier et se pose à nouveau la question d'une liaison directe ferroviaire entre la métropole lilloise et le bassin minier, permettant ainsi donner de nouveaux horizons un territoire qui a tant donné à la France, alors Monsieur le ministre ma question sera simple pouvez-vous me confirmer ici que l'État porte bien une vision et une envie ferroviaire pour notre territoire devenu aujourd'hui sur cette question, on a pas les mêmes policiers mortifère. Merci madame la présidente, oui, monsieur le sénateur, Frédéric Marchand, bien que, comme vous, très honnêtement je je déplore vraiment que la question essentielle de la mobilité dans les Hauts-de-France soient pris en otage, à quelques mois d'échéances électorales, présidentielles, je pense que Léo 30 méritent franchement mieux que ça, avant de servir aux intérêts politiques nationaux, je crois que la question des mobilités du maillage ferroviaire dans Valéo de France, c'est d'abord une question très concrète pour les concitoyens parce que ce n'est pas une question de le plateau TV mais franchement à une question du quotidien pour se rendre au travail vous rejoigne sa famille, voire pour partir en vacances, je me permettrai donc si vous me le permettez, monsieur le sénateur de de répondre avec précision à votre question : à la demande de la région Hauts-de-France une phase de concertation autour des évolutions de dessertes TGV a débuté avec la SNCF à partir de février 2019 compte tenu des enjeux que vous avez bien décrit le gouvernement a par ailleurs demandé à la SNCF d'élargir le travail amorcé avec la région à l'ensemble des collectivités qui sont concernés, l'évolution des dessertes TGV ne peut pas se faire en effet sans la compréhension de chacun des territoires dans l'ensemble, les discussions ont permis d'améliorer le niveau de desserte TGV de ces territoires. Et si l'oeuf de service a été fortement perturbé en 2020 et en 2021 par la crise sanitaire, l'enjeu principal à court terme, c'est désormais de remettre en place progressivement les offres nominales, telles qu'elles étaient prévues au service annuel 2021 pour les petites lignes le protocole qui a été signée avec la région prévoit 825 millions d'euros de travaux dont 330 millions financés par l'État et c'est la SNCF, réseau concernant les les difficultés sur le le TER Hauts-de-France nous avons bien conscience que celles-ci ont été très importante ces ces derniers mois et très pénalisante pour les, pour c'est un sujet qui est de la compétence de la région de l'auto qui est bien sûr l'autorité organisatrice, la SNCF nous a indiqué avoir mis en place un plan de redressement de la qualité et des points réguliers sont faits entre l'autorité organisatrice et la SNCF poursuive son avancement, j'espère que ces éléments vous rend vous vous permettent de répondre à cette question essentielle, qui effectivement ne doit pas relever d'une polémique stérile. Merci, la parole est maintenant Monsieur Pierre-Jean Vergnes ELN pour le groupe, les indépendants. Madame la présidente, monsieur le ministre, ma question, enfin je repose une question que j'avais posée il y a plusieurs mois sur la virgule, Roissy et le ministre m'avait répondu que les choses avancent et très bien sûr le barreau Roissy-Picardie, c'est vrai que les choses avancent bien, c'est une très bonne nouvelle, mais sauf que ce n'était pas exactement la même ligne, moi je vous parle d'un raccordement la loi si c'est un tronçon d'un peu plus d'un kilomètre qui permettrait de raccrocher Roissy à la ligne Paris-Villers-Cotterêts Soissons, Laon, Hirson, l'enjeu puisqu'on est dans le sujet du maillage territorial, il est extrêmement important dans un territoire difficile ça permet la mobilité de ceux qui habitent dans l'et qui irait travailler à Roissy, ça permet à ceux qui habitent sur le territoire de Roissy éventuellement de venir vivre sur des territoires sur j'ajoute que dans quelques mois, ouvrira Villers-Cotterêts la cité, comment la Cité de la francophonie où la langue française, qui représentera à l'intérêt touristique important et qu'il est également important que les touristes puissent de Roissy, venir, venir à Villers-Cotterêts, donc il y a une étude qui a été lancé il y a quelques quelques mois qui avait été acté dans le CPER entre l'État et la région, une étude prêt auprès opérationnel mené par SNCF réseau à hauteur de 150000 euros de de chaque côté, ce que je voulais savoir, Monsieur le Ministre, c'est ce que vous pouvez nous confirmer qu'SNCF réseau a avancé sur les études que les résultats, nous les aurons bien au mois de juin et réaffirmer ici la volonté de l'État d'aboutir sur un sujet ô combien structurant pour un territoire comme la haine oh combien au coeur d'un sujet qui est celui de l'aménagement du territoire et puisqu'on parlait d'autre France juste avant le conseil régional, lui, a affirmé les choses, ils étaient déjà prêts à financer à partir sur ce dossier, on attend autant de clarté de la part de l'État, merci. Si le ministre. Merci madame la présidente, oui, monsieur le sénateur, hé bien écoutez, effectivement je, je, je vais tenter de ne pas faire l'erreur de répondre sur le l'autre question qui qui est quand même extrêmement intéressant de, je dois dire pour pour pour votre territoire parce que là, l'amélioration de la desserte ferroviaire en entre l'aide et l'Île-de-France avec la réalisation du du nouveau barreau ferroviaire entre Paris-Laon et la ligne à grande vitesse d'interconnexion, elle mène quand même à l'aéroport de Roissy, c'est une revendication de vote. Territoire mais j'ai bien compris que votre votre question ne ne portait pas essentiellement sur ce sujet, bon pour pour réponde de manière précise sur l'attractivité du territoire axonais et la façon de de le développer, puisque c'est bien là je si je comprends bien votre votre préoccupation, l'État a décidé de financer en 2021, à hauteur de 150000 euros, une nouvelle étude fonctionnelle et technique, cette étude qui se poursuit à l'heure où je vous parle, va permettre d'alimenter les réflexions globales à conduire sur l'ensemble des opérations qui sont prévues sur le réseau Nord et en particulier au sein de de la plateforme, services et infrastructures qui réunit État, collectivités, SNCF, réseau alors le le financement et et le calendrier de la suite des études, ils vont pouvoir être abordée tout simplement dans un cadre qui est le cadre classique des négociations autour du volet mobilité 2023 2027 du contrat de le CPER Des Hauts-de-France en toute la rencontre des options qui ont été déjà retenue à l'issue de l'étude, financée en 2021, donc voilà, si vous me le permettez, monsieur, je pense que c'est, c'est ce qui recouvre l'objet de de votre question, ce sur quoi nous nous engageons pour les années qui viennent, sur le territoire qui vous intéresse.

Madame la présidente, monsieur le ministre, la période de crise sanitaire que nous traversons depuis 2 ans, a mis en avant de nouveaux modes de vie pour nos concitoyens, parmi ceux-là, le lieu d'habitation. Le marché de l'immobilier des villes moyennes, situées à 100 kilomètres de Paris, a été pris d'assaut pour autant ces nouveaux habitants ont conservé leur travail sur la capitale ou sa banlieue. L'idée a été proposé d'expérimenter des trains Directs entre les agglomérations situées dans un rayon de 100 kilomètres et Paris sur décision peu utilisé en dehors des horaires de pointe, ces villes de taille moyenne, forment un cercle autour de Paris et sont elles-mêmes au son d'une étoile ferroviaire leur propre département. La politique ferroviaire dont a besoin notre pays pour répondre aux nouveaux comportements passe non pas uniquement par la réouverture par la réouverture parfois utopique de toutes les petites lignes, mais par une optimisation des moyens déjà à disposition en cohérence avec les financements possibles, vous l'avez tout à l'heure, dit Monsieur le Ministre, l'on sait que le temps politique n'est pas le temps, ferroviaire, en 93, lancer la réflexion sur la réouverture de la ligne Chartres Orléans il aura fallu 27 ans pour réaliser un tronçon de 27 kilomètres entre Chartres et Voves, qui permet à l'Eure-et-Loir d'être rattaché à la capitale universitaire qui est tour sans parler des moyens financiers dont disposent des branches SNCF qui ne permettent absolument pas de rattraper le retard immense pris durant plusieurs décennies sur les réseaux, la ville de Chartres, dont je suis l'élu travaille par exemple à cette modernité depuis plusieurs années avec la région Centre Val de Loire, autorité organisatrice des transports et le groupe SNCF le vaste programme Polgar a permis la modernisation Express de l'outil de travail SNCF mais hélas largement financé par les collectivités territoriales

vous, vous le savez la crise sanitaire a déjà profondément rebattu les cartes du rapport au travail et par conséquent les les besoins également en termes de mobilité dans les entreprises et et les salariés sont adaptés avec de télétravail le recours visioconférences il y a quand même encore difficile de dire si l'évolution de ces comportements et durable et si elle va s'inscrire dans dans le temps, lorsque la crise ce sera derrière nous et pour continuer d'attirer les les usagers notre réseau ferroviaire va prendre en compte bien évidemment ces évolutions et que vous l'avez souligné le le temps ferroviaire n'est pas toujours le temps de constituer si j'que nos concitoyens et et des évolutions de de la société, alors pour répandre plus précisément à votre question en grande couronne parisienne, vous le savez, le besoin de desserte des villes intermédiaires est élevé au regard de la très forte densité de de population la capacité de l'infrastructure ferroviaire, elle est directement liée au différentiel de vitesse entre les très rapide et les circulations lente, notamment celles qui comportent des des arrêts multiples un très rapide et il est consommateur de de capacités ferroviaires dans dans les zones denses de circulation où figurent des trains qui comportent, eux, de leur côté, plusieurs arrêts les lignes entre entre Paris et ses villes de surcroît sont principalement de de la responsabilité des régions donc il leur revient de négocier et notamment de négocier avec Île-de-France mobilités l'insertion éventuelle de ces nouvelles dessertes je j'attire donc également votre attention que en région parisienne et il pourrait justement être difficile d'insérer des trains rapides dans un système ferroviaire qui est déjà relativement saturé, alors je crois que ces négociations et et permettez-moi de le dire, c'est ces rapports de France entre la région qui est la vôtre, mais également Île-de-France mobilités doivent exister pour essayer de voir dans quelle mesure on peut améliorer un quotidien dont je conçois qu'il soit difficile pour celles et ceux qui sont finalement habitant lointain et pour autant, travaillant dans la région parisienne. Je vous remercie, la parole est maintenant monsieur Guy Benarroche pour le groupe écologiste solidarité territoire. La présidente, chers collègues, nous le savons, le le ferroviaire est un outil incontournable de la transition écologique assurer un maillage équilibré dans chacun des territoires signifie pour l'État, se donner les moyens d'engager une véritable politique ferroviaire, or aujourd'hui votre politique globale des transports est loin d'être structuré et de parvenir à l'objectif ambitieux de part modale fixé par la loi climat et résilience certes votre gouvernement commence à répondre au manque d'investissement criant des dernières décennies, mais pas assez pour rattraper le retard et conforter l'attractivité du rail 2 3 milliards d'euros sur 3 ans, sont destinés à SNCF réseau mais les besoins estimés c'est l'avoir réalité à 3,5 milliards c'est des petites lignes à 700 millions parole encore les crédits alloués sont bien insuffisants, 310 millions vous savez que la poursuite des trajectoires actuelles entraînerait la condamnation de nombreuses lignes l'enclavement de territoire déjà isolé le réseau ferroviaire peinent à sortir de son état, dégradation, aucun modèle de financement n'a été défini pour sa modernisation loft de transport Lenny équilibrée ni structurée et un manque de transparence sur le fléchage des coups et notable n'a possibilité de transfert des petites lignes aux régions dans la loi 3DS sous couvert de les responsabilités risque de constituer un véritable fardeau pour elle alors qu'elle porte déjà la plus grande partie du coût du coût de renouvellement pensez-vous donc telle politique, assure un maillage équilibré du territoire, avez-vous vraiment actionner tous les leviers pour enfin, entamer une véritable réforme du système ferroviaire et lancé un plan d'investissements à la hauteur des enjeux. Merci madame la présidente, oui, monsieur le sénateur Ben, mesdames, messieurs les sénateurs, bon les. Les Liens entre les territoires et les citoyens sont souvent relatifs à la qualité des dessertes fines du territoire. Qui constitue vraiment une 9 de transport adapté aux enjeux d'aménagement des territoires et et de transition écologique qui sont les nôtres, auquel je, je, vous savez Monsieur le Sénateur, particulièrement attaché, mais je le suis aussi, tout en n'étant pas le le ministre en charge des Transports parce que nous avons déjà discuté de ces questions, nous avons 9000 kilomètres de petites îles françaises qui irriguent aujourd'hui nos territoires, ce gouvernement il a oeuvré comme aucun gouvernement auparavant, je le disais tout à l'heure en en dans mes propos limiteur liminaire, pardon à la renaissance de ces lignes, nous avons engagé en 2020 avec les régions, un plan de remise à niveau de de Séville lignes et de remise à plat de leur gouvernance en 2022 ne poursuivant cet effort massif, l'État va engager plus de 200 millions d'euros sur les petites lignes pour un bilan de plus de 550 millions d'euros sur la période 2020, 2022

ce travail 3 de de concertation avec les régions puisqu'il y a 9, protocole d'accord qui sont déjà signés ou qui sont adoptées par les assemblées régionales délibérante pour un montant de 5,8 milliards d'euros, concrètement, c'est la preuve que ces 7000 kilomètres de lignes qui 107000 et 9000 vont pouvoir être sauvés et je crois qu'il s'agit là effectivement d'une politique qui est une politique qui tranche considérablement si c'est avec ce qui s'est passé précédemment et qui correspond bien aux engagements qui étaient ceux à la fois du président de la République et du gouvernement de faire en sorte que leur ferroviaire redevienne une priorité, on peut toujours considérer qu'on peut faire plus, mais je dois dire que ce qui a été fait sous ce quinquennat et tout à fait remarquable par rapport aux autres périodes.

assurer une trajectoire de modernisation et d'innovation, avec une participation de l'État accrue aux investissements de régénération inclure des acteurs locaux, pour aboutir à une vision partagée du maillage territorial, sur le long terme, couvrir les territoires peu denses, autant que les territoires urbains, donner plus de moyens au fret et au transport combiné, garantir une concurrence saine entre les opérateurs, la France est encore bien loin de ce tableau, la coopérative ferroviaire Railcoop l'a très bien rappelé un maillage sur l'ensemble du territoire va requérir des aides de l'État, monsieur le Ministre, les effets d'annonce ne suffisent pas pour parvenir au part modale de 18 % pour le fret et de 17 % pour les voyageurs, il va falloir actionner davantage de mesures concrètes pour le rail. Merci, la parole est à monsieur Gérard Lahellec, du groupe communiste républicain citoyen écologiste. Vous avez la parole merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, bien qu'il soit prématuré de tirer un bilan de tous les bouleversements institutionnels intervenus depuis 2018 il y a quand même des faits qui pèse lourd et des tendances lourdes donc qui se dégage donc il convient de tirer tous les enseignements, premièrement le pacte ferroviaire qui devait conforter l'offre globale de desserte ferroviaire à l'échelle du pays, on ne peut pas dire que celui-ci est pour l'instant, produit ses effets, l'intervention de la concurrence sur les lignes TGV, on a eu l'illustration du Paris-Lyon, ceci montre bien qu'elle tend à s'exercer prioritairement sur les segments captifs, une telle concurrence, si elle devait s'exercer sur un territoire comme le mien, c'est-à-dire la Bretagne, hé bien s'exerceraient sur l'axe Paris-Rennes, se posent la question de qu'il emmènerait des trains jusqu'à Brest et Quimper, puisque plus on va loin, plus on va au bout, moins il y a de monde et moins ces captifs, enfin, le projet de loi 3 3D à se consacre en quelque sorte la partition des petites lignes ferroviaires restent divisés en 3 catégories, sachant que la dernière catégorie, si je puis dire et laisser à la charge des collectivités territoriales à 100 % donc, au fond, celles qui ont remis en état leurs lignes sont les bons élèves que l'on punit parce que de fait on leur laisse sa charge 100 % de la charge du reste à faire, enfin, je remarque aussi que les pertes de recettes qui ont été consécutive à la crise Covid elles n'ont été compensés d'aucune manière, c'est la SNCF et les régions qui ont trouvé des accords pour en assurer la charge et puis dans le cadre de la loi climat résilience ici même au Sénat, nous avons adopté des amendements qui était ambitieux pour le développement du ferroviaire, on en parle que trop peu à mon goût, donc, au fond, une seule question quelle ambition nourrit ce gouvernement pour préserver l'offre de services publics à l'échelle de l'ensemble du territoire. Moi si voulez la présidente, monsieur le sénateur Lahellec. Vous savez, dégradation du service endettement un déficit record, manque de compétitivité du réseau c'est c'est le triste résultat de décennies de sous-investissement on sait qu'on a fait en 2017, s'il n'était pas nouveau n'en était pas moins relativement amer, il faut bien le reconnaître, il est urgent de sauver le service public ferroviaire et c'est ce que nous avons fait dès le début du quinquennat avec la loi pour un nouveau pacte ferroviaire afin de transformer ce service public qui est essentiel pour le rendre plus performant et viable à long terme, alors l'objectif de cette réforme ben c'était ces améliorations pour tous pour les usagers des trains plus ponctuels, plus nombreux et plus sûr, avec des meilleurs services pour l'entreprise SNCF, tourné vers l'avenir compétitives aux finances assainies pour les cheminots, une vision claire de l'avenir de leur profession qui a beaucoup évolué pour des postes plus attractif, une vraie reconnaissance de leur rôle et pour le contribuable, tout simplement, c'est ce qui est important, une garantie que chaque Euro se dépensé le soit efficacement alors beaucoup de chemin a été fait depuis le lancement de cette réforme sur le social, la mise en place d'un cadre social harmonisé pour tous les salariés du ferroviaire, la constitution d'une branche professionnelle, la définition d'un sac à dos social pour les salariés qui seront transférés avec notamment la portabilité de leur régime de retraite, la création de d'une caisse de branches unique pour les salariés de la branche ferroviaire qui soit statutaires ou non, et pour les usagers, ben c'est l'arrivée de de Trenitalia qui a commencé son service Paris-Lyon Milan en décembre 2021 c'est l'émergence d'opérateurs comme dans du côté de l'économie sociale qui affiche l'ambition de desservir les territoires ruraux entre Lyon et Bordeaux, des à 22 ou puis d'assurer des liaisons entre Rennes et Toulouse, ou encore entre Thionville et et Lyon 23 il y a aujourd'hui une véritable appétence des opérateurs pour explorer tous les segments de marché, et pas seulement ceux considérés comme les plus rentables, c'est la meilleure preuve que le cadre d'ouverture à la concurrence que nous aurons mis en neuf fermé de de libérer les énergies et de susciter de nouveaux services au profit des voyageurs. Merci, la parole est maintenant madame Denise Saint-Pé pour le groupe Union centriste. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, le Sénat a souhaité débattre sur la politique ferroviaire menée par votre gouvernement, ce dont je me réjouis, tant les 5 années passées en bouleverser le secteur ferroviaire, en effet, si la loi pour un nouveau pacte ferroviaire et la plus longue grève de l'histoire de la SNCF à l'occasion de la tentative de réforme des retraites sont désormais derrière nous, la pandémie et l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire, sont toujours en cours, d'autres défis s'annoncent par ailleurs en matière de décarbonation des mobilités et d'aménagement du territoire, c'est pourquoi il est primordial de maintenir la qualité de notre réseau ferroviaire qui repose sur 3 piliers : un réseau à grande vitesse, un réseau structurant et les lignes de dessertes fines mais si je me réjouis que le plan de relance permettent aujourd'hui de renouer avec le développement de lignes à grande vitesse, je m'inquiète néanmoins que ces investissements ne remettent en question les objectifs de performance du réseau structurant, pourtant tout tout aussi nécessaire pour nos concitoyens, j'en veux pour illustration l'État et la fiabilité défaillant des caténaires dites midi sur les lignes du sud aquitain par exemple sur l'axe Dax, Pau qu'il faudrait remplacer par des infrastructures modernes aussi, pouvez-vous, Monsieur le Ministre, me rassurer quant à la volonté de l'État, de relancer la grande vitesse, sans porter préjudice à la modernisation du réseau structurant, je vous remercie, monsieur le ministre. Merci Vale la vraie oui madame la la sénatrice Denise Saint-Pé écoutez l'entretien et l'amélioration du réseau ferroviaire existant est une priorité sur le long terme pour le gouvernement, pour offrir une offre de qualité à l'ensemble des territoires, alors il est essentiel de, de trouver un juste équilibre où vous avez raison, entre les lignes à grande vitesse et et les lignes classiques, le développement des premières ne peut se faire au détriment des secondes, c'est cet équilibre que le gouvernement s'attache à trouver entre TGV et petites lignes régénération des trains jours relance des trains de nuit entre développement des, des lignes nationales et internationales, ce qui nous a, ce qui nous permettra d'assurer un maillage qui était un maillage équilibré du territoire pour reprendre le le titre exact d'ailleurs du débat qui nous occupe aujourd'hui, vous avez mentionné la la desserte ferroviaire de de la région paloise et je vous confirme que le gouvernement est très attentif aux études d'améliorations qui sont financés à parité par l'État et la région dans le cas du CPER 2015, 2020 de nouvelle Aquitaine à hauteur de 0,5 millions de ses études dans le rendu est attendu pour la fin du mois d'avril à 22 permettront d'identifier en concertation bien sûr avec les territoires, les modalités d'amélioration de la desserte de Pau grâce à l'optimisation des infrastructures existantes entre Dax et Pau, l'amélioration de de la desserte de peau peut également s'envisager à l'aune du du Grand projet ferroviaire ferroviaire du Sud-Ouest, le GPSO et de sa section de ligne nouvelle à grande vitesse à 350 kilomètres heure entre le sud Gironde et Dax c'est une section nouvelle qui va réduire le temps de parcours des des usagers de 20 minutes entre Bordeaux et Dax et, par extension, entre Paris et Pau, concrètement, ce sera 3 heures 50 au lieu de 4 heures 10 actuellement, c'est une section qui sera réalisé dans la continuité de la section Bordeaux-Toulouse, pour lequel le gouvernement a récemment confirmé l'engagement financier de l'État, je tiens à souligner que que la réalisation de cette nouvelle ligne n'est absolument pas contradictoire avec la rénovation et la modernisation du réseau existant puisque ce projet GPSO justement, il comprend des aménagements qui sont essentiels pour le bon fonctionnement des noeuds ferroviaires de Bordeaux et de Toulouse, qui vont permettent justement d'augmenter le nombre et d'augmenter surtout la fiabilité des circulations, ce qui est je crois un enjeu essentiel pour vous. Merci madame Saint-Pé Evry presse secondes. Merci madame la présidente, il est grand temps Monsieur le Ministre, que ce réseau sud aquitain soit amélioré et notamment les technologies de ces caténaires qui date quand même de 1937 il est grand temps de moderniser ses quatre madame, je vous remercie. Monsieur le ministre, c'est bon, nous passons maintenant Monsieur et rigole pour le groupe, du pu Rassemblement démocratique social et européen. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, en matière de politique ferroviaire : le gouvernement s'est positionné en faveur de la rénovation du réseau existant, d'ailleurs pris dans ce sens sur la ligne THT Clermont Paris pour les années à venir Line qui souffrent souvent de retard inacceptable mais je voudrais aborder aussi les petites filles du transport du quotidien, c'est-à-dire celle qui relie les métropoles intra-régional, il faut aujourd'hui plus de 2 heures 30 en train pour relier 2 métropole une même région Saint-Étienne et Clermont-Ferrand, c'est une heure de plus qu'en voiture, et pour cause : il est impossible d'effectuer ce trajet en train sans correspondance depuis 2007, les usagers se trouvent contraints d'utiliser l'autocar au plus naturellement leur voiture pour se rentrent de Clermont à Saint-Étienne dans un contexte de réchauffement climatique, vous conviendrez que la dynamique n'est pas la bonne 2016 c'est l'année de la fermeture du tronçon de cette ligne entre Thiers et bien sûr l'Union, rendant impossible la connexion entre les 2 métropoles en 2016, c'est aussi l'année de la création des grandes régions qui a vu, Clermont-Ferrand et Saint-Étienne relégué administrativement quand dans le même temps, elle se trouvait ferroviaire déconnecté. Lors de la suspension du tronçon de 48 kilomètres des travaux de régénération on est estimé autour de 50 millions d'euros, une étude de faisabilité a été lancé il y a quelques mois par la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont les conclusions, tarde à se faire connaître en réalité la région semble dans l'attente d'un engagement de l'État pour s'engager à son tour sur les dépenses d'une telle ampleur, les 2 tronçons restant clairement hier et bien Saint-Étienne sont assurées par les TER et c'est donc la région qui est l'autorité organisatrice, mais l'État ne peut se désengager de toutes ses lignes qui maillent notre région et rendent effectives les réformes administratives qu'elle a, qu'il a lui-même engendré, monsieur le ministre, nous sommes ici sur une voie qui renforce le maillage ferroviaire du territoire en reliant à la fois de métropole et plusieurs petites villes de zones rurales. Aussi, ma question est simple : le gouvernement entend-il s'engager sur ce dossier pour mettre un coup d'accélérateur à la régénération entendu de la ligne tiers. Merci madame la présidente, oui, monsieur le sénateur et rigole, vous avez commencé, vous, vos propos tout à l'heure en en saluant le les les programmes de régénération de de la ligne Paris-Clermont-Ferrand qui est un programme extrêmement ambitieux de 160 millions d'euros sur une ligne que je connais bien, par ailleurs, et donc je je. Connaît les quelques difficultés pour avoir de temps en temps cru que j'étais dans un train de nuit alors que j'étais dans un train de jour, mais vous m'interrogez plus spécialement sur la section went tiers en fait qui constitue la la partie centrale de la ligne, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne qui est classé en petites lignes ferroviaires jusqu'à Saint-Just, à l'approche de la l'agglomération de Saint-Étienne, cette section qui est, qui est la plus montagneuse, elle fait l'objet d'une suspension des circulation depuis 2016 et un service de substitution par autocar a donc été mis en place l'accord pour la relance du ferroviaire en Auvergne qui a signé le 5 octobre 2020, le président du conseil régional, avec le 1er sur la période 20 22 n'a en effet prévu aucun investissement sur la section went le président de la région Auvergne Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé en février 2021, le lancement d'une étude pour expertiser les besoins et envisager une réhabilitation à un coût moins élevé que celui estimé jusqu'à présent, c'est en effet à la région qui est l'autorité organisatrice des des transports en en la matière, de définir les modalités de service envisageables sur ce tronçon qui inclut le recours à des choix qui sont des choix technologiques innovants alternatif au au ferroviaire lourd et si un projet viable venaient à émerger, soyez assuré, monsieur le sénateur, que l'État est vraiment prêt à accompagner les acteurs territoriaux dans dans cette démarche par ailleurs les résultats de cette étude permettront d'alimenter les discussions relatives à l'élaboration du protocole d'accord État-Région sur l'avenir des petites lignes ferroviaires qui est en cours de négociation entre l'État, donc à la région Auvergne-Rhône-Alpes mais soyez assuré que si la décision est prise ainsi et que si la région suit la volonté qui est exprimé par les habitants, l'État sera au rendez-vous. Monsieur Gold 5 secondes. Sur la petite île, Monsieur le Ministre, quelle que soit l'autorité organisatrice de la mobilité, mais il faut une impulsion forte de l'État, aujourd'hui il n'y a pas de visibilité sur ce projet, sur cette ligne. le dérèglement climatique est un voyage sans retour le volet transport contribue très largement aux émissions de gaz à effet de serre le ferroviaire constitue un levier important de progrès, il fait indéniablement partie de la solution, c'est pourquoi nous devons permettre à tous nos concitoyens d'accéder à ce mode de transport vertueux tant au quotidien que pour partir en vacances, je tiens à vous alerter sur les inquiétudes des Lotois concernant la ligne Polt Paris-Orléans, Limoges, Toulouse, en effet, il semblerait que les arrêts dans le Lot, ne soit pas sanctuariser et que certains trains s'arrêteront à Brive, privant mon département de desserte, or cette ligne est essentielle pour le Lot, surtout dans le Nord, située à une heure 30 de Cahors, où les habitants ne sont pas concernés par la future ligne TGV Toulouse-Bordeaux : nous ne comprendrions pas d'être abandonné parce que ruraux, gagner la bataille du climat, c'est être volontariste, beaucoup plus qu'aujourd'hui, en matière ferroviaire, c'est reconquérir des usagers, lassés, qui se sont détournés par manque d'opportunités d'arrêt de tarifs adaptés et de commodités diverses, le changement de nos habitudes et si important à réaliser qu'il nous faut une stratégie non seulement robuste mais très fortement incitative, l'ouverture à la concurrence ouvrent de nouvelles perspectives, une société coopérative à but non lucratif, dans mon département, que vous avez cité Railcoop s'inscrit d'emblée dans une complémentarité avec la SNCF sur des lignes qu'on va dire plutôt délaissé mais quel soutien lorsqu'elles rencontrent des freins alors qu'elle propose des offres plus qu'intéressante pour le fret et les trains de nuit, le défi est immense, un choc de l'offre s'impose le volontarisme de façade n'a plus sa place, ouvrir une ligne fermée il y a peu, n'est ni une victoire ni suffisant, quelle sera votre stratégie pour donner toute sa place au ferroviaire pour tous usager et nouveaux acteurs, Merci madame oui madame la sénatrice, vous évoquez de sujets vous évoquez à la fois. L'axe structurant Paris-Orléans, Limoges, Toulouse, qui est, qui est un axe sur lequel des travaux de régénération représente une enveloppe de 1,6 milliard d'euros financé par SNCF réseau pour des opérations commencées en 2015 prévu jusqu'en 2025, ce qui crée effectivement des des désagréments et qui concerne les voies, les ouvrages d'art, les caténaires et qui va garantir à l'horizon 2025, des performances importantes pour cette ligne, alors il y a des travaux de modernisation qui sont en plus réalisé en complément soyez, soyez sûrs d'une chose c'est que en plus il le matériel roulant, va être à l'horizon 2026 me paraît matériel plus rapide qui est matériel plus confortable, il avait l'État investit pour cela 800 millions d'euros, dont 450 pour Paris Limoges Toulouse

qui sera mis en oeuvre en 2026 telle qu'il a été négocié, il y a 2 ans, vous n'avez pas donc d'inquiétude particulière sur un sujet effectivement que je citais tout à l'heure qu'il est le le sujet qui est franchement une initiative inédite en France qui réunit sous la forme de CIC : plus de 11000 sociétaires, ce qui est ce qui est la preuve d'une d'une prise en compte collective et citoyenne, j'allais dire de de ce sujet avec en plus quelques personnes morales 180 entreprises, pour être clair, qui sont, qui sont concernés et des entreprises publiques également, en décembre 21 à la suite de saisine de plusieurs régions, l'ART a donné son autorisation à Railcoop pour l'exportation aussi d'autres lignes, donc le gouvernement est intervenu auprès de la SNCF afin de faciliter l'arrivée de la concurrence sur le réseau ferré national a-t-il personnel, j'ai organisé, y compris des réunions avec la Caisse des dépôts a conscience désignation pour que nous arrivions

nouvelle que nous avons vraiment soutenu Madame la sénatrice otite du secrétariat d'État. Madame prévu l'ivresse 10 secondes merci monsieur le ministre, donc. Merci pour votre réponse, mais on attend toujours que l'État soit au rendez-vous, et notamment en termes d'investissements, les belles annonces qui sont des voeux pieux laisse

Merci madame la présidente, monsieur le ministre, les lignes de desserte fine du territoire, souvent appelée petites lignes représentent environ un tiers du réseau ferroviaire français, elles accueillent 17 % du trafic de trains régionaux et constituent souvent des moyens de déplacement pour les habitants des territoires ruraux et les villes moyennes en 2018 le rapport le rapport Spinetta préconisé la fermeture de 200 petites lignes ferroviaires fortement déficitaire, ceci après des décennies de sous investissement, l'État ayant privilégié, c'était normal, la rénovation des lignes à grande vitesse et la maintenance des TER urbain et et des réseaux, ce qu'il a été moins évident, l'État a depuis promis de remettre en marche les petites lignes souvent fermé ou remplacé par des bus toutes ces lignes jusqu'ici exploitée par la SNCF, mais sur la responsabilité des régions comme le rap rappeler certains collègues tout de suite, le gouvernement souhaite ainsi investir plus de 7 milliards d'euros sur 10 ans pour sauvegarder certaines lignes, mais il laisse aux régions, le choix de prendre en charge la rénovation des lignes traversant des territoires moins denses, combien cela va-t-il coûter aux régions et donc aux contribuables, alors que vous avez déjà effacé 35 milliards d'euros de dettes contractées par SNCF réseau si certaines régions ne veulent pas ré-exploiter certaines petites lignes parce qu'elle préfère privilégier le bus, d'autres sont attachés au maintien, voire à la récupération d'un Patrimoine de voies ferroviaires évidemment toutes les régions n'ont pas les mêmes moyens pour développer ces plans, mais la plupart ont une stratégie de reconquête ferroviaire ne peut-on pas trouver une alternative en exploitant le réseau ferroviaire avec des enjeux de transition écologique d'aménagement du territoire et de soutenabilité économique je pense particulièrement à Taxi Rail une société bretonne installée dans les Côtes d'Armor qui vient de finaliser la version fret d'un train autonome pour passagers qu'elle a conçu dès 2017 et qui sera mis en service en 2025, ce type de train sans chauffeur peut très certainement sauver certaines petites lignes ferroviaires déficitaires, grâce à un coût de fonctionnement considérablement réduit, alors évidemment restera le problème de la réhabilitation des voies souvent très détériorée.

3 milliards d'euros par an, moi pour moi ce n'est pas un investissement à perte, une fois celui-ci rénové, il va être possible de faire circuler plus de trains avec une fiabilité accrue aussi le ferroviaire va retrouver une nouvelle attractivité permettra puisqu'aujourd'hui de constituer une véritable alternative à l'usage de la voiture sur de nombreux axes vous savez pour avoir connu les trains de nuit, à l'époque où on pouvait réserver ses couchettes que la veille pour le lendemain, il était évident qu'après on vous disait qu'il n'y avait que 5 voyageurs dans train, c'est-à-dire les 5 initiés qui connaissait la rue il faut réserver la veille pour le lendemain et dont, dont les usagers habitués dont je faisais partie, sa vie, quelles étaient les les méthodes, je crois vraiment qu'il va y avoir une véritable alternative à l'usage de la voiture sur de nombreux axes et à l'heure où nous interrogeons sur des situations qui nous interrogions sur des situé à solutions qui permettent de diminuer la part des transports dans les émissions de CO2, je crois que la valorisation du réseau excite hésitant est un atout qui est tout à fait considérables, y compris d'ailleurs avec des innovations que vous citez, vous citez taxi mais il y en a d'autres et il y a des innovations qui sont bien entendu à prendre en compte, c'est ce que je disais tout à l'heure sur des problématiques comme la ligne que citer de notre collègue, votre collègue pendant Gold concernant la ligne Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, alors c'est dans cet esprit que le gouvernement a fait réaliser une étude sur le redéploiement des réseaux de trains Intercités de jour et de nuit, cette étude qui doit être complétée par des approfondissements bien évidemment sur le mode de financement des très nécessaire à l'équilibre économique potentielle des dessertes envisagées met l'accent sur l'effet réseau qui est nécessaire pour attirer une nouvelle clientèle sur ces lignes, le fait, nous en parlions avec la sénatrice Réville tout à l'heure que la coopérative Railcoop envisage de développer sur ses lignes, un certain nombre de dessertes contre bien qu'avec un nouveau modèle économique, l'exploitation, il est possible de développer de nouveaux la desserte de certaines lignes, qui avait été. ministre-maire. Si. La parole est au président nos jours. Oui merci madame la présidente, monsieur le ministre, parler de politique ferroviaire aujourd'hui nous amène à dresser un bilan et le bilan est clair, selon leur territoire, nos concitoyens ne sont pas égaux face à la mobilité ferroviaire, je peux vous dire indique mon collègue demi-auquel je souhaite un prompt rétablissement, que l'année 2021 a été particulièrement difficile pour les voyageurs TER dès août Des Hauts-de-France, notre région est en dernière place du classement de régularité, les plaintes pour retards, annulations et dysfonctionnements ne cessent de se multiplier, la SNCF a déployé un plan d'urgence fin octobre mais les aléas ont continué à perturber le trafic, les bonnes résolutions ne suffiront pas, j'ai alerté le président de la SNCF à ce sujet le 15 décembre dernier lors de son audition devant notre commission d'aménagement du territoire, il est urgent de réagir, cela concerne près de 200000 voyageurs par jour, assurer un maillage équilibré, c'est d'abord assurer la régularité des lignes existantes, répondre aux besoins de mobilité de nos concitoyens au quotidien, nous pouvons comprendre les difficultés liées à la crise sanitaire ou les problèmes ponctuels liés aux intempéries, mais pas que ces problèmes soient systématiques au point de faire des Hauts-de-France, la Moselle, le mauvais élève récurrent des classes de régularité, monsieur le Ministre, nous souhaitons une politique ferroviaire venant répondent aux fractures et au sentiment d'injustice que vivent beaucoup de nos concitoyens qui peine dans leur transport que quotidien quelles mesures vont être prises pour répondre à cette Hi-Fi ces difficultés dans nos territoires, je vous remercie pour la réponse qu'on ne manquerait pas d'apporter à mon collègue demi-. Monsieur le ministre. Merci à la présidente oui Monsieur le Monsieur le Président, permettez-moi de de me joindre aux voeux de rétablissement pour le sénateur, Stéphane Demilly et j'allais dire, mon ex-collègue de l'Assemblée nationale, d'abord, soyez assuré et que Stéphane Demilly soient rassurés, également, le gouvernement est vraiment très soucieux de la qualité des services ferroviaires TER dans la région des Hauts-de-France, les TER de cette région, il représente 1250 francs et 200000 voyageurs par jour, c'est tout à fait considérable, alors j'ai forcément eu une pensée pour les, pour les usagers qui connaissent des difficultés pour aller pour aller au travail le matin pour rentrer chez eux le soir je souligne qu'en l'état, en application du principe de libre administration des collectivités territoriales, on n'intervient pas dans la dans l'organisation des services TER qui relève uniquement de la compétence du conseil régional, dit dans le suivi de leur exploitation par SNCF voyageurs depuis septembre, les TER de le de l'Oise et plus généralement des Des Hauts-de-France ont connu des difficultés de de production qui ont engendré d'une régularité très dégradée des trains supprimés, vous l'avez dit, il s'agit d'une part de de causes externes à l'entreprise, qui ont d'ailleurs augmenté de 30 % depuis septembre, tels que des des bagages oubliés des accidents de personnes Des heurts avec notamment des des animaux et puis des des problèmes évidemment également de d'indisponibilité de rames endommagées ou de personnel, faute de formation, retardée par la crise sanitaire et des difficultés de de recrutement alors grâce au plan d'action que. Elle a présenté en octobre dernier à la région SNCF présente des résultats en nette amélioration, notamment au niveau des trains supprimés, c'est une dynamique qui doit se poursuivent grâce à un complément d'agents roulants une homogénéisation du parc et une réindustrialisation de de la maintenance, la SNCF va également proposer un plan de qualité et un travail précis sur 9 lignes en s'engageant à baisser le taux de trains supprimés à 3 % au lieu de 8 et demi % observée aujourd'hui, la SNCF a d'ailleurs donné sans son accord de principe pour effectuer les remboursements des des abonnements aux usagers et un effort va être effectuée pour améliorer la communication et l'information des usagers en cas de retard ou de suppression, je crois qu'il est essentiel que qu'un dialogue constructif puisse se poursuivent entre la SNCF, si Monsieur pour résoudre ses difficultés. La parole est maintenant à monsieur Gillet pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. avant le mois d'avril 2022, le gouvernement sera amené à prendre une ordonnance créant la société publique de financements pour lancer des appels d'offres ou du GPSO Grands projets du Sud-Ouest, la relance de la LGV Bordeaux-Toulouse par le 1er ministre il y a quelques mois, s'inscrit dans un calendrier présidentiel qui n'échappera à personne 4 milliards d'euros sont donc promis, sous réserve de l'engagement de l'ensemble des collectivités concernées en imposant d'englober Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax ces dernières en délibéré, une majorité d'entre elles, avec les 2 régions ont acté leur participation mais il manque encore 340 millions d'euros bruts à l'appel d'autres incertitudes perdurent, notamment sur le financement européen attendu à hauteur de 20 monsieur le Ministre, le gouvernement est-il en mesure de prendre l'ordonnance citée avant le mois d'avril est-elle d'ores et déjà transmise au Conseil d'État, où en sont les négociations avec l'Europe pour obtenir les 20 % de financement attendus qui imposeront la liaison vers l'Espagne, quel est le calendrier qu'envisagez-vous pour le franchissement de la frontière espagnole et le passage au Pays basque, compte tenu de ces interrogations financières et techniques, pensez-vous que le Conseil d'État donnera in fine et un avis favorable à ce projet et sur la maquette financière: confirmez-vous le lancement des travaux en 2024 et avez-vous une date pour la signature de l'ordonnance et enfin comment concilier le maintien et le développement des petites lignes et des lignes d'équilibre du territoire avec de tels investissements, plus de 14 milliards d'euros, je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci la présidente, alors je n'ai pas monsieur le sénateur, réponse à tous les éléments de, de, de votre question, pour autant, ce que je peux vous affirmer d'abord c'est que vous avez une inquiétude sur le financement, vous avez cité un manque de 340 millions d'euros et la région Nouvelle-Aquitaine c'est parfaitement engagée à compléter le financement pour la part que les collectivités territoriales n'apporterait pas au final, donc nous avons déjà c'est cet engagement au-delà, vous me posez la question de de l'ordonnance et de la saisine du Conseil d'État, le Conseil d'État est saisi aujourd'hui alors, vous me permettrez de ne pas faire de commentaires sur la façon dont le Conseil d'État vient bien évidemment analyser la situation, il lui appartient et à lui seul d'avoir un avis sur sur l'ensemble juridique et financier que constitue la saisine, qui a été la sienne au travers de de cette ordonnance au-delà, c'est un peu la la même question que celle qui avait été posée tout à l'heure, moi je crois qu'il y a un subtil équilibre à trouver entre des lignes qui sont des lignes à grande vitesse et des lignes qui sont des lignes, on va dire, on va dire d'aménagement du territoire, des lignes de desserte plus fine régional c'est c'est tout l'enjeu de l'ensemble de ces contrats que nous signons avec Once avec les différentes régions de façon à ce que nous soyons pas d'un côté, obligés, obligés de de faire en sorte que nous soyons de mer entre guillemets, dépossédé de moyens pour pour ne plus financer finalement de ce qui, sur le vrai de de l'intérêt régional et de l'intérêt locale nous y arrivons, jusqu'à présent, nous y arriverons sur ce projet de GPSO je sais. Monsieur Monsieur Gillet ivresse 24 secondes. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, vous m'apprenez que le conseil régional s'est vraiment engagé à cofinancer à financer les 340 millions brut manquant, je n'ai pas vraiment entendu cette information là mais je ne je la vérifierai mais elle est publique maintenant, nous verrons bien, en tout état de cause ou portée par l'ensemble des informations nécessaires et je le regrette parce que dans le cas de ce débat, c'eût été nécessaire un débat qui est souvent un monologue d'ailleurs, je le regrette. La parole est maintenant, monsieur le Ministre. Excusez-moi, j'avais pris de mauvaises habitudes, non mais c'est simplement madame la présidente, pour vous dire que, il y a une une solution sur veut des détails techniques sur un débat comme celui-là qui me semble extrêmement intéressant, il y a une solution, ce qui est de faire connaître la question précise parce que je, personne ne peut, au gouvernement, être omniscient et avoir une réponse sur les moindres détails d'un projet ferroviaire, quel qu'il soit. Monsieur le ministre, j'ai indiqué donc auprès du ministère, le thème du sujet quand on y regarde un peu plus près, il ne faut pas être grand clerc pour savoir toutes les questions qui se posent autour de la mise en oeuvre effectivement de ces 2 axes Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax donc très honnêtement votre réponse me semble insuffisante par rapport à la nature des débats qui sont posés aujourd'hui sur ces sujets-là. Par ailleurs, vous me confirmez bien qu'il y a bien 2 axes Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax parce que jusqu'à maintenant, le 1er ministre s'est exprimé surtout sur Bordeaux, Toulouse. 4 milliards d'euros qui sont sur Bordeaux, Toulouse, donc il va falloir que l'État apporte aussi un complément financier sur Bordeaux-Dax et là j'aimerais bien avoir une confirmation de l'engagement complémentaire financier sur Bordeaux-Dax parce que l'ensemble des parties prenantes attendent vivement cette réponse. Si la parole est maintenant Monsieur Rémy Pointereau pour le groupe Les Républicains. Oui merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues politique ferroviaire et maillage équilibré du territoire devrait tout de se retrouver dans le même sens lexical malheureusement pour bon nombre de territoires, notamment ruraux, c'est loin d'être le cas, je suis élu d'un département qui attend impatiemment le ce maillage équilibré, lequel du permettrait de sortir d'un enclavement qui plombe notre démographie notre tissu social et économique, plus concrètement, je souhaite vous interroger sur l'avenir des lignes du quotidien que l'on appelle aussi ligne de desserte fine sur lesquels l'État n'a pas tenu son rôle d'aménageur du territoire quelques exemples 1er lieu et il est, il y a la ligne Polt cette ligne historique et la colonne vertébrale des territoires du sud de la région Centre, sur cette ligne historique dans les années 60 le Capitole rouler à plus de 160 kilomètres heure aujourd'hui la vitesse moyenne des plus que de 120 kilomètres heure, voire moins, beaucoup d'annonces ont été faites concernant cette ligne, mais les travaux n'avancent pas, où en sommes-nous, ensuite il y a, il y a la ligne Bourges Montluçon, c'est une ligne en déshérence et je pèse mes mots, et pourtant c'est la ligne par excellence de rabattement des voyageurs des territoires ruraux, qui vont du nord de l'Allier vers Bourges et vers Paris, elle est en situation de spirale infernale, le mauvais état oblige, moins de vitesse, donc beaucoup de retard, donc moins de voyageurs, donc moins d'desserte conséquence la SNCF ne voit pas l'intérêt d'augmenter le nombre de dessertes et d'investir plus rapidement dans la modernisation de cette ligne, ce qui oblige la mise en place de bus pour aller de Montluçon à Saint-Amand-Montrond, puis à Vierzon, par voie d'autoroute, bravo pour la décarbonation. L'État envisage-t-il d'agir enfin sur cette ligne fine, elle est la clé de du maillage équilibré de nos territoires.

et dans la régénération sera prise en charge à 100 % par SNCF réseau à partir de 2024 et elle est vraiment, je connais son intérêt pour ce territoire que je connais particulièrement bien, elle est vraiment symbolique de la mise en oeuvre est justement du plan de revitalisation des petites lignes ferroviaires qui est lancée par le gouvernement depuis février 2020 avec la signature d'un protocole d'accord entre l'État et la région Centre Val de Loire qui définit la stratégie d'investissements pour les 10 ans à venir. à fin 2022 leur l'État aura mis en place 66 millions d'autorisations d'engagement sur les petites lignes Centre-Val-de-Loire pour la période 20 22 soit 100 % de ses engagements pris dans le cas de l'avenant au CPER du 8 juillet 2020 en particulier l'État à financer des investissements de régénération de la Bourges Montluçon en Centre Val de Loire, à hauteur de 91,5 % conformément à ses engagements, soit plus de 26 millions d'euros pour des travaux à réaliser en 23 le complément de 8 et demi % étant apporté par SNCF réseau donc la la poursuite de ce programme de régénération par SNCF réseau a compté 2000 2024 permettent de maintenir les infrastructures de la ligne à niveau et avec elle, bien évidemment, la qualité des dessertes ferroviaires que vous appelez de vos voeux et je le comprends parfaitement pour connaître cette région qui a des problèmes d'enclavement sérieux quant à l'axe structurant par Lorient, Limoges, Toulouse Polt, il fait l'objet de travaux gérer génération qui présente une enveloppe de 1,6 milliards d'euros, qui est financé par SNCF réseau pour des opérations commencées en 2015 prévu ce en 25, cette opération concerne les ouvrages d'art, les caténaires et vous garantir des performances d'infrastructures à horizon 2025 les travaux de modernisation sont réalisés en complément, ces travaux s'élève à un montant de 385 millions d'euros dans les 2 tiers sont déjà financés par l'État, les régions desservies tant sollicité sur le dernier tiers, et enfin le matériel roulant, va être remplacé à l'horizon 2026 pour un matériel 9, plus rapides et plus confortables, l'État investit pour cela 800 millions d'euros, dont 450 pour la ligne Polt la ligne Paris-Match. Merci, la parole est maintenant à Jean-Claude pour le groupe Les Républicains. Monsieur le ministre, monsieur le président, mes chers collègues à l'Occitanie en Aveyron, en particulier l'État vient de signer 2 protocoles d'accord de financement avec plusieurs collectivités territoriales le 1er pour la ligne à grande vitesse, Montpellier, Perpignan en 2040 secondes pour 15 lignes de desserte fine du territoire dont Brive-Rodez et Teissonnière Rodez certainement pour l'horizon 2030, il est heureux également que la ligne de nuit Rodez Paris ne soit pas fermée mais ces constats positifs ne doivent pas masquer l'autre partie de la réalité, en effet, le train de nuit Rodez Paris est symptomatique de l'état du réseau ferroviaire en France hors ligne à grande vitesse, évidemment, et plusieurs collègues l'ont soulevé premièrement, les travaux pour cette ligne s'éternise et cause de dysfonctionnement qui irrite les usagers, deuxièmement les trains souffrent de l'absence de modernisation pour le confort des passagers comme nombre de nos concitoyens, je déplore la lenteur des animaux, des améliorations sur le terrain, par ailleurs, Monsieur le ministre, nous tenions à vous féliciter pour la rapidité de la mise en oeuvre du train de nuit Paris- Berlin qui roulera à partir de la fin 2023 mais ailleurs en France, dans les gares desservies par les petites lignes la ou les machines automatiques ont remplacé les agents de la SNCF, les usagers devront attendre une dizaine d'années afin de voir avant de voir l'amélioration des lignes une politique ferroviaire ciblée sur les petites lignes aurait entraîné leur modernisation rapide, d'autant que les problèmes étaient connu, à l'inverse, vous avez engagé tardivement des rénovations à tous les niveaux, à un horizon aussi lointain que la cohérence poursuivi est introuvable, toutefois, monsieur le ministre, en prenant le lait pour exemple l'Aveyron, pouvez-vous essayer de nous montrer que votre politique ferroviaire s'est intéressé aux petites lignes locales Berlin c'est bien mais Rodez, c'est bien aussi. Monsieur le Ministre. Merci madame la présidente, mais, Monsieur le Sénateur, Angela je des déjà je pense que vous avez raison, Rodez, c'est bien aussi. Puis-je me permettre également de faire une petite incidente, parce que je dois être le seul membre du gouvernement, être allé en voyage officiel dans l'Aveyron, en utilisant le train de nuit Paris-Rodez voilà c'est c'est un peu une gageure parce qu'il y avait un dysfonctionnement du du chauffage, il faisait trop chaud mais mais mis à part ça, je tenais à le faire parce que j'ai un certain militantisme dans les trains de nuit, vous le savez, alors le protocole d'accord que vous citez, avec la région Aquitaine que le 1er ministre a signé la semaine dernière, concerne 16 petites lignes et un investissement de 774 millions d'euros, c'est un investissement qui est inédit en faveur des des petites lignes de la région, malheureusement, ce serait trop sème ça n'efface pas par un coup de baguette magique des décennies de sous-investissement chronique alors dans le cas de France relance on a engagé au total 300 millions d'euros pour accélérer les travaux les plus urgents, combler le retard accumulé concernant la régénération du réseau concernant les dysfonctionnements que vous évoquez, sur la ligne de train de nuit Paris-Rodez, ils sont de plusieurs ordres : ils sont en partie liées aux conditions météorologiques, mais aussi à certaines difficultés qui sont liées à la situation sanitaire, notamment pour la présence des agents ayant pris ce train comme je vous l'ai dit et comme vous le savez, j'avais fait remonter également la difficulté que nous avions eu à réserver ce qui peut aussi être une cause de dysfonctionnement un peu particulière et je crois que depuis les choses se sont bien améliorées, parce que l'exaspération des usagers était légitime, on y est vraiment très attentifs et les services du ministère des Transports font désormais le point régulièrement avec la SNCF sur ce dossier sur lequel je vous le garantis, nous sommes très vigilants Paris-Berlin est une autre affaire. La parole est maintenant Monsieur Jean-Marc Boyer pour le groupe des Républicains. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, les Auvergnats sont exaspérés de plus en plus face à l'isolement ferroviaire croissant de nos territoires de l'Auvergne et du Puy-de-Dôme, il y a bientôt 5 ans Madame Élisabeth Borne, ministre des Transports nous avait fait des promesses d'amélioration substantielle de nos mobilité et de la ligne de train Paris-Clermont-Ferrand les dysfonctionnements récurrents et intolérable de la ligne devaient être résorbés, elle devait être plus rapide, or la situation n'a pas évolué à la hauteur des attentes du territoire et de ses habitants et de ses forces vives et vous venez de souligner tout à l'heure monsieur le Ministre des travaux de sécurisation et de modernisation de la ligne sont certes en cours toutefois ce à prévoit pour 2028 ne sont pas financés et le gain de temps de trajet sera minime, c'est pourquoi, comme l'a suggéré le vice-président aux transports du conseil régional Auvergne Rhône Alpes il apparaît absolument indispensable de reprendre, étude de la ligne grande vitesse LGV Paris-Orléans, Clermont-Ferrand, Lyon, dites POCL, telle que cela avait été acté par Madame Borne enfin désenclaver durablement à moyen et à long terme, l'Auvergne et le Massif Central, les progrès techniques sur les voies et les rames ont réduit les temps de trajet depuis les années 50 en effet, le rétrécissement de la France par le train à grande vitesse, démontre que, durant les 60 dernières années les les 10 plus grandes villes françaises se sont rapprochés à moins de 2 heures de Paris. Une carte de France ils au trône démontre bien qu'aujourd'hui, seule la capitale auvergnate et métropoles de Clermont-Ferrand est resté au mieux à 3 heures 20 de trajet de la capitale française et se retrouve ainsi sur la Côte-d Azur, par conséquent, si la sécurisation de la ligne Clermont Paris s'avère indispensable, les études de la réalisation d'une ligne grande vitesse sont primordiales pour réaliser désenclavement de l'Auvergne et du Massif Central et nous y veillerons particulièrement avec Rémy Pointereau, président de l'association LGV grand centre. Monsieur le ministre. effectivement, il répond à un double objectif qui répondent à la situation de la ligne à grande vitesse Paris-Lyon et améliorer l'accessibilité de de l'Auvergne et du Centre de la France, alors le le comité d'orientation des transports intérieurs enfin le le comité d'orientation le que ce coït je sais pas faire quelque chose d'abominable dans son rapport du DG du 1er février 2018 places l'horizon et l'engagement des travaux après 2038, la mise en place pour 2025 du projet de performance à grande vitesse sud-est de la ligne grande vitesse, Paris, Lyon et l'utilisation de de 2 rames plus capacitaire qui ont repoussé le, l'horizon de la saturation de la ligne après 2040 et remporte ainsi la la pertinence de réaliser une LGV dans ce contexte, la priorité du gouvernement s'est porté sur l'entretien de la ligne Paris-Clermont-Ferrand et et sa modernisation, on sait quand même, je le citais tout à l'heure mais ce schéma directeur, il prévoit un programme de régénération des voies mené par SNCF réseau en dehors de du secteur d'Île-de-France de 760 millions d'euros il y a des opérations visant à améliorer la fiabilité, la sécurité de la ligne pour 45 millions d'euros inscrit au contrat de plan État-Région, le renouvellement du matériel roulant lui aussi dans l'arrivée est prévue progressivement à partir de fin 2023 c'est un montant de 350 millions d'euros pour les trains qui circuleront sur la ligne Paris-Clermont-Ferrand et un programme de modernisation à hauteur de 130 millions d'euros dans les 2 tiers sont financés par l'État est également engagé en ce programme de modernisation qui fait l'objet d'une convention de cofinancement d'ailleurs avec la région Auvergne-Rhône-Alpes les études préliminaires ont été conduites par SNCF, réseau, elles ont permis de préciser les mesures nécessaires à l'accueil des nouvelles rames à l'horizon 2024 et à l'amélioration des temps de parcours entre Paris et et Clermont-Ferrand à horizon de 2026 je crois que, très honnêtement, c'est une ligne, je la connais bien pour l'emprunter, souvent c'est c'est une ligne qui nécessité des travaux importants car il n'y a pas que Clermont-Ferrand où il y a quand même des villes intermédiaires ryan Moulins, Vichy et également Nevers et je je pense qu'il était nécessaire d'avoir une vision de l'aménagement du territoire. Urgent le Ministre merci et la parole est enfin Monsieur François qu'elle veut pour le groupe des Républicains. Merci madame la présidente, monsieur le ministre vous ne serait pas étonné que je vous interroge sur la politique ferroviaire dans les Pyrénées-Orientales, un département qui est particulièrement décevant désavantagée en la matière, tout d'abord, je n'ai d'autre choix que de revenir sur le projet de la ligne grande vitesse Montpellier Perpignan qui se hâte, on ne peut plus lentement, nous devrions nous réjouir car il est enfin prévu d'engager des travaux mais malheureusement seulement sur un 1er tronçon Montpellier, Béziers, à l'horizon de 10 ans, puis sur le 2ème tronçon, Béziers, Perpignan à l'horizon de 20 ans pourtant, le projet de la nouvelle ligne a été initiée dans les années 90 pour construire une ligne de 140 kilomètres, il va falloir au mieux 20 ans pour que cette ligne grande vitesse voit le jour alors qu'il est s'agit d'une véritable urgence pour la ville de Perpignan et franchement est-ce digne d'une politique nationale, c'est pourquoi je me dois d'insister monsieur le ministre, il faut réaliser les travaux en une seule fois pour finir, je me dois d'aborder la question de l'exploitation de la ligne du train rouge dont la pérennité est menacée par l'état désastreux du tronçon Rivesaltes Cody, ce qui représente les 3 quarts de la ligne pour assurer la saison touristique 2021, il a fallu réaliser en urgence des travaux d'un montant de 100000 euros, la subvention de 1 1000000 et demi d'euros qui viennent d'être débloqués permettra seulement d'effectuer les travaux nécessaires à l'exploitation de la ligne jusqu'à la fin de l'année, mais pas au-delà, les derniers investissements importants sur cette ligne date de 2011, 2012, je me réjouis donc que le préfet de région missionné le préfet des Pyrénées-Orientales pour réunir dans les plus brefs délais, un comité de pilotage, mais j'aimerais avoir des précisions sur ce qu'il est prévu afin d'assurer la pérennité de cette ligne. Monsieur le Ministre. Merci madame la présidente, oui, Monsieur le Sénateur Calvet le le projet de ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, il vise à répondent durablement à la demande croissante de mobilité aux problèmes de congestion sur l'axe ferroviaire unique du Languedoc Roussillon, il va permettre également de créer un service à haute fréquence, le long de l'axe littoral et d'assurer la continuité de la grande vitesse ferroviaire entre la France et Barcelone sur la façade méditerranéenne au bénéfice bien sûr de tout l'arc méditerranéen, la ligne nouvelle mixte, fret et voyageurs entre Montpellier et Béziers va permette de gagner 18 minutes entre Montpellier et Béziers ainsi Perpignan, soit près de la moitié en fait des gains de temps de parcours qui sont permis par l'ensemble du du projet de loi d'orientation des mobilités prévoit la réalisation faisaient de la de la LNM P, en commençant par l'engagement d'ici à la fin de la décennie, des travaux de la liaison mixte, fret et voyageurs entre Montpellier baiser Béziers, c'était un peu plus de 2 milliards d'euros, puis dans un second temps, de la section, Béziers, Perpignan, un peu moins de 6 milliards d'euros on on est sur une logique de finir en 2035 2 dès la première phase et d'État 2000 45 sur la sur la 2ème phase ce qui peut effectivement être d'une moyenne à 2040, comme vous le comme vous l'indiquiez alors l'État a souhaité accélérer la réalisation du calendrier de cette opération tout en assurant la sécurité juridique du dossier avec une enquête publique, de la section Montpellier-Béziers qui s'est terminée le 27 janvier comme vous le savez, dans cette perspective, les différents co-financeurs, l'État, la région Occitanie, les collectivités locales ont acté lors du comité de pilotage du 2 septembre 2021, leur accord de principe sur la répartition des financements pour la réalisation de la section Montpellier baiser avec une participation de 40 % de l'État à parité avec les collectivités, une contribution de l'Union européenne, qui est attendu autour de de LNP pardon, c'est à la création d'une société de financement dédié à la BNP est à l'étude et là aussi je pense que que que vous le savez, mais le le protocole d'intention de financement pour la réalisation de la première phase de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan a été signé par le 1er ministre et le samedi 22 janvier

Oui je j'attends la réponse sur le train rouge mais il n'y a pas eu le temps de de me répondant, Monsieur le Ministre, et il ne peut s'il le veut. Par écrit sur ce cet aspect de la question du sénateur. Merci, la parole est maintenant, pour conclure ce débat au président l'ange au président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Merci madame la présidente, madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, avant toute chose, je tiens à remercier chacun des intervenants pour ce débat riche, riche, je le pense et je pense aussi nécessaire, comme l'a indiqué notre collègue Philippe Tabarot, nous sommes à une période charnière de mise en oeuvre des dernières réformes ferroviaire: l'ouverture à la concurrence du transport national des voyageurs conventionnés ou non la possibilité pour les régions de reprendre des lignes de desserte fine du territoire ou encore la signature d'un nouveau contrat de performance entre l'état et SNCF, réseau sont autant de paramètres qui modifie en profondeur le système ferroviaire national et son modèle économique et qui soulève un grand nombre d'interrogations au niveau local, grand nombre de d'interrogations que certains de mes collègues ont souhaité vous Monsieur le Ministre, Monsieur le Ministre, l'étendue des questions qui ont été posées, mais aussi leur précision montre, en effet, à quel point ce sujet est d'actualité et ce sujet suscite des inquiétudes inquiétudes légitimes, il me semble que ce débat a permis de mettre en lumière 4 points d'attention et de vigilance, le 1er point qu'il me semble important d'évoquer et l'impact de la crise sanitaire sur le système ferroviaire dans son ensemble et ses potentielles conséquences en matière de desserte de nos territoires, d'une part, la crise a provoqué des bouleversements, des comportements des usagers en matière de mobilité dont les effets sont encore incertains à long terme, nous avons par exemple constaté, comme l'a justement souligné Daniel Guéret qu'une partie de nos concitoyens ont choisi, à la faveur du télétravail de s'éloigner des zones les plus urbanisées, au besoin, déjà existant en matière de desserte du territoire s'ajoutent donc de nouveaux besoins,

le Sénat a d'ailleurs été moteur pour inscrire dans la loi loi climat et résilience du 22 août 2021, les objectifs de développement de la part modale du transport ferroviaire, le second point qui fait consensus puisqu'un grand nombre d'interventions sur tous les bancs et de toutes les régions l'ont mentionné s'apparente davantage à un regret, les moyens déployés pour le maillage du territoire en matière de transport ferroviaire sont loin d'être à la hauteur des enjeux et des objectifs en matière de développement du transport ferroviaire, monsieur le Ministre ne transformez pas ses objectifs en incantations et donné au transport ferroviaire sur l'ensemble du territoire, et pas uniquement au niveau des plus grandes agglomérations, les moyens d'attendre, d'atteindre les ambitions que nous nous sommes fixés ensembles qu'il s'agisse des petites lignes des trains d'équilibre des territoires, des réseaux structurant des capillaires fret, nous avons pu constater des améliorations, mais à ce stade, le compte n'y est pas certains de mes collègues ont d'ailleurs évoqué des cas de figure absolument déplorable, avec un réseau ferré très dégradée, à l'image du réseau sud Aquitaine évoquée par notre collègue Denis Saint-Pé à l'heure où il est question, pour les régions de reprendre un certain nombre de petites lignes un accompagnement financier un engagement à long terme dans le réseau et dans certains cas de figure, le matériel roulant a est absolument indispensable, faute de quoi l'égalité de nos concitoyens en matière de mobilité serait signifie significativement affaiblis, le 3ème point qui me semble devoir être soulignés concerne les discussions en cours au contrat de performance entre SNCF, réseau et l'État, ce contrat qu'on évoquait, mes collègues, Philippe Tabarot et Olivier Jacquin, vous l'avez sans doute compris, Monsieur le Ministre, ce contrat, nous sommes là, vont devoir être amendée pour sortir d'une stricte vision budgétaire et définir une stratégie stratégie ambitieuse de développement du train sur l'intégralité de notre territoire, espérons que les consultations des différentes parties prenantes permettent d'ajuster ce projet de contrat conformément aux alertes que nous avons fait au tout début de l'année, le 4ème et dernier point que je souhaitais évoquer devant vous, monsieur le ministre, de nos échanges concernent la vision stratégique, stratégique ambitieux, ce que nous appelons de nos voeux les évolutions que j'ai évoqué il y a quelques instants, ouverture à la concurrence, crise sanitaire régénération des petites lignes ont des conséquences importantes sur le modèle de financement du système ferroviaire dans son ensemble qui reposait jusqu'à présent en grande partie sur le TGV et invite à la réinterroger pour faire du train, un véritable outil outil au service d'un maillage équilibré du territoire et d'une mobilité durable et monsieur le ministre en charge de la ruralité nous comptons sur vous. Oui, monsieur le président. Je vais maintenant suspendre la séance se sont reprises en quelques instants, pour le débat sur le suivi des ordonnances, la séance est suspendue.

Notre ordre du jour appelle le débat sur le suivi des ordonnances. Monsieur le Ministre. Madame le président de la délégation du bureau chargé du travail parlementaire du contrôle du suivi des ordonnances. Mesdames et messieurs les présidents, mes chers collègues, nous nous retrouvons cet après-midi pour débattre, c'est la première fois, du suivi des ordonnances qui sont prises en application de l'article 38 de notre constitution, je voudrais saluer Marc Fesneau, ministre en charge des relations avec le Parlement, qui répondra au nom du gouvernement aux questions du Sénat, je voudrais rappeler que ce débat répond à la volonté exprimée par notre assemblée depuis un certain nombre d'années, volonté d'encadrer davantage le recours aux ordonnances et d'en améliorer le suivi. Il fait suite aux préconisations du groupe de travail sur la modernisation des méthodes de travail du Sénat a adopté le 25 mars 2021 et à la dernière réforme de notre règlement qui a consacré l'importance du contrôle des ordonnances par le Parlement est un porteur de chaque loi sont désormais, je le rappelle, au-delà de ce débat, chargé de suivent la publication des ordonnances publiées sur leur fondement. Le gouvernement, pour sa part, doit présenter au début de chaque session ordinaire, un programme prévisionnel de la publication des ordonnances et des demandes d'inscription à l'ordre du jour des textes de ratification. Pour faciliter le contrôle des ordonnances et leur ratification le Sénat rend public depuis un an maintenant, un suivi hebdomadaire du recours aux ordonnances qui permet à tous les acteurs de la loi, mais aussi aux citoyens de consulter les chiffres actualisés. Les habilitations accorder des ordonnances publiées et aussi de celles qui ont été ratifiées. Ces chiffres illustrent un recours très soutenue

20 % des ordonnances publiée lors de ce quinquennat ont été à ce jour ratifié. Cette raréfaction s'accentue, seulement 10 % des ordonnances publiées ces 3 dernières années ont été ratifiées. C'est le niveau le plus bas qui ait jamais été observée. Je crois que ce débat dans le permettent de tirer à la fois la sonnette d'alarme, d'obtenir des réponses farce à une évolution que je juge pour le Parlement assez préoccupant, je vais donc donner la parole à la vice-présidente en charge du travail parlementaire, du contrôle et du suivi des ordonnances qui va nous présenter le bilan de l'année 2021, madame la présidente, Pascale Gruny. Je vais vous donner la parole. un débat en séance publique sur les ordonnances prises en application de l'article 38 de la Constitution, comme vient de le rappeler notre président, je me félicite de la tenue de ce débat dans les ordonnances se sont multipliées ces dernières années, jusqu'à venir concurrencer la loi comme de normal d'élaboration des textes à valeur législative, monsieur le ministre, vous connaissez la position du Sénat sur la question des ordonnances, elle n'est pas nouvelle et nous vous achetons régulièrement sur ce sujet, j'ai moi-même eu l'occasion de vous faire part de notre préoccupation lors du débat sur l'application des lois, l'an dernier, personne ici ne ni l'utilité des ordonnances tant qu'elle porte sur des sujets techniques comme les travaux de codification à droit constant, il est donc acceptable que le gouvernement sollicite des habilitations à légiférer par ordonnances dans des proportions raisonnables et à condition que le débat parlementaire soit permis permis lors de la ratification des ordonnances mais les ordonnances désormais constituer un mode normal d'élaboration de la loi, cette année, malgré les efforts constants du Sénat pour limiter le recours aux ordonnances en supprimant des habilitations ou réduisant leur périmètre, les chiffres sont alarmants : 90 ordonnances ont été publiées en 2021 en ne tenant pas compte de l'année 2020 qui, reconnaissons-le, fut exceptionnelle ce chiffre constitue le record du nombre annuel d'ordonnance publiée sous la 5ème République, c'est également le double de la moyenne annuelle d'ordonnances publiées depuis 2007, or seulement 10 ordonnances sont en lien Direct avec l'épidémie de Covid 19, contrairement à l'année précédente, le recours élevé aux ordonnances ne se justifie donc pas par la réponse apportée aux conséquences de la crise sanitaire sur l'ensemble du quinquennat à la date du 1er janvier 2022, nous atteignons le nombre impressionnant de 326 ordonnance publiée, soit presque 3 fois plus qu'au même stade du quinquennat 2007, 2012 et moitié plus qu'à la même période du quinquennat 2012, 2017, mes chers collègues, en 2021 pour vous donner un ordre de grandeur pour 90 ordonnance publiée 64 3 64 lois ont été promulguées 58 % des textes intervenant dans le domaine de la loi, ont donc été par des ordonnances, désormais, hé bien qu'une ordonnance n'est souvent pas une portée équivalente à celle d'une loi, il y a chaque année davantage d'ordonnances publiées que de loi promulguée et ceci est une spécificité du quinquennat actuel en parallèle, seuls 65 ordonnances ont été ratifiées depuis le début du quinquennat soit moins de 20 % du total des ordonnances publiées, comme l'a rappelé, notre président Gérard Larché sur les 3 dernières années, ce chiffre s'il se situe même à 10 et encore, c'est en partie grâce aux efforts du Sénat qui a intégré par la voie d'amendement des ratification d'ordonnances, ce sont des chiffres que nous ne pouvons que déplorer en particulier à la suite du revirement récent de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui s'estime compétent pour traiter à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité des ordonnance non ratifiée dans le délai d'habilitation a expiré en résumé, nous assistons à une hausse du recours aux ordonnances il y a une chute du taux de ratification, le Sénat ne peut cautionner une telle évolution lors du débat sur l'application des lois, de juin 2021 vous aviez monsieur le ministre a reconnu que les ordonnances était devenu un moyen comme un autre, de faire la loi, je me permets de vous citer pour parler franchement, le constat d'une forme de banalisation me semble difficile à contester, vous expliquer ensuite cette banalisation par l'inflation législative par le gain de temps que permettrait les ordonnances et trouviez des circonstances atténuantes dans la crise liée à la pandémie de Covid 19, je tiens à vous répondez à vous interroger sur ces points, tout d'abord s'agissant de l'inflation législative et de l'encombrement de l'ordre du jour, c'est le gouvernement qui en est le principal responsable, par ailleurs, sauf dans le cas d'habilitation des très restera comme ce fut le cas pour le 1er texte d'urgence sanitaire, avec des délais d'un mois, les ordonnances ne permettent pas de gagner du temps avant d'être publié une ordonnance doit d'abord faire l'objet d'une demande d'habilitation, par définition, le temps de publication d'une ordonnance inclus le temps d'adoption de la loi contenant l'habilitation ainsi hors texte, financiers, le délai moyen d'adaptation d'une loi a été de 250 jours lors de la session 2020, 2021 tandis qu'il fallait 436 436 jours entre le dépôt d'une demande d'habilitation par le gouvernement et la publication d'une ordonnance sur le plan sanitaire, nous avons votées des habilitations, que vous nous avez demandé en 2020 dans les textes d'urgence sanitaire et nous continuons de reconnaître que les chiffres de l'année 2020 ne sont pas représentatifs, en revanche, comme je viens de le dire, l'année 2021 Marc à la fois un niveau soutenu de publication d'ordonnance, mais aussi une banalisation du recours aux ordonnances puisqu'en comparaison avec l'année 2020, elles ont porté sur des sujets très divers qui ne sont pas liées à la pandémie de Covid 19 et aurait très bien pu faire l'objet qui ne loi classique, je pense par exemple à leur donnant sur la réforme de la haute fonction publique ou encore celle sur la mise en oeuvre et de la création de la 5ème, branche du régime général de la Sécurité sociale, relatives à l'autonomie, publié en 2021, en réalité, ces exemples illustrent que le recours aux ordonnances apparaît davantage comme un moyen de contourner le débat parlementaire que de gagner du temps, le débat parlementaire peut non seulement être contourné par le recours massif aux ordonnances, mais plus grave encore bridé en effet chaque habitation consenti a pour conséquence concrète : un dessaisissement du Parlement puisqu'il ne peut lier légiférer sur le sujet tant que le délai d'habilitation n'est pas expiré, quand bien même l'ordonnance ne serait finalement pas publié, j'en viens donc à ma 1ère question : la banalisation du recours aux ordonnances est-elle une méthode d'action assumée et revendiquée par le gouvernement, je vous cite une seconde fois, monsieur le ministre, cette fois-ci pour vous interroger sur la politique du gouvernement en matière de ratification, vous nous avez dit lors du débat sur l'application des lois, de juin 2021, qu'en ce qui concerne la ratification des ordonnances par le Parlement, le gouvernement s'engage généralement au moment de la demande d'habilitation et s'agissant de sujets d'intérêt pour les parlementaires à inscrire à l'ordre du jour le projet de loi de ratification, s'il est vrai qu'en 2021, l'ensemble des 62 projets de loi de ratification a été déposé à temps sur le bureau de l'une des 2 assemblées, seuls 3, soit moins de 5 % ont été ont été inscrits à l'ordre du jour par le gouvernement, nous sommes donc loin de l'engagement qui a été pris, l'année dernière, devant nous, l'absence de ratification pose des problèmes concrets à 2 reprises au cours des dernières semaines, le gouvernement a transmis aux assemblées des demandes de désignation dans des organismes extraparlementaires en vertu d'ordonnance non ratifiée, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ont refusé d'y donner suite, considérant que le gouvernement préjugés ainsi de l'avis du Parlement et que ces saisines était donc prématuré l'une d'entre elles a même été envoyée alors qu'était en cours d'examen, le projet de loi de ratification de l'ordonnance créant l'organisme en cause le conseil d'administration de l'Autorité des relations sociales, des plateformes d'emploi la disposition prévoyant la présence de parlementaires au sein de au sein de ce conseil ne figure d'ailleurs plus dans la version finale du texte qui a été adopté la semaine dernière, cette précipitation était donc bien inutile, j'en arrive donc à ma seconde question devant un engagement qui ne sont visiblement pas avoir été tenu, pourriez-vous nous indiquer si et comment la politique du gouvernement en matière de ratification d'ordonnances à évoluer, monsieur le ministre, le Parlement, c'est la voix du peuple, il ne faut pas la négliger merci. Merci madame la présidente. Vous avez maintenant la parole à au ministre délégué auprès du 1er mini-chargé des relations avec le Parlement et la participation citoyenne. Monsieur le ministre. Avez la parole. Monsieur le président, madame la présidente, Pascale Gruny, mesdames et messieurs les présidents de commission, mesdames et messieurs les sénateurs, je tiens tout d'abord à remercier la présidente Pascale Gruny, ainsi que l'ensemble des présidents de commissions et les services du Sénat pour leur travail de grande qualité qui va nous permettent d'échanger sur un sujet particulièrement important et sensible pour le Parlement, comme pour l'ensemble de nos concitoyens, celui des ordonnances votre assemblée a depuis la dernière réforme de son règlement 2021, décidé de mettre en oeuvre un suivi systématique de cet outil, prévue à l'article 38 de la Constitution et par lequel le Parlement délègue temporairement au gouvernement une partie de sa compétence de législateur, comme j'avais pu l'indiquer en conférence des présidents, le gouvernement salue avec intérêt cette initiative du Sénat, il s'agit du 1er débat que nous avons en la matière, je forme le voeu qu'il soit fructueux que ce dialogue entre nos institutions soit source d'amélioration de recherche de bonnes pratiques ou d'évolution, je sais que cela est possible, si je me réfère au travail mené sur l'application des lois par votre assemblée depuis de nombreuses années, il y a dans cet exercice de contrôle une réelle utilité, qui sera une nouvelle fois démontré ce soir, je n'en doute pas, celle de nous améliorer le recours aux ordonnances apparaît souvent comme une nécessité afin de concilier les contraintes de calendrier parlementaire et les exigences liées à la la voir ration de certaines dispositions législatives particulièrement technique, le gouvernement n'y a pas recours par volonté de court-circuiter le Parlement mais dans un souci d'apporter avec la plus grande avec le plus d'efficacité possible une réponse à un problème juridique pour répondre à l'une des questions de Madame, la présidente Gruny, madame la présidente, vous avez souligné comme d'autres, ne manqueront pas de le faire, j'imagine le nom très important d'ordonnances que le gouvernement a été habilitée à prendre sous ce quinquennat ainsi que les délais d'habilitation et le taux de ratification regardons ces chiffres avec lucidité, tentons de les comprendre et voyons si le reflet des dysfonctionnements auxquels le gouvernement pourrait ou peut répondre, il est exact, en effet, d'indiquer que le gouvernement a pris depuis 2 ans, un nombre record d'ordonnance dans des domaines très variés, je tiens à rappeler cependant qu'une grande partie de celle-ci ont été, pour faire face à l'urgence de la crise sanitaire et à l'impossibilité de réunir le parlement de manière continue, elles ont permis, dans un contexte nécessitant une adaptation permanente face à la crise d'apporter des réponses au plus proche des préoccupations de nos concitoyens et ce, alors même que nos administrations, à l'image de nombreux secteurs de notre pays était sous tension : nous devons garder à l'esprit que cette situation inédite, vous l'avez d'ailleurs rappelé, madame la présidente, qui rend cet exercice de comparaison avec le quinquennat précédent un peu difficile, même s'il faut comparer des choses ainsi sur les 2327 ordonnances prises depuis 2017 93 étaient ainsi liées à la crise sanitaire, selon nos calculs, si nous mettons cette situation exceptionnelle de côté le nombre d'ordonnances prises par le gouvernement s'élève depuis le début du quinquennat 234, un nom qui reste élevé mais qui s'inscrit dans une tendance longue et se situe entre le quinquennat de François Hollande avec 271 ordonnance et celui de Nicolas Sarkozy, avec 152 ordonnance ce phénomène va de Pair avec une croissance toujours continue du nombre de lois promulguées, on peut dès leur remarquer que hors convention internationale, la part des ordonnances dans la production législative s'élève à 53 % sous ce quinquennat sous un taux à peine de 2 points supérieur à celui du précédent, nous sommes donc loin d'une quelconque dérive quand on recourt aux ordonnances de ce gouvernement contraire loin d'être une sorte de de la génération spontanée, le nombre des ordonnances est le symptôme d'une inflation normative, je l'avais dit effectivement continue et généralisée à laquelle nous devons collectivement réfléchir au fond tout le monde a sa part et nous le savons, pour beaucoup d'entre nous, par delà les statistiques, il n'est pas toujours aisé de manier entre 2 quinquennats et qui ont connu chacun leur lot de difficultés de surprises ou de bouleversements, je souhaite vous redire également qu'à chaque fois qu'il a pu le gouvernement s'attache où s'est attaché à transformer les demandes d'Haditha d'habilitation endroit substantiel travaillant pour se la main dans la main avec le Parlement, en particulier d'ailleurs avec le Sénat, je pense par exemple au projet de loi portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid 19 de 4 articles, nous étions passés à 61, inscrivant dans le dur, au fond, un certain nombre d'habilitation, qui avait été initialement était prévu, il n'est pas aisé de retrouver des chiffres globaux concernant cette pratique, mais elle permet aux parlementaires au cours de la navette de renoncer à se dessaisir de la compétence qui est la leur, en travaillant de concert avec le gouvernement. Par ailleurs, j'entends parfois et ce n'est pas toujours faut que la législation par ordonnances serait plus lente que le recours à la procédure législative classique, vous l'avez rappelé, madame la présidente j'entends cette critique et je sais que le Sénat veille et verra ce que des délais d'application des lois dont les ordonnances sont parfois un élément important, soient les plus réduits possible dans ce domaine, j'observe que le gouvernement actuel demeure soucieux de prendre des ordonnances dans un délai inférieur à l'habilitation parlementaire ainsi le gouvernement adopte ces ordonnances plus rapidement que sous les 2 précédents quinquennats en moyenne 2 tiers du délit d'habilitation est utilisée contre 78 % pour le quinquennat de François Hollande et 82 % pour le quinquennat quinquennat pardon de Nicolas Sarkozy, le Parlement fixe donc un délai butoir au gouvernement pour légiférer et celui-ci essaye au mieux de le réduire pour accélérer la production normative, c'est d'ailleurs l'objectif j'aborderai enfin la question de la ratification j'ai déjà fait l'objet l'an dernier, des débats, vous avez indiqué, madame la présidente, qui est, qui ne manquera pas de susciter de nombreuses remarques, aujourd'hui je le sais : ah la la, président Gruny a regretté que le le Parlement et plus particulièrement le Sénat ne soit pas saisie de projet de loi de ratification des ordonnances prises par le gouvernement de manière plus générale, j'entends la critique des parlementaires qui déplore être privés d'un débat sur des mesures contenues dans les ordonnances, je voudrais vous apporter des éléments de réponse à ce sujet, tout d'abord, il est utile, je crois, de d'accorder un temps nécessaire au débat sur les réformes substantielles et de réserve aux ordonnances les écritures les plus techniques il y les plus urgent, c'est d'ailleurs leur fonction étant donné la densité de lors du jour, il n'est pas toujours possible ni même souhaitable d'inscrire trop de trop nombreux, texte dont l'examen ne susciterait pas le plus grand enthousiasme les plus grandes controverses, le débat,

de la justice pénale des mineurs, le Parlement demeure au demeurant libre d'inscrire à son nord du jour notamment de contrôle la ratification d'ordonnances dont il souhaite débattre ou amender le contenu, le gouvernement est bien entendu à sa disposition pour se plier à cet exercice de contrôle de son action, je remarque cependant que davantage qu'une ratification du Sénat souhaite souvent sur certains sujets, faire connaître son point de vue au sujet de la réforme de la haute fonction publique, c'est le Sénat lui-même qui a refusé la ratification d'une ordonnance, quitte à la modifier, alors qu'il avait pourtant inscrite de son propre chef à l'ordre du jour, le Parlement a donc bien la capacité de ratifier les ordonnances de sa propre initiative et de débattre avec le gouvernement de toute réforme, y compris celles mises en Oeuvres par les ordonnances, le problème n'est donc pas toujours l'acte juridique de ratifier mais plutôt la capacité et vous avez raison, madame la présidente, dont les chambres disposent d'un scrutin, texte de ratification, alors l'Ordre à leur ordre du jour et dans l'exercice ne fait pas toujours consensus on peut regretter que le Parlement se sont dessaisis de sa prérogative législative avec son autorisation, je tiens toutefois à le rappeler mais après une année parlementaire de tous les records pour reprend les termes du rapport d'activité du Sénat 2020, 2021, je ne crois pas qu'il aurait été objectivement envisageable d'inscrire à l'ordre du jour des textes supplémentaires, un meilleur dialogue sur ce point entre le gouvernement et le Parlement devrait davantage permettent d'identifier des points de tension que soulève telle ou telle ordonnance et qui justifierait en effet l'examen d'un texte ad-hoc ou d'une disposition particulière de ratification, restait à savoir quelle forme peut prendre le dialogue, il faudra sans doute y réfléchir pour conclure mon propos, enfin, je souhaite rappeler que le recours aux ordonnances est un outil précieux à la disposition du gouvernement est prévue dès 1958 à la fois pour mettre en oeuvre rapidement des réformes techniques nécessaires et pour agir aussi vite agir vite pardon face à une situation de crise et c'est bien à cela que le gouvernement a entendu se tenir ce mode de législation ne sera en aucun cas remplacer le débat parlementaire auquel vous le savez nous sommes et je suis particulièrement attaché, celui-ci peut d'ailleurs aboutir, comme c'est souvent le cas, à mieux définir une habilitation ou en restreindre la portée je fais donc le voeu qu'un équilibre soit trouvé entre les attentes des députés et des sénateurs et les nécessités qui s'impose parfois au gouvernement, tout comme le souci de ne pas surcharger inutilement l'ordre du jour des 2 assemblées, le débat que nous tenons aujourd'hui comme le travail opéré par madame la présidente, tout au long de l'année, ainsi que par le secrétariat général du gouvernement, que je tiens à saluer pour la grande qualité de son travail, participe de cet objectif, c'est une première étape, je suis certain que cet exercice inédit aujourd'hui trouvera la même efficacité que celui qui se tient chaque année concernant l'application des lois, et c'est bien pour cela que c'est une innovation précieuse, je me tiens donc à présent à votre disposition pour répondre aux présidentes et présidents de commission, ainsi qu'aux orateurs de chaque groupe, je vous remercie. Merci monsieur le ministre, nous allons maintenant procéder au débat sous forme interactive, il a 2 minutes au maximum, avec la possibilité, Monsieur le ministre, elle est souhaitée d'une réponse du gouvernement pour une durée équivalente de 2 minutes dans ce débat, la parole est aux représentants des commissions et je vais donner la parole à la présidente de la commission des affaires économiques Madame Sophie Primas vous avez la parole. Merci beaucoup monsieur le président, monsieur le ministre, le constat qui a été dressé par notre collègue Pascale Gruny sur le recours aux ordonnances est éloquent, vous savez que nous n'aimons pas beaucoup les ordonnances elle dessaisissent le Parlement, elles ne permettent pas d'aller plus vite et elle donne souvent l'impression de soustraire le débat à la représentation nationale aussi notre commission économique a été particulièrement vigilante lors de l'examen de la loi climat résilience l'été dernier sur la réforme particulière du code minier par voie d'ordonnance, c'est un euphémisme de dire que cette réforme était très attendue, elle est naturellement technique, elle est sensible, mais à l'heure où la souveraineté minière apparaît plus que jamais comme une nécessité, notre commission a souhaité que le Parlement, il prenne toute sa part je saisis donc l'occasion de ce débat pour vous demander un point d'étape sur l'avancée de cette réforme du code minier, à l'initiative de Daniel Gremillet plusieurs dispositions initialement renvoyés à l'ordonnance ont été inscrites dans le dur, pouvez-vous nous confirmer, monsieur le Ministre, qu'il s'agit là bien d'un acquis que le travail du législateur sera complété et n'ont pas modifié par les autres ordonnances voire dénaturé par ailleurs, le Sénat avait souhaité que les parties prenantes soient associés au mieux à l'élaboration des ordonnances, pouvez-vous me faire un point d'étape sur ce sujet, et enfin en commission mixte paritaire, le délai d'habilitation a été ramenée à 15 mois, le gouvernement ayant d'ailleurs indiqué que l'entrée en vigueur du nouveau code minier d'ici la fin de l'actuelle législature constituerait une garantie pour la réforme engagée comme le timing est de plus en plus, je voulais savoir si ces délais seront tenus, merci monsieur le Ministre. Oui, monsieur le président, madame la présidente, Prima, vous m'interrogez sur la réforme du code minier par voie d'ordonnance, qui a été inscrite, effectivement, je me souviens de discussions que nous avions eu à l'époque dans la loi climat et résilience examiner l'été dernier, vous soulignez, cette réforme est très attendue et revêt une importance stratégique pour notre pays et beaucoup de territoires de notre pays, l'Arctique 80 la loi du 2 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique qui renforçant, renforcement de la résilience face ou à ses effets habilite le gouvernement à réformer le modèle Mini et le gouvernement dispose de 30 mesures d'habilitation qui expire le 21 novembre 2022 la rédaction des textes portant réforme du code est actuellement en cours de finalisation le lancement des consultations obligatoires, notamment des consultations du public du Conseil national d'évaluation des normes et des collectivités d'outre-mer est imminente, je tiens ici à vous rassurer les dispositions de ces textes ne remettront pas en cause des dispositions insérées dans la loi, à l'initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques, elles seront simplement compléter dans le strict cadre des articles d'habilitation unique l'ensemble des parties prenantes, a été étroitement associée à l'élaboration des ordonnances ainsi le projet de réforme du code minier a été présentée aux acteurs, à une douzaine d'occasions depuis le mois d'octobre 2021

une réunion interministérielle s'est encore tenue hier, réunissant l'ensemble des ministères sur les assurés que le gouvernement met tout en oeuvre pour que cette réforme tant attendue, voit le jour dans les meilleures conditions et dans les délais qui était parti. Merci le donner la parole à notre collègue Olivier Cigolotti, vice-président de la commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées, qui remplace le président quand bon monsieur le président, vous avez la parole. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, comme vous le savez les textes législatifs, présentés par le gouvernement et voté par le Parlement sur les secteurs de compétence, d'une autre commission détermine en profondeur l'action menée par nos armées et par notre réseau diplomatique à travers le monde, c'est pour cette raison qu'il est essentiel que lorsque ces loi habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance le Parlement soit à nouveau consulté et puis s'exprimer sa position sur des sujets dont les conséquences de long terme se révèle souvent structurante à ce titre-Monsieur le Ministre, nous regrettons que le projet de ratification des 4 ordonnances prévues par l'article 30 de la loi de programmation militaire du 13 juillet 2018 n'est toujours pas fait l'objet d'une inscription à lors du jour de l'Assemblée nationale. Alors même que l'esprit de la LPM et d'associer la représentation nationale, nous regrettons la suspension du processus législatif sur des sujets aussi importants que la reconversion dans la fonction publique de nos anciens militaires ou l'extension du congé du blessé aux combattants engagés dans des missions sur le territoire national, par ailleurs, mes chers collègues, sur un autre sujet, donc chacun de nous mesure l'importance nous regroupons nous regrettons le choix qui a été fait de ne pas associer la représentation nationale au travail d'adaptation de notre droit pour tenir compte du Brexit, alors même que le Sénat a développé une expertise réelle sur ce sujet au travers du groupe de suivi coprésidé par les présidents Christian Cambon Jean-François Rapin, pourquoi ne pas associer le Parlement enfin le projet de loi ratifiant diverses ordonnances sur les conséquences du Brexit déposé à l'Assemblée nationale, dès février 2021 n'a jamais été débattue, ce qui laisse peu d'espoir quant à l'examen de ce texte par notre assemblée en conclusion, Monsieur le Ministre, notre commission salue le renforcement du suivi des ordonnances engagée par le bureau du Sénat, nous appelons simplement le gouvernement à inscrire systématiquement ses projets de ratification à l'heure du jour des assemblées pour nous permettent de tenir un débat contradictoire sur des décisions importantes, je vous remercie. Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Cigolotti vous m'interrogez sur 2 séries d'ordonnances prises en vertu d'habitation que votre commission examiné sous ce quinquennat sur lesquels vous alerter également le président Cambon dans les 2 cas, il s'agit de sujets d'importance, vous avez raison, comme vous l'avez souligné puisque ces ordonnances ont trait à la programmation militaire et au Brexit s'agissant de ce 2ème sujet : le Brexit donc pourra représenter le gouvernement au Parlement à l'époque sur ce texte d'habilitation, je garde en mémoire des débats importants qui ont eu lieu, tant sur le fond que sur la forme, partant d'un texte initial prévoyant une habilitation à légiférer par ordonnance de 30 mois ce qui nous amené au delà de l'élection présidentielle, c'était bien cela qui avait été souligné la commission mixte paritaire a abouti à une rédaction limitant cette délégation à 12 mois seulement, je tiens à rappeler que cette évolution était le fruit d'une négociation et d'un dialogue tout à fait légitime entre le gouvernement, les députés et les sénateurs chacun convenant qu'un compromis pouvait et devait être trouvée, le Sénat a par ailleurs adopté après un débat fournit l'essentiel de l'habilitation, même si j'entends vos regrets concernant l'absence de ratification, je crois que le débat a pu avoir lieu sur ce sujet, y compris d'ailleurs sur le recours aux ordonnances, s'agissant de la loi de programmation militaire, je sais que votre commission est très attaché au suivi de sa mise en oeuvre, particulièrement dans la période de tension forte au niveau international que nous connaissons, je comprends que ça n'est pas tellement la méthode du recours aux ordonnances qui sont posés une difficulté puisque votre mission on avait adopté le principe, conformément au texte de l'Assemblée, mais là encore, l'absence de débat parlementaire ultérieures et j'en ai parlé tout à l'heure votre question s'inscrit donc dans la suite du propos que j'ai tenus préalablement il somme nécessaire qu'un travail de concertation puissent être menées puissent être menées pardon entre le gouvernement et le Sénat afin d'identifier des textes de ratification dont celui-ci souhaite débattre, je vois mal comment on pourrait le faire pour tous les textes bon moins d'identifier les textes de ratification dont celui-ci, le Sénat où l'Assemblée éventuellement pourrait débattre ici pas apparaît difficile à de compléter à l'infini lors du jour, nous pourrions tirer ces enseignements du travail de suivi des dans des ordonnances et c'est bien l'utilité, me semble-t-il de ce 1er exercice afin de mieux anticiper les ratifications jugées comme nécessaire par votre assemblée. Madame la présidente, Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Merci monsieur le président, 2 ans et 5 mois, c'est le temps qu'il aura fallu pour prendre l'ordonnance numéro 2021 tirs à 611 du 19 mai 2021 relatives au service aux familles une période pendant laquelle le Parlement a été dépossédé d'un sujet pourtant peu technique et qui intéresse le Sénat au titre des compétences des collectivités territoriales sur les modes d'accueil de la petite enfance, rappelons que cette ordonnance a été prise sur le fondement de l'article 99 de la loi 2020 tiret 15 25 du 7 décembre 2020 d'accréditation, une simplification de l'action publique cette habilitation du gouvernement par la loi pour une durée de 6 mois à compter de la promulgation de la loi résulte de l'incapacité du gouvernement de publier l'ordonnance dans le délai de 18 mois à compter de la publication de la loi 2018 727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance et SoC dans l'Arctique 50 donnait déjà habilitation au gouvernement, c'est un peu compliqué, pris du délai prix pour cette publication 7 heures donnant s'est caractérisée par une forme d'habilitation rechargeable prise à titre conservatoire ou de précaution que nous voyons malheureusement trop souvent l'étude d'impact de la loi ASAP indiqué qu'un projet demain s'était établie dès l'Automne 2019 mais des concertations avaient mis en évidence le besoin de prendre des dispositions complémentaires, je cite, il est apparu opportun de laisser la possibilité de compléter le projet d'ordonnance préparé en 2019 par d'autres mesures d'ordre qui pourrait être proposé à l'issue de la réflexion lancée à la demande du président sur les 1000 premiers jours et de la mission de l'IGAS sur la PMI l'habilitation retenus par la loi ASAP donc plus large que celle de la loi et le Sénat avait supprimé tant l'article 50 de la loi que l'article 99 de la loi ASAP en première lecture, force est de constater que la suite des événements lui a donné raison. Monsieur le Ministre. notamment en matière d'accueil du jeune enfant et de la soutien à la parentalité, le délai d'habilitation était de 6 mois à compter de la publication de la loi, donc le 7 juin 2021 cette relance a nécessité des consultations qu'il s'agisse des acteurs de la société civile, mais aussi des commissions consultatives, ainsi que des collectivités, ces consultations se sont terminées fin mars 2021 et le Conseil d'État a été saisi rapidement après le 19 avril 2021 donnons, ça a été publié au JO du 20 mai 2021, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de rigueur, le projet de loi de ratification de l'ordonnance a ensuite été déposée sur le bureau des assemblées le 13 juillet je vous précise que l'ordonnance est désormais appliqué à 90 % puisqu'un décret d'application doit encore être publié concernant les modalités d'application de l'article 9 de l'ordonnance relative à la possibilité pour les autorités compétentes d'organiser leur coopération en matière de service aux familles en vue de favoriser le développement des services aux familles à l'échelle d'un département d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une commune la finalisation du projet de texte est en cours et il est prévu qu'il soit transmis pour consultation obligatoire en ce début d'année 2022. Merci, la parole est maintenant au président Longeau, président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Merci monsieur le président, monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ce débat à l'occasion de rappeler à quel point le recours aux ordonnances et fréquent, alors même que l'on constate que le gouvernement ne prend pas toujours les ordonnances, pour lesquels il y a pourtant demandé au Parlement de se dessaisir de son Champ de compétences, je citerai un exemple dans le domaine des transports que l'on pourrait qualifier d'habilitation de confort l'ordonnance prévue à l'article 83 de la l'homme visant à définir les conditions de la prise en charge par l'employeur de certains frais de transport n'a toujours pas été publié l'an dernier nous avait été répondu que l'opportunité de recourir à une ordonnance sera évalué sur la base d'un bilan et du baromètre forfait mobilité durable, comment le gouvernement peut-il demander au Parlement de prendre des mesures du domaine de la loi pour engager des réformes dont il n'a même pas pris le soin d'évaluer l'opportunité cette pratique quand Thierry a dépossédé législateur de sa compétence, elle m'inspire une question : pourquoi ne pas faire davantage confiance au Parlement et aux parlementaires, et c'est une question de temps ou d'agenda médiatique des exemples pourtant que lorsque le gouvernement joue le jeu du travail parlementaire, nous pouvons aller plus vite et faire mieux, je citerai pour cela 3 exemples tirés de la loi climat est résiliant le premier exemple : la réforme du code minier, le 2ème exemple : l'adaptation des territoires littoraux aux changements climatiques et le recul du trait de côte côte 3ème exemple : la création du Bureau d'enquêtes accidents sur les risques naturels, la rédaction de projets de loi autonome pour au moins 2 de ces 3 sujets, nous aurait permis de mieux travailler et de prendre un an de prendre le temps de la discussion avec toutes les parties prenantes, récemment, nous avons encore pu voir l'importance de l'étape de la ratification parlementaire des ordonnances, à l'instar de l'examen du projet de loi ratifiant l'ordonnance relative à l'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises en Alsace, ce qui a permis d'en améliorer si ni Facchetti le contenu à la grande satisfaction des élus alsaciens cette démarche reste trop rare en conclusion, j'insisterai sur 2 points : la nécessité d'une plus grande confiance entre le gouvernement et le Parlement et l'importance de la sérénité du travail parlementaire avec le gouvernement. Merci, Oui, monsieur le président, Monsieur le Président, longeant d'abord vous dire par rapport à ce que vous disiez le l'utilisation des ordonnances, je voudrais rappeler que sous ce quinquennat sauf cas exceptionnel, les demandes d'habilitation ont systématiquement donné lieu à la prise d'une ordonnance. ça vous a un taux de 95 % des habilitations données par le mot, le Parlement, qui ont été utilisées contre 87 % sous le quinquennat précédent et 79 % sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'est juste pour remettent les chiffons en perspective sur la la prise en compte des ordonnances, vous m'interrogez sur l'ordonnance prévue à l'article 83 de la l'homme qui vise à définir les conditions de la prise en charge par l'employeur de certains frais de transport, qui n'a pas été encore publié, je vous précise tout d'abord que cette habilitation expire le 23 avril 2022 puisque, comme vous le savez, le délai de 24 mois a été prolongé de 4 mois, en vertu de l'article 14 de la loi du 23 mars 2020 sur le fond, le plafond d'exonération de cotisations et de charges sociales du forfait mobilité durable avait déjà été relevé à 500 euros dans la loi de finances pour 2021 lors des débats sur la loi climat et résilience les parlementaires l'ont à nouveau relevé à 600 euros en cas de cumul avec le remboursement des transports publics, conformément à l'esprit de la l'homme, il s'agit d'un dispositif facultatif dans la décision et les modalités de versement sont laissés au dialogue social, la mise en place du forfait mobilité durable est récente puisqu'elle date de mai 2021 2020, pardon, les retours d'expériences sont encore insuffisants, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement considère à ce stade, ne pas avoir assez de recul pour décider ou non de rend le dispositif obligatoire dans le secteur privé le la voie privilégiée pour ce forfait reste donc la discussion au sein de l'entreprise ou de la branche, le gouvernement a lancé le 15 février 2021 baromètre forfait mobilité durable afin dresser un 1er : état des lieux du déploiement de ce nouveau dispositif, les premiers résultats publiés en avril 2021 sont encourageants et souligne l'importance d'améliorer la connaissance du dispositif qui aujourd'hui limite son déploiement au sein des entreprises, le gouvernement a ainsi mis en oeuvre, on a un plan d'action incluant notamment des actions de communication pour une large diffusion du forfait Mobilité, un second baromètre a d'ailleurs été lancé enfin une évaluation des accords collectifs, portant sur la thématique des mobilité domicile/travail issu des négociations annuelles obligatoires est prévue par l'article 83 de la cette mission d'évaluation a été confiée à la dame qui la pilote de façon à Pau à à la fois qualitative et quantitative pour une Yves rasions de l'évaluation finale au printemps 2022. La parole est maintenant au président Jean-François Rapin, président de la commission des affaires européennes. Monsieur le président, monsieur, monsieur le Ministre, les ordonnances sont devenus un vecteur privilégié de transposition des directives européennes et de mise en oeuvre des mesures d'application imposée par les règlements européens se sont ainsi succédé des textes de portée générale, faisant une part importante aux directives, la loi pacte où la loi l'homme ou encore des textes destinés à permettre la transposition de textes européens sectorielles dit d'adultes, le recours à des ordonnances en la matière n'est pas nécessairement condamnable dans son principe, en particulier lorsqu'il s'agit de refondre des codes existants pour les mettre en cohérence avec les textes européens, encore faudrait-il que l'objet et les limites de l'habilitation soient clairement définies ainsi, lorsque le texte européen ouvre des options, le législateur est en droit d'être informés des intentions précises du gouvernement à cet égard, avant de l'autoriser à prendre des ordonnances, or si l'étude d'impact du projet de loi signale expose parfois les motifs d'une surtransposition proposer les habilitations sollicité reste quant à elle très imprécise et ne permettent pas de connaître l'usage que le gouvernement envisage de faire des options ou des marges de manoeuvre ouvertes par la directive ou le règlement, concernés depuis janvier 2018, la commission des affaires européennes du Sénat assure une mission de veille sur les surtranspositions de textes européens dans le droit interne avec le souci de ne pas surcharger les acteurs économiques d'obligation qui ne seraient pas imposés à leurs concurrents par le droit européen, les observations qu'elles formule sont fondées sur une analyse de texte européens notamment des options et des marges de manoeuvre qu'ils autorisent et des justifications présentées par le gouvernement, en particulier dans l'étude d'impact à l'appui des transpositions qu'il propose, si elle n'est pas le cas, le rapporteur de la commission des Affaires européennes, attire l'attention de la commission, saisie au fond sur l'existence d'option et l'imprécision de l'Abitibi invitation sollicité dès lors seul un suivi des ordonnances de transposition permet de s'assurer que toute surtransposition est effectivement justifiée au regard d'un intérêt général, dans le respect du cadre européen, or ce suivi est d'autant plus malaisée que la transposition se fait souvent de manière morcelé et échelonnée, il serait donc de bonne méthode que les demandes d'habilitation, soit très précisément documentée sur les intentions de surtransposition et que le Parlement puisse disposer pour toute habilitation a transposé du droit européen de la liste des ordonnances envisagée de leur périmètre et de leur date de publication : je vous remercie. monsieur le président, Monsieur le Président Rapin, hein, je souhaiterais d'abord souligné la qualité du travail. Qui est réalisé par la commission des affaires européennes du Sénat, notamment ceux qui concernent la veille sur les transpositions de textes européens dans le droit interne pour parvenir à maintenir un taux de transposition, le plus élevé possible, le gouvernement a recours à des projets de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, connu sous le nom plus communément répandue de Dadu ses textes comportent un certain nombre de demandes d'habilitation à légiférer par ordonnances et ainsi permettent de traiter efficacement des questions souvent très techniques, tout en laissant aux parlementaires le soin d'apprécier la portée qui donne à la méditation, et s'il le souhaite, de davantage les circonscrire pour exclure certaines disent surtransposition qu'il jugerait indésirables et d'ailleurs, vous l'avez rappelé monsieur le président, en effet, si le Parlement ne peut étend le Champ d'une habilitation, il peut toujours en réduire le Champ et la portée et en ce domaine, on sait et on convient assez volontiers qu'il faut toujours être vigilant, je voudrais également souligner que le gouvernement partage au votre préoccupation et a pris le parti d'éviter autant que faire se peut les surtranspositions, comme en atteste la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de leurs impacts qui précise notamment qu'une vigilance particulière sera portée à la transposition des directives européennes et que toute mesure allant hausse au-delà des exigences minimales de la directive est en principe proscrite les dérogations à ce principe qui peuvent résulter de choix politique suppose la présentation d'un dossier explicitant et justifiant la mesure qui sera soumise à l'arbitrage par ailleurs il est requis dès lors qu'un projet de loi comporte une disposition prise pour la transposition d'une directive européenne de joindre au dossier de saisine du Conseil d'État, un tableau de transposition afin que ce dernier puisse apprécier non seulement l'exactitude de la transposition ponctuelles qui lui est soumise mais aussi sa complétude ces informations se retrouve dans les études d'impact, ce qui doit permettre au Parlement d'apprécier à l'appui du 1er acte de transposition, l'ensemble des textes qui seront nécessaires pour assurer la complète transposition de la directive enfin monsieur le Président, j'ai bien noté vos demandes d'amélioration pour voir l'ensemble des dispositions pour mieux exercer les prérogatives qui sont les vôtres, en particulier sur votre souci vigilant et constant d'éviter les surtranspositions inutiles. Merci, la parole est maintenant aux présidents Vincent Eblé, qui remplace le président Claude Raynal, président de la commission des finances, vous avez la parole. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je souhaiterais faire 2 observations et interrogé le gouvernement sur une ordonnance, la première observation concerne l'unification du recouvrement des taxes et impositions par la DGFIP et la refonte des impositions et amendes le Sénat s'était en effet largement opposée à une habilitation à légiférer par ordonnances au Champ, considéré comme très large aux objectifs peu clairs, nous observons d'abord que plusieurs prolongations de l'habilitation ont été nécessaires et que l'ordonnance vient seulement d'être publié en décembre par ailleurs la codification ne s'est pas faite à droit constant, il revient ainsi au seul gouvernement d'arbitrer sur la codification de certaines interprétations de la doctrine fiscale ou sur les corrections à apporter ou non aux dispositions pouvant méconnaître le droit de de l'Union européenne, ce qui n'est pas satisfaisant, on peut noter que la loi de finances pour 2022 porte une nouvelle habilitation pour un délai, cette fois-ci rallongé de 24 mois afin de prendre des mesures complémentaires, il sera absolument nécessaire qu'un bilan de cette réforme soit présenté au Parlement plutôt que celui-ci en soit totalement dessaisi la deuxième observation concerne la généralisation de la facturation électronique pour les entreprises, le gouvernement a été habilité à légiférer par ordonnances par la loi de finances pour 2021 et celle-ci a été publié le 15 septembre. 2021 dans les délais prévus, toutefois, contrairement à ce qui était indiqué dans l'étude préalable, les délais de mise en oeuvre ont été décalées à 2024 pour les grandes entreprises 2025 pour les établissements de taille intermédiaire

enfin je voudrais interrogé le ministre sur la réforme du régime de responsabilité pécuniaire des comptables publics et la refonte des juridictions financières, il a été proposé de recourir à une ordonnance, dans le cas du projet de loi de finances pour 2022, il s'agit en effet d'une réforme d'ampleur qui devait trouver son application au 1er janvier 2023 ayant fait l'objet d'intenses et longues discussions entre le gouvernement, la DGFIP et la Cour des comptes auraient mérité d'y associer pleinement les parlementaires, le ministre peut-il justifier cette démarche et nous donner des indications sur les échéances de publication de cette ordonnance à laquelle nous serons bien sûr très attentifs. Oui, monsieur le président, Monsieur le Président, mesdames et messieurs les sénateurs, vous vous souvenez, un certain nombre d'interrogations, il y a 2 observations à une question, je commence par les observations. M'avait interrogé sur le choix du gouvernement de demander au Parlement une habilitation à légiférer par voie d'ordonnance pour la génération généralisation, pardon de la facturation électronique pour les entreprises, il s'agit d'un chantier de très grande ampleur qui nécessite des travaux exploratoires de longues années, il a paru nécessaire au gouvernement de ne pas attend la loi de finances pour 2022, et de donner au fond aux entreprises et à tous les acteurs concernés dès 2021, la plus grande visibilité possible pour leur permette de d'assimiler d'anticiper, très en amont, ce mécanisme et de s'y préparer tactiquement, quand bien même celui-ci ne rentreraient que progressivement en vigueur, en fonction de leur taille, entre le 1er juillet 2024 et le 1er juillet 2026, vous m'avez indiqué par ailleurs une fin, une deuxième observation sur le la logique qui concerne la l'unification du recouvrement des taxes et impositions par la DGFIP et la refonte des impositions et amendes par voie d'ordonnance étant donné l'ampleur du chantier qui sera mis en Oeuvres par étapes dans un calendrier se terminant en 2024 par ailleurs cette habilitation permet la codification. De la fiscalité sectorielle numéro 2021 1822 du 22 décembre 2021 satisfait ces 2 objectifs, mais j'ai bien entendu votre demande d'un bilan de ce qui sera fait dans le cas de cette ordonnance enfin concernant l'habilitation pour la réforme du régime de responsabilité pécuniaire des comptables publics et la refonte des juridictions financières, le gouvernement a pris le soin de préciser dès l'habilitation les grandes lignes de la réforme, notamment la suppression de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables, le Champ des justiciables les infractions, les sanctions et l'organisation juridictionnelle comme cela été noté par le Conseil d'État dans son avis sur le PLF pour 2022 cet article d'habilitation particulièrement long et détaillé, répondait à une intention claire de permettre au débat parlementaire, de s'engager sur les points structurant de cette réforme d'une grande complexité d'une grande technicité, compte tenu du nombre de textes à modifier le recours à une ordonnance semblait se justifier, c'est pour ça qu'il a été fait recours le processus consultatif va maintenant être lancé par le gouvernement et le texte devrait être publié au cours du mois de mars, après délibération du conseil des ministres. Merci. La parole est au président François Noël Buffet, président de la commission des lois, monsieur le président. Merci monsieur le président, s'agissant, s'agissant, pardon, des thématiques de la commission des lois, monsieur le ministre, 3 types d'usage des dispositions de l'article 38 de la Constitution m'apparaissent, si ce n'est critiquable en tous les cas discutables, le 1er est celui où le gouvernement n'utilise pas l'habilitation qui l'a demandé, c'est juridiquement naturellement son droit le plus strict mais cela dénote une pratique qui doit être dénoncée, c'est celle de la demande d'habilitation, filet de sécurité que le gouvernement se réserve d'utiliser en cas de besoin c'est oublier d'ailleurs que, constitutionnellement, le Parlement ne peut alors plus se saisir lui-même des matières qui la déléguée et que le gouvernement en multipliant ces habitations bloque en réalité l'action du législateur pour des périodes qui vont parfois jusqu'à 2 ans, exemple récent, le gouvernement a fait voter dans la loi, engagement proximité une habilitation sur le régime des débits de boissons, le délai a expiré en avril 2021 sans que leur donnant cet été prise le gouvernement va-t-il solliciter à nouveau le parlement dans l'affirmative, utilisera-t-il cette habilitation 2ème situation critiquable dans le projet de loi sur l'activité professionnelle indépendante, le ministre des PME d'alors, expliquait sollicité une habilitation je ne qualifierai pas celle-ci, parce qu'il fallait parce qu'il lui fallait du temps pour concerter avec les professionnels et pour décider quoi écrire dans l'ordonnance destinée à modifier les structures d'exercice professionnel libéral, c'est un peu étonnant, et cela même revient à donner un blanc-seing à l'exécutif, ce qui n'est évidemment pas l'esprit de la Constitution, dernier exemple de dévoiement, l'absence de ratification d'ordonnances importante que le gouvernement juge parfois trop technique pour justifier une ratification en bonne et due forme sur ce point, je voudrais vous interroger sur l'ordonnance du 15 septembre dernier 2021 portant modification d'Exposition du livre VI du code de commerce sur les procédures collectives, ce texte apporte des infections particulièrement importante au droit des faillites et exerce où n'exercent pas sur le cas des options ouvertes par les textes européens, il y a matière à discuter de ces choix, le gouvernement entend-il dans ce cas-là, engager la ratification Express de ce texte, pour laquelle d'ailleurs nos collègues ici François Bonhomme et Thani Mohamed Soilihi ont d'ailleurs déposé une PPL de ratification, merci monsieur le ministre. Monsieur le Ministre. monsieur le président, Monsieur le Président, buffet, mesdames et messieurs les sénateurs. Sur 3 points : vous m'avez d'abord interrogé sur la méditation visant à réformer les débits de boisson, prévue par la loi, engagement et proximité effectivement qui n'a pas été prise et pour laquelle le débat d'idées d'habilitation en effet expirer le 26 avril 2021. D'abord rappeler et en préalable que l'Euro gouvernement à peu recours à ce que vous appelez ça pourrait être, s'apparente à parfois à ça à cela parfois à des filets de sécurité puisque, je le rappelais 5 % simplement des habilitations, ne donne pas lieu cette ordonnance visait à rénover le régime du droit des débits de boissons, s'inscrivant dans la continuité des travaux interministériels entamée début 2019 sur l'égide des ministères de la Santé, de l'Intérieur et de la mi-délicat. mi-délicat. 1000 pardon l'application du plan national de mobilisation contre les addictions, il s'agissait de simplifier cette réglementation complexe issu d'une succession de réformes mais également d'encadrer la vente d'alcool pour protéger les mineurs et limiter les consommations à risques toutefois dans le contexte de crise au regard de la situation très particulière dans laquelle elle a placé, reconnaissons-le, les débits de boisson, il n'était pas opportun, il ne vous a pas paru opportun d'intervenir sur les conditions de vente des boissons alcoolisées et de leur dosage en alcool, c'est ce qui a conduit le gouvernement à ne pas se saisir de cette habilitation mais je le rappelle, cette situation est exceptionnel puisque seulement 5 % des habitations ne donne pas lieu à une ordonnance, vous m'interrogez également sur la ratification Express de l'ordonnance du 15 septembre 2021 relatives au livre au livre 6 du code de commerce qui concerne les procédures collectives, selon l'article 196 de la loi 2019, 480 tirer 486 du 22 mai 2019 relatives à la croissance et à la transformation des entreprises, le gouvernement disposait de 4 mois jusqu'au 14 janvier 2022 pour déposer un projet de loi de ratification qui a bien été déposé sur le bureau du Sénat le 5 janvier dernier, le Sénat a également déposé le 16 novembre 2021, une proposition de loi ratifiant modifiant et complétant cette ordonnance, manifestant ainsi sa volonté de se prononcer sur certains importante réforme de notre droit des entreprises en difficulté, force est de constater que ce texte n'est pas encore pu trouver sa place dans l'ordre du jour tant par votre assemblée que par le gouvernement dans ces derniers mois de quinquennat mais évidemment, c'est un sujet qui est devant nous, quant au 3ème, point, je dois avouer que je n'ai pas la réponse mais je vous Fourniret dans les délais les plus rapides, merci. Je vais donner la parole à notre collègue Stéphane Piednoir, vice-président en remplacement de Laurent Lafon, président de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, vous avez la parole monsieur le président. C'est le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, dans le cas de la loi du 29 juillet 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le gouvernement avait obtenu une habilitation extrêmement large lui permettant de déroger, par voie d'ordonnance aux règles en matière de voirie, d'environnement, d'urbanisme et de construction dans le but de faciliter la réalisation des travaux de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le Sénat s'était toujours opposé, estimant d'une part que ces dérogations n'apparaissait pas vraiment utile, et d'autre part qu'elle risquait de faire peser des doutes sur l'exemplarité du chantier de Notre-Dame et de mettre à mal la crédibilité de notre législation en matière de protection du Patrimoine. Alors même que cette habilitation, fut la cause de l'échec de la commission mixte paritaire sur ce texte, le gouvernement n'a finalement jamais pris aucune ordonnance bien sûr le fait qu'il n'ait été donné aucune suite à cette habilitation donne raison a posteriori au Sénat, mais quel dommage, dans ces conditions, que le gouvernement et les députés, six soit arc-boutée au point de passer à côté du consensus et de l'unité nationale que ce drame aurait pourtant dû susciter, comment comprendre que le gouvernement n'est finalement pas fait usage de cette habilitation. Peut-on espérer qu'à l'avenir, sait-on jamais, des efforts soient entrepris pour que les habilitations ne soit sollicitée qu'en cas de réelle nécessitée et avec le chant le plus circonscrit possible, je vous remercie. Oui, monsieur le président, Monsieur le Président, moi vous m'interrogez sur l'habilitation permettant, au gouvernement, mesdames et messieurs les sénateurs, pardon, vous m'interrogez sur l'habilitation permettant au gouvernement de déroger par avoir d'ordonnance. Aux règles en matière de voirie, d'environnement, d'urbanisme et de construction, prise dans le cadre de la loi du 29 juillet 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, cette habilitation avait vocation à faciliter la réalisation dans les meilleurs délais, dans des conditions de sécurité satisfaisantes des opérations de travaux de la cathédrale, en effet, en l'absence d'une définition précise du projet de restauration de la cathédrale, ainsi que des opérations connexes à ces travaux au moment de la discussion du projet de loi au Parlement, et compte tenu du calendrier. Fixé, il est apparu nécessaire et ça rentre sans doute dans la catégorie de ceux qu'il appelle Félix et le filet de sécurité du président Buffet par précaution mais par nature, nous avions besoin de ces précautions d'anticiper des difficultés que nous pourrions éventuellement rencontrer personne ne savait à l'époque, monsieur le sénateur, et je crois que le consensus l'été à l'époque, il n'est toujours aujourd'hui ce que pouvaient être les difficultés ou les contraintes qui pourraient peser sur cette rénovation, compte tenu de la volonté que nous avions tous d'avancer assez rapidement cette habilitation a été circonscrit un certain domaine identifiés au besoin qui pouvait être anticipée le délai expirait le 28 juillet 2020 et il a été prolongé de 4 mois, soit jusqu'au 28 novembre. 2020 dans le contexte particulier que vous connaissez de la crise sanitaire, une seule dérogation a été introduite en application de cette habilitation, il s'agit de l'ordonnance du 18 novembre 2020 dispense sans obligation de compatibilité avec les schémas régionaux des carrières, les décisions d'exploitation de carrières justifiée par les besoins de la les besoins spécifiques de la restauration de Notre-Dame, cette possibilité de dérogation n'a toutefois finalement pas été utilisées, l'établissement public chargé de la conservation et la restauration, venant de passer avec un quartier, un marché de fourniture de Pierre compatible, du point de vue esthétique physico-mécaniques et chimiques avec les pierres d'origine. Quand en place sur voilà la réponse que je voulais vous apporter, il n'était pas possible dans le cadre précis de d'être un peu à peu près complètement certain de des dispositions des dérogations, nous avons besoin, c'est pour ça que nous avions eu recours à l'ordonnance, vous vous féliciter au fond d'avoir eu raison trop tôt, mais parfois on peut aussi se féliciter de prendre des précautions sur des projets qui sont très complexes, et vous le savez aussi bien que moi merci. Merci beaucoup alors maintenant la suite de notre débat, chaque orateur des groupes à 2 minutes maximum, le gouvernement je le ministre a lui aussi une durée équivalente, je donne la parole monsieur Alain Richard pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants, vous avez la parole. Monsieur le président, ce de ce débat est bien sûr bienvenu prend en réalité la suite de débats que nous tenions dans un cercle moins large, plus large, ou alors, je dis bien au titre de l'application de la loi, mais c'est un c'est un progrès, je souhaiterais nuancer quelque peu les observations présentées par la président Gruny quant à la masse des des ordonnances réalisée, la elle a bien sûr souhaité mettre à l'écart les ordonnances prises en 2020 au titre de la santé des des questions de crise sanitaire mais quand elle a fait la comparaison entre quinquennat elle les a réintégrés, or si on les retire, on observe en effet que le nombre d'ordonnances de cette, de ce quinquennat aura été inférieur à celui du quinquennat précédent, donc il me semble qu'on peut voir les choses avec un peu de nuance je souligne aussi les déjà fait sans aucun succès que aujourd'hui il existe un dispositif qui permet de compter les textes non pas simplement pour un texte contre un texte, mais en fonction de leur longueur puisque Legifrance tient un compteur, mot par mot des différents textes et que donc, si on voulait faire une comparaison du poids réel des ordonnances, il pourrait le faire en fonction de leur contenu en droit je voudrais aussi souligner que la comparaison quant à la durée entre la loi et l'ordonnance doit être revu, parce que quand une quand on commence à compter le délai d'une loi si au moment où le projet de loi est déposée devant le Parlement, mais bien évidemment une quantité massive de travaux préparatoires ont été faits avant qui dure en général, plus d'une demi-année fréquemment une année et que des tas de de comment dire de de concertation sont nécessaires avant le projet de loi comme avant la le projet d'ordonnance, mais dans le projet de loi, ils n'ont pas été comptée dans le délai j'en profite d'ailleurs pour souligner que pour une fois, monsieur le Ministre, il y a eu une concertation pendant le cours d'une ordonnance, dans le cas que vous citiez sur le code minier, le tout à l'heure et je pense que c'est très c'est une habitude à prendre ce n'est pas faute de vous de l'avoir déjà demandé. faudra il faudra améliorer les ratifications mais nous savons tous que sur les ordonnances, il y en a 80 ou 90 % dans la ratification se ferait sans débat, donc il faut que nous soyons sélectif et à mon avis, c'est le travail de nos commissions, ce devrait être un débat en bureau de commission de savoir quelles sont les ordonnances du Champ de la commission dont on demande la ratification et on devrait se mettre d'accord avec le gouvernement pour le faire, on législation en commission. Monsieur le ministre. effectivement la difficulté à faire une évaluation à faire une comptabilisation qui soit tout à fait précise point du numérique, mais aussi, parfois, d'un point de vue juridique sans doute cet exercice, monsieur le président, montre à quel point il faut que nous avancions sur ces sujets d'évaluation sur les ordonnances pour avoir des critères qui puissent être partagées entre le secrétariat général du gouvernement, l'Assemblée nationale et Sénat parce que, à ce moment-là on pourra être sur des données et des chiffes qui seront plus précis vous dire effectivement, j'ai bien noté votre remarque sur le code minier parce qu'effectivement, c'est un travail très spécifique qui a été menée qui était assez atypique par rapport à ce que nous faisons d'habitude et 3ème point, alors là, il ne m'appartient pas, évidemment, de m'immiscer dans le choix d'organisation des travaux du Sénat mais en tout cas le gouvernement me semble-t-il, est disposé à réfléchir à la manière dont, sur un certain nombre d'ordonnances, on pense que celles-ci sont prioritaires et justifierait nécessiterait d'un débat, je sais pas ça partage assez le sentiment qu'elle vote, je l'ai dit d'ailleurs dans mon propos liminaire du fait que dans un certain nombre de cas pour la pas dire la très grande majorité des cas, elles ne donneraient pas lieu à des débats qui justifierait peut-être d'être en séance et dans d'autres cas effectivement et justifierait des débats, et ça c'est le travail que nous devons mener ensemble désormais. Parole est notre collègue Alain Marc, pour le groupe, les indépendants, vous avez la parole. le nombre d'ordonnances publiées ne cesse d'augmenter cette tendance se poursuit, même si la bataille des chiffres ne fait pas rage au Sénat, il n'y a aucune qui fasse orageux mais je vous donne un discuter entre 2012 et 2018, il est un fait avéré, leur nombre dépasse celui des lois adoptées selon la procédure ordinaire et cette progression s'est accentuée depuis le début de la crise sanitaire ainsi au cours de la session parlementaire en 2019, 2020, ce sont 100 ordonnance qui ont été publiés, contre 59 durant la session précédente précédente et leur part au sein des textes relevant de la loi s'élève à 70 % nous avons le désagréable sentiment que la loi n'est plus considéré comme le processus normal de législation et par là même que l'exécutif dépossède les parlementaires de leur pouvoir législatif, quelques exemples ont été donnés par notre collègue Pascale Gruny, par exemple sur la haute fonction publique untel recours abusif aux ordonnances je ne reflète pas l'esprit initial de la Constitution de 1958 d'exceptionnel, ce phénomène est désormais devenue habituelle à autre la ratification de la grande majorité des ordonnances s'effectue dans des conditions qui ne donne pas la possibilité aux assemblées parlementaires d'examiner les mesures qu'elles instaurent les projets de loi de ratification des ordonnances sont déposées par l'exécutif afin qu'ils ne soient pas caduques, mais leurs discussions n'est pas inscrite à l'ordre du jour, cela est source d'inquiétude bien légitime par ailleurs accentué par la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel, en effet, dans une décision en date du 28 mai 2020, le Conseil constitutionnel a considéré que si le projet de loi de ratification avait été déposé dans les délais l'ordonnance non ratifiée acquéraient une valeur législative, de façon rétroactive dès la fin du délai d'habilitation, monsieur le Ministre d'inscription à l'ordre du jour des projets de loi de ratification des ordonnances revêtent une importance cruciale pour la démocratie parlementaire, envisagez-vous d'y apporter une vigilance accrue. Oui, monsieur le président Monsieur mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, à la marque, vous m'interrogez sur le taux de ratification des ordonnances et puis sur les décisions du Conseil constitutionnel Vous m'avez interrogé sur le nombre d'ordonnances en particulier faisant référence à la à la session 2019, 2020 reconnaissance dans la session 18 19 2020 nous avons tout le 1er semestre 2020, je ne suis pas sûr que, pardon de vous le dire ainsi, que ce soit la meilleure comparaison que nous ayons quand on sait à quel point dans le printemps 2020 avec le soutien et le concours du Sénat d'ailleurs souvent nous avons dû recourir à des ordonnances parce que là, nous étions face à un impondérable que vous connaissez. Toutes et tous, deuxièmement vous avez fait état de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, en effet, si dans sa décision de la QPC sur la QPC du 28 mai 2020 10 de force 5 le Conseil constitutionnel a semblé assimiler une ordonnance non ratifiée à une disposition législative dès lors que le délai d'habilitation était échu la fait uniquement s'au sens et pour l'application de l'article 61 tirer 1 de la Constitution, c'est-à-dire pour déclarer cette QPC le juge constitutionnel a d'ailleurs eu l'occasion de préciser cela dans une décision du 3 juillet 2020, il a également rappelé qu'une ordonnance qui n'est pas explicitement ratifiée devant le Parlement, demeure un acte réglementaire susceptible de recours devant le juge administratif, cela peut être le cas, notamment lorsque le pouvoir exécutif outrepasse les limites de l'habilitation en aucun cas les prérogatives du Parlement ne sont donc atteinte par cette jurisprudence dont le Conseil d'État considère qu'elle ne modifie en rien son rôle de garant de la conformité de l'ordonnance à la loi de l'habilitation elle permet simplement de transférer au Conseil constitutionnel l'intégralité du contrôle de la conformité des lois et des ordonnances aux droits et libertés fondamentales sur apport de la lisibilité à notre état de droit et garanti au fond une meilleure protection des libertés de nos concitoyens. De l'or, le gouvernement n'a pas considéré que ces décisions devaient avoir un impact sur sa pratique de ratification, j'ai rappelé les éléments de réflexion qui devait être les notes sur les ratifications, partant du constat que s'il fallait ratifier l'ensemble des ordonnances, nous verrions nous pardon de d'ordonnancement de l'Ordre du jour qui serait assez difficile devant nous, mais qu'en revanche nous devions faire un travail avec le Sénat et avec l'Assemblée sur certaines ratification d'ordonnances. La parole est à notre collègue Stéphane Le Rudulier dans le groupe, les républicains. Merci Monsieur le le président, Monsieur le Ministre, je vais être dans la droite ligne de mon collègue Alain Marc, son entrée effectivement dans une bataille de chiffres, on assiste indéniablement une banalisation des ordonnances et l'absence, pour la plupart d'entre elles de la procédure de ratification et ça pose véritablement un problème quant à l'équilibre de nos institutions et surtout la séparation des pouvoirs, un acte émanant du du gouvernement ne saurait être d'une manière ou d'une autre, avoir une une valeur législative, le désistement, le désistement du du Parlement est consacré, que vous l'avez dit, les décisions du Conseil constitutionnel du 28 mai et 3 juillet 2020 pour lequel le Conseil constitutionnel se reconnaît compétent, une fois le délai d'habilitation expiré pour examiner, par la voix de la QPC les dispositions des ordonnances non ratifié intervenant dans le domaine de la loi, ces 2 décisions ont donné le coup de grâce à la protection du Parlement, j'aimerais, si vous le permettez, revenir à la jeunesse de notre constitution, toutes les dispositions portant sur la rationalisation du parlementarisme ont été inscrits avec un postulat le fait qu'il n'y aurait pas de fait majoritaire, c'est donc pour soutenir potentiellement un gouvernement fragile que la rationalisation du parlementarisme, a été mis en place avec le rôle spécifique du Conseil constitutionnel de stabiliser le gouvernement est de permettre au gouvernement en place, de faire adopter ses réformes aujourd'hui l'esprit de la Constitution et pratiquement inversée avec le soutien d'un gouvernement fort et d'un Parlement affaibli alors Monsieur le Ministre, pensez-vous réellement que l'on puisse réformer et gouverner notre pays par ordonnances, alors même que la confiance des Français dans nos institutions et dans notre fonctionnement démocratique s'étiole de plus en plus, ne faut-il pas donner un coup d'arrêt à cette évolution néfaste pour nous a suivi nos institutions et je déplore sincèrement que la PPL sur n'est pas prospérer à l'Assemblée nationale.

merci de votre question, alors, au fond vous poser problème, plusieurs questions : la première, c'est celle qui a été posée sur la question du Conseil constitutionnel, vous l'avez dit, d'ailleurs, elle est dans la prolongation de ce qui a été dit par votre collègue, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit au fond la la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne change pas la méthode et la pratique relatives aux ordonnances et d'ailleurs ça n'est pas la volonté du gouvernement la 2ème chose vous avez dit la banalisation, je crois que c'est le mot que vous avez employé du recours aux ordonnances reconnaissons hors crise Covid même si nous avons pris note, nous devons prendre notre part, si vous me permettez cette expression or crise Covid c'est vrai que le recours aux ordonnances est à est assez important dans les 3 derniers quinquennats et celui-là ne fait pas exception à la règle, je mets de côté la partie crise crise sanitaire la réflexion qu'il faut que nous ayons, me semble-t-il Monsieur le Sénateur, c'est que la la réalité, c'est que nous sommes un pays qui légifère beaucoup que ce soit par voie d'ordonnance ou par voie classique, le projet de loi ou PPL et que c'est, c'est là-dessus, peut-être qu'il faudrait qu'on nous ayons de mener un travail de régulation, je le dis comme ministre des Relations avec le Parlement, j'ai et aussi comme un ancien président groupe à l'Assemblée nationale, ce que j'ai vu les choses et j'ai vu comment les choses se sont passées, peut-être que c'est là-dessus qu'il faut que nous travaillons, j'entends votre vigilance sur le moyen et le véhicule, si vous permettez cette expression qui est utilisée, à savoir l'ordonnance, mais il faut aussi que nous réfléchissions sur un pays qui essaie toujours de régler par la loi, des sujets qui pourraient être réglées de nature différente, et ils ne sont que c'est un mal non pas de cette majorité au ce gouvernement, c'est un mal un peu français, on peut se le dire entre nous. Merci, Monsieur le Ministre, nous donner la parole au président Guillaume Gontard pour le groupe écologiste solidarité territoire, monsieur le président. le Monsieur le Président, je vais poursuivre et et et comme vous nous l'avez un invité rappeler brièvement les chiffres à 345 habilitation par ordonnances ont été accordés sous le quinquennat Macron cela a doublé en 10 ans et c'est peut-être ça qu'il faut, sur lequel il faut appuyer ses ce ce ce doublement sur cette sur cette période et puis la part d'ordonnance ratifiée qui elle est en supplie là 20 % sur le sur le quinquennat qui est aussi quelque chose qui doit nous alerter, vous l'avez rappelé la décision du Conseil constitutionnel du 3 juillet 2020, précisant qu'une ordonnance non ratifiée avait valeur législative est venu jeter le trouble et on peine encore à comprendre cette décision des sages qui entre en conflit avec le 2ème alinéa de l'article 38 de la Constitution, précisant que les ordonnances ne peuvent être ratifiés que de manière expresse, le Conseil d'État conteste explicitement cette jurisprudence et se considère qu'on est compétent pour juger d'une ordonnance non ratifiée c'était également le cas du Sénat et cela a été rappelé, il faut dire que cette décision vient achever de priver le Parlement de son pouvoir législatif, la législation délégué est un mécanisme mis en oeuvre pour faire face à l'instabilité gouvernementale de la IIIe et IVe Républiques et au besoin d'accélération des temps parlementaire avec l'évolution de notre société avec la révolution industrielle et la Montdidier mondialisation quand la constitution d'assassins qui Vème République est venu encadrer cette pratique jamais ses rédacteurs n'imaginez disposer d'une majorité nette et fidèle à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, la conjugaison du fait majoritaire et de la rationalisation du parlementarisme réduisent la représentation de se faire valoir et le prive donc de son rôle de législateur

Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Président, comptable d'abord j'ai. J'avais espéré pouvoir vous convainc dans mon propos précédent sur la question du Conseil constitutionnel pas moi personnellement, je pense que, à plusieurs reprises, il a été indiqué par des millions juriste que la décision du Conseil constitutionnel ne changeait pas fondamentalement la question du recours aux ordonnances. Et la manière dont il devait être appréciée, simplement il était acté que le fait que, en cas de recours et de QPC c'était le Conseil constitutionnel qui s'en saisirait mais que par ailleurs, c'était bien, par la voix qui était habituellement choisis, que les choses se déroulent et l'esprit de la constitution, comme la jurisprudence du Conseil constitutionnel sont clairs sur ce point, le Parlement habilite le gouvernement à légiférer par ordonnances à des fins fins bien précises et dans un Champ déterminé et le Conseil constitutionnel censure comme il l'a fait d'ailleurs l'an passé, à l'occasion de sa décision sur la loi sécurité globale toute rédaction qui permettrait au gouvernement de poursuivent d'autres finalités. Que celles prévues par la loi d'habilitation, on est bien dans l'épure et dans la l'objectif qui était ce sel ce pardon des objectifs qui étaient ceux de la capacité à légiférer par ordonnances 2ème élément, Monsieur le Sénateur, je, pardon de le répéter, mais sur l'ensemble des des ordonnances, je l'ai dit, un grand nom sont liés à la question de la crise sanitaire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un recours important mais il n'y a pas, j'ai essayé le démontrer dans mon propos liminaire d'éléments majoritairement plus grand, plus important dans ce quinquennat que dans les précédents, simplement c'est vrai qu'il y a recours aux ordonnances de manière continue depuis les précédents quinquennats et celui-là ne fait pas exception à la règle 3ème élément sur les ratifications, il me semble que la voie que nous pourrions envisager, ça sera une voie qui permettent d'identifier dans les projets de loi d'habilitation des ordonnances qui nécessiterait un débat sous les formes et moi, il y a les voies et moyens que déciderait le Sénat et l'Assemblée nationale, voilà ce que je voulais vous répond.

mes chers collègues, je crois, et à défaut, à me pour me répéter cela a déjà été dit le recours aux ordonnances a dangereusement augmenté, cela a été dit également : pas moins de 345 habitations depuis 2017, soit une hausse de sensible % par rapport au quinquennat de Nicolas Sarkozy de plus de 6 % par rapport à celui de François Hollande, et seulement en parallèle 20 % ont été ratifiées contre 60 et 80 % pour ses prédécesseurs, j'entends ce que vous venez de répondre à Monsieur le Ministre, mais je crois qu'en dehors du motif Covid et comme l'Europe, pour reprendre les mots du rapport sénatorial, nous sommes toujours à un niveau exceptionnel et finalement l'usage débridé de cet outil, combinée à la récente jurisprudence du Conseil constitutionnel devient forcément inquiétante puisque contre la révision constitutionnelle de 2008, qui impose une ratification Express des ordonnances, les juges ont considéré qu'elles avait valeur législative, passé le délai d'habilitation sans être ratifié exonérant ainsi le gouvernement d'un examen du texte devant le Parlement, hé oui, effectivement, il y a des inquiétudes, mais il y avait des inquiétudes, y compris si l'on reprend un récent article du journal Marianne faisant état du programme d'un futur candidat potentiel, actuellement président de la République, qui visait à dire que l'objectif était de réduire le travail législatif et le temps consacré à l'examen des textes de loi et l'on voit bien là, comment il peut y avoir finalement une possibilité pour l'exécutif de s'engouffrer dans la brèche de l'évitement du débat démocratique en piétinant mais cela a déjà été dit la légitimité du travail parlementaire et finalement en constatant que jour après jour la verticalité du pouvoir se renforce nous Hurion donc connaître la position du gouvernement sur la ratification Express des ordonnances et s'il souhaite aller plus loin dans le transfert du pouvoir législatif vers le pouvoir exécutif, avec un parlement qui décrirait plus la loi. Monsieur le Ministre. le recours aux ordonnances est un recours qui est important depuis les précède le plus aucun ce quinquennat ne fait pas exception à la règle, mais il existe depuis un certain nombre d'années pour des raisons que j'essaie d'expliciter dans mon propos liminaire 2ème sujet la crise Covid a quand même qu'on le veuille ou non produits, il suffit de regarder les textes qui ont été concernés par le recours à l'ordonnance, un certain nombre de textes qui ont été nécessaires dans l'urgence et l'état de crise dans lesquelles nous êtes nous étions la présidente d'ailleurs là l'évoquer, même si nous partageons pas tout à fait les mêmes données mais ça ça participera de l'évaluation, me semble-t-il, que nous ayons, je l'ai dit tout à l'heure, les mêmes données 3ème élément, ce n'est pas un objectif à moyen de contournement du Parlement et je répète la la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne vient pas remettent ceci en cause et là je peux aller dans votre sens, il faut que nous regardions sur les questions de la transposition de la la ratification des ordonnances, les voies et moyens pour voir quels sont les ordonnances qui justifieraient que dans un certain nombre de domaines, il puisse y avoir des débats à l'Assemblée nationale et au Sénat et ça pour le coup, je me sens que c'est là-dessus que nous pourrions avancer et travailler mais je reconnaissons que quand même sur l'ensemble des ordonnances toutes toutes ne se relève pas du même Champ et de la même du même degré d'importance quand on est dans une simple codification ça non, on n'est pas du même degré d'importance que comme nous l'avons fait par exemple sur l'ordonnance des mineurs où là pour le coup, il y a eu un débat d'ailleurs au sénat et à l'Assemblée nationale qui a été je crois un débat de qualité. Merci, la parole est maintenant, madame la présidente, Annick Billon pour le groupe de l'Union centriste. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, notre Haute assemblée est en pointe sur le suivi des ordonnances comme cela a été rappelé la dernière réforme de notre règlement à renforcer le suivi des ordonnances publiées sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, on retrouve ainsi sur le site du Sénat, un tableau de bord détaillé, ainsi qu'une synthèse d'analyse pour chaque trimestre si l'année 2020 a représenté un record absolu en termes de publications d'ordonnance, celui-ci s'explique partiellement par le recours massif aux ordonnances pour répondre aux conséquences de la pandémie de Covid 19 67 % d'entre elles ont été publiées sur ce fondement, bien qu'en recul, le nombre d'ordonnances publiées en 2021 se maintient à un niveau exceptionnel, on voit donc à quel point les récents outils de contrôle introduit par le Sénat sont d'actualité, ils permettent notamment de constater qu'au-delà de la hausse des recours aux ordonnances jamais très satisfaisant pour le parlementaire qui se trouve relégué au rang de spectateur d'un travail législatif hors les murs, il est plus inquiétant de voir chuter le taux de ratification de ces ordonnances, or les statistiques du dernier trimestre 2021 font apparaître que ce taux de ratification est sensiblement plus faible qu'au cours des 2 quinquennats précédents, cela a d'ailleurs été évoquée par notre collègue vice-présidente Pascale Gruny en début de séance, alors Monsieur le Ministre, comment expliquer ce phénomène, cela n'est évidemment pas satisfaisant et pose un vrai problème au Parlement pour rappel, et les chiffres ont été déjà été rappelé pour la session 2019, 2020 environ sans ordonnance avant 2007, il n'y avait que 14 ordonnance publiée par an et, depuis 2017 environ 64 ordonnance publiée par an en moyenne je vous remercie. Monsieur le Ministre, 27 en 2018 57 en 2019 la tendance avant la crise sanitaire se situe donc à un niveau tout à fait comparables est similaire à celui observé lors des précédents quinquennats, même si on peut faire les mêmes remarques au fond sur les précédents quinquennats menotté dans ce niveau c'est en 2020 que 124 ordonnances ont été prises, représentant 38 % des totale des ordonnances prises sous ce quinquennat ça, ce sont les les chiffres au fond que vous avez d'ailleurs rappelé pour une le le sujet que vous avez évoqué des sujets qui doit justifier notre vigilance et c'est d'ailleurs Monsieur le Président, si vous me permettez tout lu toute l'utilité du débat que nous avons aujourd'hui grâce au choix que vous avez fait au Sénat en en modifiant votre règlement d'avoir un débat sur les ordonnances, c'est l'occasion de ratification c'est là-dessus qu'il faut que nous travaillons et ce sont là-dessus que nous entendons travailler gouvernement avec le secrétaire général du gouvernement pour faire en sorte que nous ayons un taux de rectification, avec les précautions ou avec les éléments de diagnostic et d'évaluation qu'il faut avoir sur une ratification qui peuvent justifier d'un débat ou pas sur ces ordonnances à l'Assemblée et au Sénat, c'est vrai que là nous avons un point de vigilance particulier parce que nous constatons que vous là pour le coup, nous sommes conformes sur les questions de chiffre, un taux de ratification qui est faible sur sur le la la partie que nous avons de d'ordonnance, donc voilà là dessus, les éléments que nous sur lequel nous devons travailler Monsieur le Président, pour faire en sorte que cet exercice d'évaluation permettent, je vous rappelle d'ailleurs, comme vous le faites sur le taux d'application des lois d'améliorer le taux de ratification et d'avoir des éléments tangibles et précis d'évaluation sur la ratification au nom de telle ou telle ordonnance. Merci monsieur le ministre. Donner la parole à notre collègue Jean-Yves gros pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen chers collègues. Président, monsieur le Ministre, chers collègues, vous connaissez le peu d'appétit que le groupe RDSE nourris pour le recours aux ordonnances la récente enrichissent prudence du coincé constitutionnel nous rassure par puisque le délai d'habilitation passer des dispositions pourront être regardés comme des dispositions législatives, il existe bien dans une banalisation de l'article 38 de la Constitution, certains y verront le signe d'une utilisation outrancière, j'y vois pour ma part le fait que nous légiférons trop précipitamment au risque que ce que nous votons tombe dans des abysses ou soit potentiellement dévoyés par quelques représentants d'intérêts, ce risque est évidemment majorée lorsque nous arrivons en fin de législature et que les majorités nouvelles n'auront pas forcément pour priorité de les proposer au débat parlementaire janvier 2 questions concrètes : la loi 3 déçu sur laquelle nous avons passé quelques heures de débat qu'on prend beaucoup d'ordonnance depuis la création des EPR pour réaliser des projets d'infrastructures, l'article 9 quater la clarification des compétences, des organismes français solidaire ou à l'article 48 relative au CEREMA et aux conditions de la participation des collectivités territoriales au financement de ces missions de règles relatives à la publique cité foncière je pense aussi à l'amélioration de la prise en charge des conséquences du aux situations de sécheresse ou excusez du peu, l'habilitation pour adapter les dispositions de la loi, un Polynésie française ou en nouvelle Calédonie de même mes chers collègues, nous examinerons la semaine prochaine, le projet de loi portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, 2 articles, le 7 et le 9 prévoit encore des ordonnances de ratification relative à l'assurance contre les aléas climatiques à l'agriculture, ainsi qu'à l'organisation du fonds de secours pour l'Outre-mer, or le dépôt du projet de loi d'habilitation doit intervenir avant 3 mois, est ce bien raisonnable de procéder ainsi, monsieur le ministre, en cette toute fin de législature, quel sort réserve ou à ces ordonnances présentes et futures, qui touche à la vie quotidienne, mais aussi à l'égalité de nos concitoyens de la loi. Oui, monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, où vous m'interrogez sur un certain nombre de la végétation, en particulier les habitations inscrite dans le projet la relatif à la différenciation. La décentralisation et la déconcentration et pour faute en différentes mesures diverses mesures de simplification de l'action publique locale dit projet de loi 3 DS. Je ne ferai pas l'injure de vous dire que ce texte est en cours de finalisation d'examen puisque la commission mixte paritaire qui s'est tenue hier, est parvenu à un accord, ce dont je me félicite, et le gouvernement se félicite le texte devrait désormais définitivement adopté en séance publique au début du mois de février, le projet de loi initial comportait 12 mesures d'habilitation non qui devrait être sensiblement similaire il y a pas eu d'inflation sur ce, je suis là dans le texte issu de la commission mixte paritaire, en outre, depuis le 1er janvier 2022 de loi portent chacune d'une mesure d'habitations ont été adoptées par le Parlement, vous m'avez interrogé en août sur le fait que, il y a un certain nombre de mesures d'habilitation qui arrive en fin de quinquennat pardonnez-moi de vous dire que, d'ailleurs, c'est valable pour les précédents quinquennats autant que je me souvienne, il y avait des mesures d'habilitation dans le quinquennat de de fin de quinquennat du de François Hollande et de même nature sous la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, il ne faut pas comment on pourrait faire grief à un gouvernement au fond à une majorité d'ailleurs à un parlement de coups de se saisir de questions par voie d'habilitation à légiférer par ordonnances, à quelques mois, quelques semaines de l'examen de d'un débat démocratique qui va avoir lieu, auquel cas, sinon nous fiche Orient les positions à partir de je ne sais quel moi d'ailleurs, et nous savons que jusqu'au dernier moment il faut il faut à la fois assumer le travail du gouvernement qui est celui du gouvernement, du Parlement, celui de légiférer et d'habilité éventuellement à légiférer par ordonnances et puis 3ème élément, il y a quand même une forme de continuité républicaine, pardonnez-moi, y compris le travail d'évaluation et d'habilitation et de, de, d'évaluation de la méditation continue à faire le Parlement continue à siéger à l'issue des débats démocratiques peuvent s'interrompt pendant les les moments électoraux et donc il y a une forme de continuité républicaine dont on peut se féliciter si nous devions à chaque fois qu'il y a un an, épisode électoral arrêtez d'habilité à légiférer par ordonnances, je pense que nous aurions un phénomène d'embouteillages de blocage qui serait un peu néfaste, voilà les éléments de réponse que je voulais vous faire.

ne soit jamais en état de débattre d'une réforme aussi importante que la réforme de la haute fonction publique, suppression du corps des préfets, des inspections générales de l'élan notre assemblée, le Sénat a adopté le 6 octobre 2021, une proposition de loi marquant son opposition à la ratification de l'ordonnance qui avait trait à cette réforme, cela s'est traduit par un vote de 225 voix contre la ratification 32 pour, j'ai demandé à Madame, la représentante du gouvernement ce jour-là et j'ai réitéré ma demande quelles conclusions le gouvernement tirer de ce vote n'ayant jamais eu de réponse Monsieur le Ministre, je vous demande quelles conclusions vous tirer de ce vote du Sénat, ceci est assorti d'une 2ème question, monsieur le président, lors de sa séance du 4 novembre 2021, le Sénat a adopté par 322 voix pour et 22 contre une loi constitutionnelle garantissant le respect des principes de la démocratie représentative et de l'état de droit, en cas de législation par ordonnances devant ce vote massif 322 voix pour tous 22 contre, j'ai demandé à Madame, la représentante du gouvernement cherché que la fonction publique, quelles conclusions le gouvernement tirer de ce vote massif du Sénat, elle n'a articulé aucune réponse j'ai réitéré la question, je n'ai toujours pas eu de réponse donc ma 2ème question est clair, monsieur le président, Monsieur le Ministre quelles conclusions tire le gouvernement de ce vote. Monsieur le ministre. Monsieur monsieur sur Monsieur le sénateur sur vous avez parlé à la fois. De la haute fonction publique, de la ratification de l'ordonnance sur la haute fonction publique et 2ème élément d'une loi qui a été votée, loi constitutionnelle votée au Sénat sur la question des ordonnances sur le 1er point, vous me permettrez de rappeler que vous êtes saisis vous-même de cette question par la voix d'une PPL si j'ai bonne mémoire, qui elle-même n'a pas fait l'objet d'un accord de ratification puisque je crois qu'au Sénat il y avait pas d'accord entre les différentes parties prenantes qui a fait le ce qui a fait que cette PPL a été rejetée par tient pas discuter de cette voie qui a été choisi qui était évidemment tout à fait dans les prérogatives du CSA, du Sénat, de se saisir de la ratification d'une ordonnance, permettez que le gouvernement est à la fois accepter le

sur le 2ème point, reconnaissons que nous sommes dans un débat qui est un débat qui fait partie du Champ démocratique, il ne m'a pas échappé que nous sommes à un moment particulier de la vie politique qui s'est vu du moment joyeux des élections et du moment du débat électoral, qui est un débat qui est tout à fait sain il appartiendra à chacun de faire des propositions pour améliorer les voies et moyens du travail parlementaire, ce sont des débats constitutionnels je rappelle d'ailleurs que nous avions initié une loi constitutionnelle pour faire un certain nombre d'évolutions et qu'elle aurait peut-être trouvé là aussi une voix et moyens malheureusement on n'a pas pu aller jusqu'au bout, mais c'est vrai que c'est des questions qui sont devant nous cette me semble-t-il, si vous me permettez cette remarque un peu plus compliqué que ce qu'on dit parce qu'on voit bien qu'on aurait de toute façon, un sujet d'ordre du jour parlementaire s'il s'il s'avérait que toutes les habilitations faisait l'objet d'une ratification en séance comme c'est comme vous le souhaitez, au fond, et donc on a quand même besoin, me semble-t-il, par la pratique monsieur sur nous on him sans que nous avons besoin, par la pratique, sans forcément passer par une loi, et là c'est dans le dialogue avec le gouvernement, il faut que le gouvernement porte lui-même une exigence d'ailleurs dans ce domaine-là, je n'ai pas dit autre chose en cette fin d'après-midi que cette exigence que nous devons avoir monsieur le Président, de faire en sorte que sur la question des ordonnances, nous améliorions les choses, je ne suis pas sûr que nous ayons là encore besoin d'une loi pour ajouter à la loi des choses qui pourraient simplement relevé de la bonne pratique et du dialogue sain et démocratique entre les assemblées, c'est plutôt ça que j'que j'appelle à faire entre les assemblées et le gouvernement, quel qu'il soit. Bien, merci Monsieur le Ministre, merci, mes chers collègues, pour ce 1er débat sur les ordonnances, je ne sais pas s'il faut une loi Monsieur le Ministre, mais en tous les cas, il faut que dans les manières dont nous. Tenons les relations entre exécutif et Parlement le Parlement soit respectée, qu'il puisse débattre qu'ils puissent échanger, vous avez dit, pardonnez-moi, c'est inhabituel qu'un président de séance près de la parole, mais comme président du Sénat je suis extrêmement attentif à ce que les droits du Parlement soit respecté, je pense que il y a des progrès de part et d'autre à faire, et. Nous en porterons aussi notre part et je dois dire que je remercie encore une fois, le groupe de travail et sa présidente, de nous avoir fait cette proposition et que nous ayons pu le le mettre en oeuvre. Il faudra en tirer, nous semble-t-il des enseignements que ce ne soit pas simplement un débat qui s'inscrirait dans une forme de liturgie mais qui s'inscrivent dans une exigence de progrès pour la qualité de la législation et j'allais dire le rôle de la démocratie représentative, je vous remercie les uns les autres je vais maintenant lever la séance, qui va être reprise à 21 heures 30 pour le débat sur les conclusions du rapport mieux protéger notre Patrimoine scientifique et nos libertés académiques, la séance est suspendue.